La séance est ouverte, le compte rendu intégral de la séance du jeudi 1er février a été publié sur le site internet du Sénat : il n'y a pas d'observation, je n'en vois pas le procès-verbal est donc adopté. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a été publié cette candidature sera ratifié si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. informé le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité est parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2000 Et dans la discussion générale, la parole est à Madame, Laura Flessel Ministre des Sports. Monsieur Monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires culturelles, madame la sénatrice Muriel Jordan messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, le sport mis au service du rayonnement de notre pays de notre territoire, du développement économique et social, telle est l'enjeu de l'accueil de jeux olympiques et paralympiques en France, cette édition des Jeux qui reviennent sur notre sol en 2024 et notre victoire à tous. Elle est une chance pour notre pays, je ne suis pas sûr, je ne suis pas indifférente aux réserves que ce projet a pu sauter dans certains pays tentés par l'organisation des Jeux, je ne suis pas non plus indifférente à la nécessité de poursuivre le travail de mobilisation auprès de nos compatriotes au cours de ces 6 ans qui viennent, je le suis d'autant moins que je ne suis pas là en tant que ministre des Jeux olympiques et paralympiques je suis la ministre des Sports de toutes les pratiquantes et de tous les pratiquants et je n'ai jamais conçu ce projet autrement que comme un vecteur inespéré pour développer la pratique du sport dans notre pays, l'intérêt de ce jeu, c'est l'héritage que nous pouvons construire ensemble autour d'eux dans une France fatigués par des années de crise, l'accueil des grands événements sportifs internationaux tels que les Jeux, la guéguerre l'Euro féminin de hand ball la Ryder Cup, la Coupe du monde féminine de football ou la Coupe du monde masculine de rugby est une nouvelle démonstration de notre capacité à construire notre destin commun à travers le sport pour cela nous devons saisir notre chance, montrer la voie et préparer l'avenir, le gouvernement auquel j'appartiens, s'inscrit dans cette approche, parce que nous concevons l'accueil de jeu comme un levier qui nous permettra de mieux faire vivre les multiples fonctions du sport dans notre société. Au terme d'une phase de candidature qui aura réuni athlètes mouvement sportif partenaire économique acteurs publics et de la société civile, nous nous préparons déjà pour une nouvelle aventure en persévérant, cette unité. Nous avons s'étant un peu moins de 7 ans pour livrer le je voulais réussir et en faire un moteur de transformation d'innovation sociale, il ne fait pas de doute qu'ils seront un accélérateur d'investissements, un atout pour le rayonnement de notre pays, un facteur de développement pour les territoires, néanmoins je construis mon action ministérielle pour qu'il soit pas que cela, car nous souhaitons que ces Jeux soient un levier au service de la cohésion sociale qu'il renforce le destin national et européen de la France en contribuant à mettre un mouvement, un mouvement sa société 7 territoire qu'il puisse nous permettre de faire du sport, un outil au coeur et au service de la société que la sobriété et l'intégrité de l'art et la responsabilité, les caractérisent. Nous lèverons les bras après avoir franchi la ligne, mais nous avons pris un bon départ depuis le 13 septembre 2 nous sommes mis en ordre de marche afin de respecter nos engagements un délégué interministériel aux Jeux, a été nommé Jean Castex, la société de livraison des Jeux olympiques, Nicolas Ferrand et la comité et le comité d'organisation des Jeux, présidée par un artisan essentiel à notre victoire, Tony Estanguet, ont été créés et sont déjà au travail. Un projet de loi olympique et paralympique vous est aujourd'hui présenté dans le but de répondre à nos engagements, moins de 6 mois après l'attribution des Jeux à notre pays. Vous savez, cette loi olympique et paralympique est une procédure classique, qui n'est pas propre à la France mais qui s'applique à tous les pays organisateurs des Jeux. Il faut la percevoir comme une nouvelle Pierre à l'édifice que nous sommes tous en train de construire, elle vise 3 objectifs principaux respecter nos engagements et les garanties apportées à l'État en face de candidature. De livrer les Jeux dans les temps en respectant le budget. certains de nos jeux d'âge intègre et exemplaire, c'est d'ailleurs tout l'objet du titre IV dédié à la transparence et à l'intégrité, une section du texte introduite à l'initiative de la France. Parce que la transparence et l'intégrité nous protège. Parce que les Français allaient le réclament, à juste titre et que je pense personnellement qu'il s'agit de conditions gagnantes pour s'inscrire à la réussite de ce que le projet dans ce projet et parce que nous partageons cette ambition collective de fixer de nouveaux de nouveaux standards pour les futures éditions d'âge. Voilà donc l'objet de ce projet de loi que je vous présente aujourd'hui avec mon collègue qui arrivera tout à l'heure, Julien Denormandie, secrétaire d'État. Auprès du ministre de la cohésion des territoires qui vous prie de l'excuser de son absence à l'occasion de sa discussion générale en raison de problèmes de transport, je tiens à remercier sincèrement les rapporteurs, les commissaires et l'ensemble des sénateurs qui ont travaillé dans un esprit de construction sur ce texte, un texte qui n'est clair qu'une partie minuscule, minuscule de l'incroyable événement que j'ai moi-même eu la chance de vivre en tant que sportive et qui dépasse très largement les quelques semaines de compétition qui se tiendront sur notre sol en 2024 par ailleurs, je sais que certains passionnés de sport parmi vous ont été frustrés par un texte technique qui nous offrent trop peu d'occasions de rappeler tout ce que le sport apporte à notre société cette frustration, je la comprends et je la partage, car là est bien notre ambition qu'à travers ce jeu qu'au delà même de ce jeu, nous puissions promouvoir le sport, ses valeurs et ses vertus parce que le sport m'a tant apporté, je ne me résous pas à ce que certains de mes concitoyens de la pratique jamais, je pense notamment aux jeunes dans certains quartiers ou territoires ruraux carencé. Aux femmes qui sachent trop souvent de pratiquer à l'adolescence ou après la naissance d'un enfant aux personnes en situation de handicap pour tous ces Français, nous devons penser autrement la pratique sportive, nous devons être innovant et volontaire, je sais ce qui préoccupe les élus de terrain que vous êtes et le territoire que vous représentez. Par-delà les médailles par delà l'événement notre enjeu de saisir l'opportunité qui nous offrent ce jeu pour que ce pour que toute la France et tous ces territoires en bénéficient, certains d'entre vous m'ont d'ailleurs alerté sur leur volonté de voir les Jeux diffusée en clair à la télévision, c'est une préoccupation tout à fait légitime et que je partage, c'est d'ailleurs dans ce but, pour que chaque Français puisse avoir à nos jeunes que je rencontre fréquemment les acteurs de l'audiovisuel afin que les négociations en cours intègre cet impératif, par ailleurs, ça je ce sont ceux de toute la France, je tiens à mentionner le grand programme de labélisation des sites de préparation de délégations étrangères qui sera lancé dès l'été 2018 par le comité d'organisation des Jeux à travers un appel d'offres ouvert à toutes les collectivités territoriales. à travers ce programme chaque territoire pourra faire valoir ses atouts touristiques économiques et sportifs et faire postuler pour recevoir des sportifs du monde entier, je le répète : au-delà des Jeux, rappelons-nous que développer le sport pour tous, celui du quotidien, surtout les-t-il territoire c'est bien cela notre ambition commune la tâche à laquelle je Mattel Mattel chaque jour dans 6 ans à l'extension de de la flamme sur le Stade de France, nous n'aurons réussi nos innove que si davantage de Français pratiquent une activité physique et sportive en 2024 que si chacun d'entre nous parvient demain partout en France, à trouver une offre sportive qui correspond à ses amphis et ses besoins, c'est d'ailleurs à cette dans cette optique que j'ai décidé. Que 50 pourcent des crédits du CNDS serait dès cette année, orienter directement vers les territoires carencées qu'il s'agisse de quartiers prioritaires de la ville de la de la ville, où des zones de revitalisation rurale, ensemble, nous devons donner plus à ceux qui ont moins et c'est cela notre enjeu et notre défi et mon engagement. Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est dans la sobriété que résidera la force du projet olympique et paralympique, c'est dans la transparence et l'exemplarité que nous le construirons c'est avec l'esprit que le sport doit changer le quotidien de tous les Français que nous le définiront je terminerai en disant que ces je dépasse les frontières et les clivages, ils sont le signe d'une France à la fois unie et ouverte sur le monde, ils seront un événement qui rassemble, créateur de commun qui mobilisera toutes les forces vives de la nation, la France d'un jeu, c'est une France qui gagne et qui rayonnent une France hier. à l'image ne sportifs qui ont déjà décollé pour la Corée du Sud et se prépare à briller sur les pistes et les patinoires des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver montrons l'exemple l'unité de l'ambition et de l'enthousiasme, je vous remercie. Merci madame la ministre, la parole est à mal à Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes. minutes. Le président, Madame la Ministre, chers collègues, vous l'avez rappelé la France va accueillir l'été 2024 les Jeux olympiques et paralympiques, nous avons été choisis le 13 septembre dernier à Lima. Quand je dis la France, il s'agit essentiellement de Paris de la Seine-Saint-Denis également de vous le savez de la la ville de Marseille, le projet de loi, nous allons examiner, a pour objectif pour objet de permettre la réussite de ces Jeux, je dirais, d'emblée, la commission des lois à travailler dans cette esprit à adhérer à l'objectif de ce projet de loi et effectivement s'est révélé majoritairement, très majoritairement favorables à ce que nous puissions réussir les Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, puisque c'est l'image de la France dans le monde, qui sera en réalité. Les Les défis à relever ne sont pas minces, j'ai pu m'en convaincre avec plusieurs de mes collègues lors des près de 90 auditions auxquelles nous avons procédé lors également du déplacement, nous avons pu faire en Seine-Saint-Denis ces ces enjeux ces défis, je dirais qu'ils sont, ils sont de 3 ordres : tout d'abord, il va falloir accueillir une manifestation sportive d'une ampleur inédite, nous n'avons jamais en France, accueilli untel événements sportifs, quand bien même, hé bien un championnat du monde de football a pu être accueilli il y a quelques années, 37 sites de compétitions 15000 athlètes 20000 journalistes 70000 bénévoles 11 millions de spectateurs qui sont prévues, je rappellerai précisément au bout du championnat de du monde de football 2,9 millions de billets avaient été vendus, ce qui permet de mettre en perspective, ce que nous attendons par rapport à ce que nous avons déjà vécu, nous devons donc être à la hauteur de cet enjeu de cet enjeu face à cette manifestation sportive d'ampleur inédite. Le 2ème défi nous avons à relever le 2ème enjeu, on en a peu parlé et nous en parlerons peut aujourd'hui également, et la maîtrise des coûts financiers un désintérêt de la candidature de la ville de Paris, a été le fait que des infrastructures étaient presque toutes construites et que l'investissement financier n'était pas très important. Pour autant, tout est relatif, il est tout de même de 6 milliards et 8 3 milliards 8 pour l'organisation, pourcent 3 milliards 7 doivent provenir normalement de de fonds privés et 100 millions doivent provenir de fonds publics mais sont entièrement dédié aux Jeux paralympiques. 3 milliards 8, donc, d'organisation, il nous reste 3 milliards pour les infrastructures qui seront à parité, financé par des fonds privés et par des fonds publics, chacun a en mémoire les dérives financières qu'ont connu toutes les villes qui ont organisé les Jeux olympiques, il est impératif que la France ne se fout, pourquoi pas, dans ses errements budgétaires qui ont pu exister et que nous continuons à maîtriser le coût qui était prévu initialement. Le 3ème enjeu. Je dirais qu'on peut le le dénommé sous vocable d'héritage, on parle beaucoup d'héritage ce que ça signifie en réalité que ce que nous attendons, et que les Jeux olympiques et paralympiques ne passe pas sur, sur la France comme un un grand vent d'enthousiasme sportif pendant quelques semaines et puis s'étioler disparaissent dès lors que la cérémonie de clôture aura eu lieu. Alors c'est un héritage, mais c'est un héritage que nous attendons dès maintenant vous l'indiqué la ministre, il faut que le sport soit mis à l'honneur pendant ces Olympiades met également en avant, il faut que toute la France souhaite impliquer la mobilisation de tout un pays, ça passe par 2 choses : ça n'est pas exhaustif mais par il y a pas de culturel tout d'abord l'Olympiade culturelle va se dérouler de 2020 à 2024 et de nombreuses manifestations sont prévues en nombres de son événement sur toute la France et pas seulement sur les sites olympiques de n'attire culturel et puis ça passe aussi, vous l'avez évoqué la ministre par les bases arrières, ce à quoi, évidemment, le Sénat est particulièrement attentif les bases arrière sont les sites sur lesquels s'entraîneront les déviations étrangères qui seront mis à leur disposition un cahier des charges va être établi, chacun dans sa collectivité pourra au regard des des moyens dont ils disposent bien candidaté pour accueillir ces délégations, ça me paraît extrêmement important que la France entière profite aussi de ces Jeux olympiques et paralympiques et soient mobilisés pour ça. L'héritage, ce sont aussi les infrastructures indiqué tout à l'heure, nous avons peu d'infrastructures à construire, puisque 95 pourcent des infrastructures existent déjà sur le territoire, il en reste néanmoins quelques unes, ce sont le stade 2 à Paris, un stade de 8000 places, le centre aquatique de la peine en Seine-Saint-Denis, le village olympique et paralympique en Seine-Saint-Denis également et le village des médias aussi en Seine-Saint-Denis, il est important évidemment que ces équipements ne soit pas ce qu'on a qualifié habituellement des éléphants blancs, c'est-à-dire des équipements qui reste déshérités après le passage des Jeux olympiques et paralympiques, on en a eu quelques exemples sur les jeux passés et il est essentiel, je dirais, à la fois pour le CIO et pour la France, que cela ne se reproduise pas, alors ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, nous savons ce qu'ils vont devenir la reine a 2 étaient déjà prévus par la Ville de Paris, c'est donc un équipement qui avait déjà une vocation avant celle des Jeux olympiques et paralympiques le centre aquatique restera un centre aquatique, bien évidemment, et sera prise en main par la métropole dans sa gestion du Grand Paris et le village olympique et paralympique, ainsi que le village des médias s'inscrivent dans des projets qui étaient déjà si je puis permettre dans les cartons des élus locaux qui ont ont été très associé à leur conception et ils deviendront des habitations, des logements sociaux en est pas des bureaux, des commerces, ils auront en tout cas une vocation postérieurement, et il est essentiel qu'elle était prévue antérieurement à la mise en oeuvre de ces constructions et aux prévisions des Jeux olympiques, je dirais que, paradoxalement, la façon dont nous traiterons l'héritage, c'est-à-dire ce qui se passera après les Jeux, hé bien sera un succès, une garantie de succès et de réussite pour les Jeux olympiques et par la Turquie se déroule tout cela sera mis en musique par de nombreux acteurs, je ne peux pas tous les citer, puisqu'en réalité il y a 14 organismes différents qui vont intervenir et de nombreuses collectivités locales et acteurs publics. Les 3 acteurs essentiels qui se dégagent sont le comité olympique pour les Jeux olympiques et paralympiques, une association loi 1901 le co-Joop qui va se charger de l'organisation des Jeux, la Solideo qui est la société de livraison des équipements olympiques qui va donc assurer la maîtrise d'ouvrage d'un certain nombre d'équipements mais également la coordination des maîtrises d'ouvrage, il n'y aura pas moins de 27 mètres d'ouvrages sur ces constructions, même si elles sont peu nombreuses, donc il est essentiel que un Epic, en l'occurrence un organisme coordonne l'intégralité des maîtrises d'ouvrage et puis le délégué interministériel, bien sûr, je vous olympiques et paralympiques qu'on appelle autrement plus communément le job, dont je ne vous explique pas la fonction qui découlent de son nom. C'est brosser à grands traits le contexte dans lequel intervient ce projet de loi, vous l'avez rappelé la ministre, 3 objectifs : d'abord mettre en oeuvre les engagements de la France, engagement pris dans ce qu'on appelle le contrat de ville hôte le contrat qui a été signé entre le CIO, le comité national olympique et sportif français, et la ville de Paris dès lors que la candidature a été validée, c'est ce contrat de ville hôte, c'est également le dossier de candidature, c'est également les 74 lettre d'engagement du gouvernement qui doivent être honorés par ce projet de loi. Le 2ème objet c'est celui qui nous a pu particulièrement occupé à la commission des lois, et l'introduction d'une série de dérogations au droit de l'urbanisme pour permettre de réaliser en temps et en heure, les équipements, les quelques équipements dont nous avons besoin. C'est un point qui peut, qui peut laisser perplexe doit dire car effectivement, il s'écoule environ 7 ans entre le moment où le choix est fait, et le moment où les Jeux olympiques se dérouleront. Il peut paraître assez extraordinaire que nous n'est pas nous n'ont pas le temps, en 7 ans de construire finalement aussi peu du type je crois que ça doit nous interroger et ça nous interroge certainement sur l'état de notre droit, et le fait qu'il est aujourd'hui dévoyé le droit et normalement un outil au service de nos projets et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, le droit est un frein et que la seule façon que nous trouvions de réaliser ses équipements dans les temps étant alité, de réduire et de d'alléger le poids des procédures qui pèse pèse sur nous et je reprendrais les propos de monsieur le ministre, Normandie nous indiquait. Qu'il fallait se libérée de ses carcans procéduraux, je crois que c'est extrêmement important et ça doit nous alerter sur l'état de notre droit, si nous n'étions pas des Cette cette dérogation, nous l'étudierons tout à l'heure, enfin le dernier point, les derniers objectifs de ce projet de loi a été effectivement de garantir l'éthique et l'exemplarité, notamment par l'intervention d'un certain nombre d'organismes que nous connaissons déjà très bien, la Cour des comptes, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et autres organismes destinés à gérer cette éthique. C'est donc sur ce projet que nous avons travaillé, la commission des lois, mais également la commission, la culture, la commission des affaires économiques et la commission du développement durable. La commission je voulais indiquer, a été majoritairement favorables à ce projet de loi mais là pour autant amendé dans le sens d'une plus grande efficacité, notamment un certain nombre de précisions ont été apportées sur le périmètre du projet de loi, nous avons également eu égard à un site de compétition qui avait été, je peux dire, dans le projet de loi initiale qui est la scène puisqu'il y aura des épreuves dans la Seine, et il a été prévu que le raccordement des établissements flottants au système des eaux usées se fasse de façon à ce que la scène faisant un bon état d'usage lorsque les nageurs ils plongeront et enfin, et j'en finirai par cela, la modification qui me paraît la plus importante est-ce que je qualifierais d'héritage paralympiques. Il y a finalement peu de choses dans ce projet de loi sur les Jeux paralympiques et sur la façon dont les personnes handicapées peuvent accéder à ces jeux, y compris en tant que spectateur. La commission des lois a estimé qu'il était nécessaire d'étendre l'allégement des procédures à la possibilité de mettre aux normes les stations du métro historique parisien pour que il y a un accès aux personnes handicapées aux personnes à mobilité réduite à ces jeux, il faut savoir qu'il y a 3 pourcent du métro historique qui était aujourd'hui accessible et ce faisant. Nous ne réaliserons peut-être pas l'intégralité de la mise aux normes, mais d'où la facilitons tous cas et c'est extrêmement important, c'est donc dans cet esprit positif que la commission a travaillé et je pense que c'est également cet esprit positif qui nous animera tout le long des débats, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Alain Châtillon, en remplacement de Madame Sophie Primas, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques pour 5 minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord excusez Sophie Primas, qui est malheureusement empêché cet après-midi et je me dois de la remplacer pour la commission économique, la France va à nouveau accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, cet événement est un enjeu majeur pour l'image de notre pays mais aussi pour notre économie et notre territoire l'impact économique et touristique des Jeux est loin d'être négligeable pour notre pays en 1000000 de spectateurs, du moins c'est ce que nous pensons sont attendus des retombées économiques sont estimées à au moins 10 milliards d'euros et 250000 emplois créés à cette occasion la commission des loi nous a délégué l'examen au fond pour l'article 12 et 13 relatives au logement.

à l'urbanisme, le projet de loi n'a pas vocation à légiférer de manière générale, en matière d'urbanisme, pas plus que de chaude mais uniquement de prévoir des dérogations ou droit droit commun indispensable pour faciliter la livraison des trois tout lecture nécessaire au jeu dans les délais impartis. Les articles 7 8 et 10 bis vise spécifiquement à accélérer ou sécuriser les procédures d'aménagement ou d'autorisation, article 7 permet de dispenser de formalités au titre du code de l'urbanisme et les constructions et aménagements temporaires nécessaires au l'article 8 prévoit qu'une opération d'aménagement ou une construction nécessaires à l'organisation et au déroulement des Jeux pourraient être réalisé, selon la procédure intégrée pour le logement, enfin, l'article 10 bis permettent aux permis de construire d'autoriser des constructions nécessaires au mais également d'autoriser le changement de destination de ces constructions après les Jeux, lorsque la destination ultérieure et comme ce qui ce qui réalise la construction des bâtiments après les Jeux et leur affectation à notre usage comme le logement par examen L'article 10 donne aux collectivités, la faculté de fusion et de libération de création de la ZAC et la libération de réalisation, il reprend une disposition issue de la proposition de loi portant, accélération des procédures et stabilisation du droit d'urbanisme droit d'urbanisme, bien sûr, de la construction de l'aménagement de nos collèges François Calvet et Marc Denis, adopté par le Sénat en 2016, la commission des affaires économiques, a émis un avis favorable à l'adoption de ces 4 articles sans proposer de leur apporter quelque modification que cela soit janvier dans un article 12 et 13 relatives au logement. Les locaux du village des médias. Et des villages olympique construit en Seine-Saint-Denis, dans les Bouches-du-Rhône ont conçue pour s'inscrire une fois les Jeux terminés dans le titre urbain des villes dans lesquelles ils sont situés, ils pourraient devenir des logements logements sociaux des logements privés, des bureaux, etc, l'article 12 du projet de loi donne la possibilité aux organismes HLM de construire et d'acquérir des locaux situés en Seine-Saint-Denis et dans les Bouches-du-Rhône et de les mettre temporairement à la disposition auprès du commerce comité olympique pendant la durée de ces Jeux avec leur transformation en logements à usage locatif. Les conditions d'utilisation de ces locaux pendant les jeux sont incompatibles avec les dispositions relatives aux conditions de mise en logements prévus dans les conventions, l'article 12 prévoit donc de suspendre les effets de la convention APL attaché à ce logement pendant bien sûr la durée de cette mise à disposition. La Commission a proposé de déroger à titre temporaire pour ses locaux au règlement des chapitres 1 et 2 du titre du livre IV du code de la construction et de l'habitation qui sont relatifs aux conditions d'attribution au plafond de ressources et au loyer par ailleurs des logements destinés à des étudiants vacants au 1er juillet 2024 et situé en Île-de-France, dans cette maritime des Bouches-du-Rhône agiront de la Haute-Garonne, mais également la Loire la Loire Atlantique, le Nord et le Rhône, pourrait être également loué jusqu'au lendemain de la clôture des Jeux olympiques et paralympiques pour accueillir les personnes accréditées, les effets des conventions APL attachés à ces logements seront suspendus en application de l'article 13 le temps de cette mise à disposition, ici aussi, la Commission a proposé de déroger aux règles du livre IV du code de la construction préciser sous réserve de l'adoption de ces modifications, la commission a émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi merci. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, on a intervention portera sur 3 points spécifiques de ce projet de loi, projet de loi qui a fait l'objet d'un avis favorable de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication, la commission a tout d'abord cherché à créer les conditions les plus favorables au succès des Jeux olympiques et paralympiques, dans le respect des engagements pris par la France, ainsi nous avons en particulier travailler en lien étroit avec le comité d'organisation locaux jobs pour sécuriser juridiquement les propriétaires olympique, c'est-à-dire l'ensemble des signes et terme distinctif qui pourront être valorisés auprès des partenaires privés, ce travail devrait permettre de rassurer le CIO sur la capacité de la France à générer les ressources nécessaires à l'organisation de jeu qui je vous le rappelle, ne pèse pèseront que très peu sur les finances publiques parce je rappelle que les ressources des partenariats représentent probablement un tiers du budget prévisionnel, le 2ème sujet concerné traite à la fois de la publicité et du respect du Patrimoine parisien, j'ai conscience du fait que la publicité est un sujet sensible, il est d'autant plus que les Jeux de Paris se dérouleront pour partie au coeur même de la capitale à l'intérieur ou à proximité de plusieurs de ses joyaux patrimoniaux le nous a garanti que l'écu bâtiment serait respecté l'attrait des jeux de Paris perte perdrait à ce que le Patrimoine de la ville, disparaissent sous des bannières commerciales en tous genre, c'est un point sur lequel je crois utile de clamer notre attention attachement et d'indiquer que nous nous y resterons vigilants, que nous sommes liés par des engagements souscrits dans le cadre du contrat, le contrat de ville hôte et que les revenus tirés de cet affichage publicitaire sont absolument nécessaires pour garantir l'équilibre financier des Jeux que nous jugeons tous essentiels, enfin les prévisions du COJO affiche que 13 millions de billets seront vendus mais que 4 milliards de téléspectateurs sont attendus : l'accès aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 se fera donc prioritairement à travers la télévision, or les droits télé ont été cédées au groupe américain Discovery qui aimerait beaucoup pouvoir vendre certaines épreuves à la demande sur sa plateforme au lieu de les diffuser en clair, le CIO n'avait sans doute pas anticipé l'évolution des usages et des modèles économiques lorsqu'il a vendu les droits des JO de 2024, il n'a pas été possible de renforcer dans la loi, l'obligation de diffusion en clair, pour des raisons de recevabilité financière mais on peut regretter que cette situation prive les Français de l'accès à de nombreuses épreuves, la question qui est posée aujourd'hui et cette question est fondamentale concerne donc la capacité de France Télévisions a acheté ces droits et nous souhaitons que l'État intègre cette dépense dans l'évolution des finances et des missions confiées au groupe public de télévision mais et quand même Tony Estanguet, la lui-même signalé souligné pardon lors de son audition devant la commission de la culture, il est primordial que les Français puissent s'approprier les Jeux pour cela nous devons répondre à 2 questions: la première concerne les conditions de réception des épreuves seront-elles majoritairement accessible en clair, c'est là un sujet sur lequel je le sais et vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, vous travaillez, la seconde est celle des conditions de diffusion dans les lieux publics et plus particulièrement lors d'installation d'écrans dans ces lieux publics pour que chacun puisse bénéficier des images et partager ces moments forts, je note que le diffuseur des dernières Coupes du monde de football ou bien des matchs de la Coupe du monde de rugby en 2015 avait explicitement prévu la gratuité pour de telles diffusion sous réserve naturellement du respect de quelques conditions cette question mérite mérite donc que l'on s'y attarde, j'espère avoir fait passer un message auprès de Madame la Ministre, voir auprès des diffuseurs Compte-tenu de ces remarques notre commission a estimé que ce projet de loi était indispensable à l'organisation des Jeux olympiques, enfin, à quelques heures de l'ouverture des JO d'hiver, souhaitons que nos portiques sportifs français se couvre d'or, je vous remercie.

Monsieur le Président, Madame la ministre Madame la rapporteur de la commission des lois, mesdames et messieurs les rapporteurs pour avis mais, chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du Développement Durable s'est réuni pour avis du projet de loi que nous examinons aujourd'hui après l'ajout en séance à l'Assemblée nationale de 4 articles relatifs au transport, la commission a examiné ces articles au fond et c'est également saisi pour avis de l'article 6 sur l'allégement des procédures de participation du public, la Commission considère que ces articles très techniques permettent de sécuriser de projets d'infrastructures stratégiques d'une part. La liaison Charles-de-Gaulle Express qui permettra aux passagers aériens de se rendre à Paris quotidiennement en moins de 20 minutes et, d'autre part, le Grand Paris Express qui vise le prolongement de la ligne 14 du métro et la création de 4 nouvelles lignes de métro automatique pour un total de 200 kilomètres de voies nouvelles dans ce contexte, elle proposé d'adopter ces articles car ils ne font que tirer les conséquences de choix antérieur, il ne s'agit plus aujourd'hui bien évidemment de mettre en cause l'opportunité de ces projets, mais bien de laisser pour assurer leur livraison pour les Jeux de 2024, du moins l'espère en nous, il serait en effet regrettable pour la France de ne pas tenir ses engagements, engagements qu'elle a souscrits dans son dossier de candidature à cet égard, Madame la Ministre, lors de l'examen du projet de loi au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement, nous avons été un certain nombre, la crainte que la réalisation du Grand Paris Express soit compromise, ce qui nuirait évidemment au bon déroulement des Jeux, ces craintes ont été suscités par le récent rapport de la Cour des comptes sur la Société du Grand Paris qui fait état d'une dérive importante dans la gestion du calendrier de livraison des infrastructures. Prévu et surtout d'un dérapage financier extravagant de l'ordre de 12 milliards d'euros en 4 ans, alors je me réjouis, Madame la Ministre, que nous puissions évoquer ces sujets avec vous aujourd'hui vous connaissez l'attente des élus franciliens concernant le Grand Paris Express qui doit renforcer, vous le savez la cohésion territoriale et sociale de la métropole le 1er ministre mène actuellement des consultations sur ce sujet et devrait annoncer le Refah sage prochain du Grand Paris Express d'ores et déjà Madame la ministre des Transports, a fait part aux élus franciliens par un courrier du 30 janvier de ça, volonté de définir un calendrier réaliste pour les Jeux et de mettre en place, 3 groupes de travail pour réfléchir au calendrier du projet à sa soutenabilité financière et aux moyens de compensation ou de substitution à mettre en place en cas de décalage des projets dans le temps, j'attire votre attention à cet égard, sur le fait qu'il serait peu opportun évidemment de ne pas réaliser la ligne 17 jusqu'au Bourget, Exposition, puisque c'est le le siège du village des médias, je doute que les journalistes du monde entier qui viendront dans notre pays, goûte le plaisir de ne pas pouvoir rejoint directement et le plus simplement possible les sites de compétition depuis leur lieu de résidence temporaire, surtout quand on connaît les problèmes récurrents du RER B et la mauvaise image qu'ont nos concitoyens des voies réservées aux Jeux sur des axes comme là où la 3 qui sont d'ores et déjà totalement saturé. Pourriez-vous, madame la ministre, à cette occasion, nous donner des précisions supplémentaires sur ce front, et au-delà sur le calendrier du Refah sage, pour la réalisation des sites des Jeux, elle a présenté un amendement qui a d'ailleurs été adoptés par la commission des lois et qui renforce la participation du public en prévoyant simplement que les réponses du maître d'ouvrage observations formulées soit obligatoire et non pas facultative, cette disposition rendra plus effective, la participation de du public qui découle d'une exigence de niveau constitutionnel pour finir notre commission de l'aménagement du territoire sera particulièrement attentive à la prise en compte de l'objectif d'accessibilité universelle des transports dans le cadre des Jeux, il en va, bien sûr, de l'image de notre pays et de sa capacité d'intégration sous le bénéfice de ses observations, la commission a donc proposé d'adopter les articles dont elle s'est saisie, je vous remercie. Merci, cher collègue madame la milice, mes chers collègues, je vous indique que je suspendre notre séance à 16 heures 15 au plus tard afin de permettre la réunion de la conférence des présidences celui prévu à 16 heures 20 conférence des présidents, qui sera suivie d'une série de questions d'actualité au gouvernement dans la suite de la discussion générale, la parole est à la Mireille Jouve pour le groupe RDSE et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, 100 ans après les huitièmes eux Olympiade de l'ère moderne, la France s'apprête à accueillir de nouveaux pour leur 33ème édition, les Jeux olympiques, pour ce faire la ville de Paris, a signé avec le comité international olympique, un contrat de ville hôte dont nous débattons aujourd'hui de la traduction législative, compte tenu des engagements déjà acté la marge de manoeuvre du législateur s'en trouve réduit très à sa portion congrue, je débuterais mon propos en insistant sur le fait que la réussite et l'équipe des jeux de Paris 2024 sont aussi importants pour la France que pour le CIO, en effet, avec la double attribution des Jeux à Paris et à Los-Angeles, nous avons tous des tous pu constater que que les candidatures pour l'organisation des JO ne sont plus légion cette raréfaction et notamment le fait des excès tout particulièrement budgétaire qu'on pu connaître de nombreuses olympiades qui conduisent certains décideurs publics à s'en détourner, gardons également à l'esprit que lorsque certaines villes candidates consulte préalablement leur population sur l'opportunité de telles candidatures, c'est généralement un refus qui se dégage, majoritairement des urnes comme à Münich ou Hambourg, la France et le CIO doivent donc conjointement redoubler de vigilance pour que ces olympiades soit exemplaire dans leur préparation et leur déroulement, le principal atout du dossier français réside dans l'existence de la grande majorité des infrastructures infrastructures dédiées : seul le centre aquatique qui verra le jour au sein de la commune de Saint-Denis est une salle multi-et une stalle multisports de 8000 places dont l'implantation est envisagée dans le nord de la capitale demeure à faire sortir de terre s'y ajouteront pour les principales installations la construction du village olympique du village des médias et de plusieurs équipements temporaires et je n'oublie évidemment pas en tant qu'élu des Bouches-du-Rhône que Marseille sera, elle aussi, ville olympique Anne accueillant les compétitions de voile et de football, s'il ne représente pas une garantie en lui-même, cet élément devrait jouer un rôle essentiel dans la maîtrise du budget de ces nouvelles Olympiades française un budget qui devra être largement abondé par les partenaires commerciaux du CIO avec la levée dans un périmètre de 500 mètres autour des sites olympiques des interdictions d'affichage publicitaire, si notre groupe peut regretter l'étendue de cette levée d'interdiction et l'ampleur de la marchandisation donc faire l'objet, ce type d'événements sportifs, bien loin des valeurs qu'il est censé véhiculer, il est toutefois conscient de l'importance de limiter le recours aux fonds publics notre afin de respecter les délais de livraison des vraies d'infrastructures, des mesures de simplification et de limitation de la consultation du public seront également exceptionnellement institué. La double consultation sera remplacée par une procédure de participation par voie électronique, là encore, les élus RDS sont conscients des impératifs qui Sam poste à nous pour l'organisation d'une telle manifestation sportive nous saluons l'amendement introduit par la commission du développement durable, prévoyant que la synthèse de la consultation mentionne tout de même, les réponses aux observations et participation du public, il conviendra également afin d'avoir une évaluation sincère du coût financier supporté par la collectivité pour l'organisation de ces olympiades de prendre pleinement en compte la mobilisation de nos forces de sécurité si aucun d'entre nous n'est aujourd'hui à même d'évaluer la mesure terroriste qui planera toujours sur la France à l'horizon 2024, nous savons d'ores et déjà que la mobilisation sera d'une très forte ampleur. Si ces gens sont porteurs d'obligations, ils n'en sont pas moins également une opportunité pour nos territoires et leurs habitants, il est prévu que la Solideo, qui livrera les infrastructures des Jeux se dote d'une charte fixant ses obligations et celle de ses prestataires en termes d'emplois, de personnes en situation d'insertion ces obligations seront étendues aux travaux de réaménagement du site grâce à un amendement de la commission des lois pour l'élaboration de cette charte, il sera sans doute utile de s'appuyer sur les collectivités territoriales concernées et tout particulièrement sur celles qui oeuvrent le plus largement en matière d'insertion, les bases avancées pour la préparation des athlètes représenteront aussi l'opportunité de mobiliser tous nos territoires dans la réussite de ces Jeux, elles étaient au nombre de 500 lors des Olympiades de Londres des outils adaptés devront permettre de faciliter les démarches entreprises par les collectivités, qui souhaiterait accueillir des délégations d'athlètes l'adhésion populaire à s'était vainement pourrait également être favorisée par l'autorisation faite aux collectivités territoriales de pouvoir retransmettre gratuitement certaines épreuves sur écrans géants, comme l'a rappelé tout à l'heure notre rapporteur Claude Kern, l'adhésion populaire passera aussi il n'élude inéluctablement par le respect d'un certain nombre de critères éthiques dans l'organisation, comme dans le déroulement de ces Jeux, tout d'abord, dans le respect des valeurs du sport et dans la lutte contre le dopage dans les prochaines lois de finance au respect des engagements pris par le gouvernement pour sortir le laboratoire de Châtenay-Malabry encore référence mondiale il y a 2 décennies de la très mauvaise passe dans laquelle se trouve aujourd'hui au-delà des athlètes celles et ceux qui porteront dans les 6 prochaines années, ces Jeux devront également être partie prenante de cette exigence de transparence, les organisateurs à travers le projet devront établir une déclaration d'intérêts et de Patrimoine auprès de la HATVP, l'encadrement des rémunérations n'étant pas envisageable pour une structure comme le colloque comme certains d'entre nous répulsion été nous satisferont de la proposition faite par la commission des lois, d'un rapport annuel mais, chers collègues, à Paris comme à Marseille, en Seine-Saint-Denis, comme dans l'ensemble des territoires qui souhaiteront s'associer à telle cette aide vainement les Français auront à coeur de démontrer leur capacité à organiser un événement qui, selon Pierre de Coubertin, constitue une fête quadriennal de la jeunesse universel du printemps humain, sommes toutes, toutes et tous ici convaincu des vertus du sport Nelson-Mandela relevait à juste titre que le sport a le pouvoir de changer le monde, le pouvoir d'inspirer le pouvoir d'unir les parce que comme les responsables politiques ne saurait le faire le sport peut créer l'exploit, c'est un instrument de paix, le groupe RDSE pardon votera donc ce texte qui nous est proposé. qui gagne, la parole est à monsieur Dominique Théophile pour le groupe, la République en marche pour 6 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'interviens aujourd'hui sur un projet de loi qui symbolise la persévérance de la France, puisque l'organisation des Jeux olympiques, lui a été accordé après que les postulé en vain 98 2008 et 2012, cette victoire est le fruit d'un investissement sans précédent de la part des différents acteurs, que je remercie chaleureusement d'abord évidemment des sportifs qui ont soutenu la candidature de la France, et bien sûr Teddy Riner ambassadeurs de Paris 2024 Ryad Salem et tous les autres, je citerai ensuite les fédérations, les membres du CIO tels que Guy doute médaillé d'or au 110 mètres au JO de Montréal en 76, sans oublier, madame la ministre des sports qui est présente aujourd'hui, enfin, nous devons remercier les citoyens français qui ont fait montre d'un soutien sans faille pour ce projet ambitieux, en préambule, je souhaiterais rappeler les mots de Pierre de Coubertin, instigateur des Jeux olympiques et défenseur des valeurs que la France a déjà porté il y a un siècle de cela lors des Jeux organisés à Paris en 1924 et disait que le soir, on va chercher la peur pour la dominer la fatigue pour en triompher la difficulté pour la vaincre ainsi pour que les Jeux olympiques et paralympiques puisse être organisé, conformément à la charte olympique et au contrat de ville hôte, le projet de loi visant à garantir les bonnes conditions des JO de 2024 marque une nouvelle étape de l'engagement de la France comme pays organisateur, ce projet est d'autant plus important que les Jeux olympiques et paralympiques ont des retombées touristiques et économiques bénéfiques pour notre pays 11 millions de spectateurs sont attendus du monde entier, 250000 emplois pourraient être créés si le budget des Jeux olympiques et paralympiques 2024 c'est lève à 6 milliards d'euros, l'impact économique pourrait quant à lui, dépasser les 10 milliards les Jeux olympiques représentent également un accélérateur d'investissements qui vont accompagner la transformation des territoires, que ce soit pour la Ville de Paris, la région d'Île-de-France je pense plus particulièrement à la Seine-Saint-Denis ou encore la ville de Marseille et plus généralement à l'ensemble des collectivités concernées, les jeux sont le moyen pour la France de valoriser son Patrimoine et son savoir-faire sur la scène internationale. Bien plus que ces jeux sont les garants d'un été un héritage mis au service des populations en Seine-Saint-Denis par exemple le centre aquatique, qui doit être construit à l'occasion de cet événement sportif accueillera ensuite les habitants de ce département, qui bénéficieront des meilleures conditions pour s'entraîner et développer leurs compétences en natation mais venons-en au fond du texte, chers collègues, ce dernier se structure autour de 4 axes majeurs : d'abord autour du respect des dispositions du contrat de ville hôte conclue entre la Ville de Paris, le CNO Seif et le CIO ensuite autour de l'adaptation et de la simplification de certaines règles et procédures d'urbanisme en 3ème lieu il traite de la sécurité des Jeux et de la question des transports, en effet, la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques est assurée par la création devra réservé aux déplacements des délégations des athlètes aussi empruntée par les véhicules de secours et de sécurité, enfin il prend toutes les dispositions qui garantissent une organisation irréprochable dès juin matière de transparence et d'intégrité à cet effet, des mesures sont prévues pour renforcer la lutte contre le dopage fléaux qui nuit à l'idéal sportif ainsi l'article 15 du titre 4 concernant les dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité prévoit que le gouvernement peut prendre, par ordonnances dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi toute l'aide toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques nécessite l'adaptation de certaines règles prévues par le code de l'environnement, notamment en matière de publicité ainsi et pour la durée des Jeux jusqu'à 15 jours après la cérémonie de clôture des monuments historiques ou des sites classés pour accueillir des panneaux publicitaires, cette dérogation se justifie, d'une part par la nécessité de donner une visibilité au juges mais aussi par le fait que les mesures de publicité n'auront aucun caractère transitoire et non définitif, par ailleurs, seuls les logements étudiants vacants des régions organisatrices au 1er juillet 2024 pourront être loués à titre dérogatoire au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, cette décision est encore une fois marquée du sceau du respect des citoyens français, vous l'aurez compris ce projet de loi relatif à l'organisation des Olympiques et Paralympiques est un texte à la hauteur du défi qu'a accepté de relever notre pays la France. Tout en facilitant et en sécurisant l'organisation des Jeux, il place au coeur de sa problématique, les valeurs sportives qui seront défendus par nos athlètes, l'éthique, la transparence et les écoute de la voix de chacun sont les garants du bon déroulement de cet événement planétaire. Ce ne sont donc pas seulement les jeux de Paris ils sont organisés par le présent projet de loi mais les jeux de tous les Français et de tous les territoires, en conclusion, nous souhaitons que les valeurs de l'olympisme, apporte une nouvelle vigueur à ceux qui font notre nation la fraternité en l'état, le groupe la République en marche votera donc ce texte. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre Legrand pour le groupe communiste républicain et citoyen, écologie et pour 6 minutes. Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons et l'acte législatif nécessaire la conséquence logique de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous soutenons l'esprit du projet mis en oeuvre telle qu'il a été rappelé lors de son audition au Sénat par le président du COJO Tony Estanguet, nous serons attaché à faire de ces Jeux, une réussite populaire est une chance pour le développement du sport pour tous, pour l'essentiel, le projet de loi consacre le contrat entre le CIO et la ville haute, nous le voterons donc en dépit de certaines dispositions qui font notamment la part un peu trop belle à la protection des sponsors, vous savez qu'au-delà de la candidature de Paris nous plaidons d'ailleurs Marie-George Buffet l'a rappelé récemment pour un processus d'attribution des Jeux plus transparent, plus éthique, plus démocratique, avec la création d'une agence internationale d'attribution des grands événements sportifs à l'image de ce qui a été obtenu pour la lutte antidopage, les scandales ayant éclaboussé certaines éditions seraient ainsi mieux prévenus et nous nous félicitons que Paris 2024 veille à se prémunir de ces dérives avec des dispositions sociales, éthiques et environnementales, renforcer l'adoption de ce projet de loi appelle toutefois de de notre part enfin brève remarque je veux exposer la première concerne l'héritage attendue des Jeux en matière de développement de la pratique sportive pour tous, vous annoncez, madame la ministre, une autre ambition : plus 3 plus de 3 millions de licenciés, mais pour être tenu cet engagement en appelle d'autres, en matière de moyens d'équipements de sport scolaire et universitaire de rattrapage des inégalités d'accès à la pratique sportive de promotion du sport féminin du handisport du sport dans les quartiers populaires et aussi du sport dans les entreprises,

Le manque d'infrastructures sportives et réelle sur le territoire, en métropole comme en outre-mer, les inégalités frappent les quartiers populaires, alors même qu'ils sont les plus jeunes héros probablement les plus gros potentiel en maths et en matière de développement des pratiques. Les choix budgétaires opérées par votre gouvernement pour 2018 baisse des dotations collectivités territoriales à la vie associative recul massif des contrats aidés fragilisation démission du CNDF sont à contresens de l'ambition espérer, voilà pourquoi nous souhaitons que le projet de loi inscrivent l'amende l'engagement de procéder au travail de diagnostic nécessaires visant la préparation et le lancement à l'Automne prochain d'un plan de programmation pluriannuel en faveur du sport. La seconde remarque concerne les transports, le réseau du Grand Paris Express et tant d'un point fort de 2024, il est aussi un des points forts de l'héritage espérer des jeux pour les transports du quotidien en Île-de-France, nous attendons des garanties sur le respect du calendrier de ces engagements, nous sommes vigilants sur ce point, en revanche, nous ne comprenons pas les articles introduits dans la loi à l'Assemblée nationale, semble-t-il, à la demande du gouvernement sur la ligne privée Charles-de-Gaulle Express cette ligne contesté et coûteuse qui risque de se réaliser au détriment des investissements et décisions nécessaires au Grand Paris Express ne figure d'ailleurs pas dans le dossier de candidature de Paris 2024 elle n'a donc rien à faire dans cette loi olympique la 3ème remarque concerne la Charte sociale Paris 2024, c'est là aussi une originalité de la candidature de Paris, Bernard Thibault, qui représente les 6 organisations syndicales françaises à l'OIT, on a été chargé, il va d'ailleurs siégé au COJO et à la Solideo, la charte sociale et validé par le COJO par toutes les organisations syndicales et par les organisations d'employeurs, nous proposons que son existence et son nécessaire respect figure dans la loi. Cette question qui concerne les emplois créés pendant les travaux de préparation et la durée des Jeux ne saurait être confondue avec la 4ème question que je veux, brièvement évoquée, celle du bénévolat, la célébration populaire appelé de ses voeux par le Cujo nécessite la mobilisation de dizaines de milliers de bénévoles, il faut donc la charte prévu dans le projet de loi aborde précisément le recours aux volontaires olympiques enfin 5ème et dernière question, la retransmission télévisée des Jeux, à l'heure actuelle, rien ne garantit que les chaînes en clair, notamment le service public puisse diffuser les épreuves aussi largement qu'elle le faisait jusqu'ici. Un accès dégradée pour les téléspectateurs de notre pays serait tout de même un incroyable paradoxe. Et pourrait même gâché en partie la fête et sa célébration populaire nous proposions de sécuriser les diffusions collective et populaire organisée autour des Jeux par les associations sportives et les collectivités territoriale en les exonérant du paiement des droits nous ne comprenons pas pourquoi ces amendements ont été jugés hier recevable au titre de l'article 40 qui n'a strictement rien à voir avec le problème posé par ailleurs sur ce point, nous demandons au gouvernement et j'ai entendu ce que vous aviez dit tout, vous avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, au gouvernement de s'engager directement dans la discussion avec les chaînes françaises, on organise en quelque sorte une équipe de France de l'audiovisuel, pilotée par le service public pour garantir l'accès des téléspectateurs à l'événement et pour faire face à la négociation des droits ensemble plutôt que de laisser faire une concurrence qui pourrait s'avérer meurtrière dans le contexte de surenchère se pratiquera le doute Discovery voilà, Madame la Ministre, les remarques que nous voulions portée avec l'objectif qui est le notre seul objectif, la promotion des valeurs olympiques et du sport pour tous et qui conduiront la majorité, la quasi-totalité à par une voix du groupe CRCE à soutenir cette loi tout en tentant de la compléter, merci. Merci, la parole est à madame Marie-Pierre de La Gontrie, pour le groupe socialiste et républicain, vous disposez de 5 minutes chers collègues. Monsieur le président. Madame la ministre. Madame les rapport. Peur et messieurs les rapporteurs pour avis mais, chers collègues, je suis très, très heureuse et assez fière de pouvoir m'exprimer au nom de mon groupe aujourd'hui pour ce qui est et nous l'avons constaté depuis le début de cette discussion générale un sujet qui nous rassemble et qui finalement ont que parfois en France même, au Parlement, nous sommes capables de porter des sujets ensemble, y compris de quinquennat au quinquennat du président de la République un président de la République, puisque ce projet a été initiée d'abord a été initiée d'abord par François Hollande. Et y compris avec Patrick Kanner, que j'ai plaisir à saluer ici évidemment. Très bien repris ensuite. Repris ensuite par le président de la République, Emmanuel Macron et vous Madame la Ministre, et bien sûr le permettrait de noter l'extraordinaire ténacité de la maire de Paris, Anne Hidalgo qui s'est dépensé sans compter et finalement la victoire a été là le 13 septembre alors aujourd'hui c'est une étape un peu technique, nous l'avons dit nous parlons assez peu de de sport dans cette hémicycle mais nous posons une Pierre supplémentaire de ce qui doit être ce projet. Si encore une fois, doit trouver dans ce projet de loi des facilités techniques mais, pour autant qu'il ne doit pas permettent de perdre de vue nos ambitions pour les Jeux olympiques, qui ne doivent pas se limiter, même si c'est important à la fierté au rayonnement international, à la grande mobilisation des sportifs et des athlètes au moment de cette pour les Français mais aussi porter un certain nombre de valeurs qui ont été évoqués tout à l'heure et se préoccuper de l'héritage qui sera laissé ensuite aux Français, alors nous savons ça été rappelé par plusieurs de mes collègues, c'est d'abord, techniquement, un produit un un méthode d'accélérateur de transformation urbaine, nous le savons, grâce au projet de transport qui ont été évoqués tout à l'heure, nous savons grâce au projet d'aménagement, même si notre coup la collègue Murray journal a rappelé à juste titre la particularité de ce projet étant que des équipements existe effectivement la transformation et parfois ma radicale que celle que nous avons pu connaître dans d'autres pays, c'est aussi un outil de transition écologique j'ai reviendra tout à l'heure est aussi un outil d'inclusion sociale, lorsqu'on est attentif aux valeurs on doit y compris dans ce projet de loi se guider pour les suivre sur la question de la transparence de l'éthique de la sobriété, la sobriété a été évoqué tout à l'heure, puisque ce projet sera moins coûteux que d'autres, la transparence et l'éthique, nous l'avons vu dans le texte des amendements viendront sur les contrôles de la Cour des comptes, la prévention des conflits d'intérêts et les auditeurs divers concernant l'enjeu territorial et social des clauses sociales ont effectivement été introduites les retombées pour les PME et pour l'activité économique du périmètre géographique sont importants, la question, madame la ministre du Grand Paris Express qui a déjà été évoquée est une question extrêmement puisque nous avons entendu qu'il était possible, envisageable, peut-être à tort, que le projet soit séquencé et que finalement une partie de l'Île-de-France n'en bénéficie pas tout de suite, c'est un sujet de préoccupation, mais aussi la question du bénévolat, qui a été évoqué tout à l'heure où la question très importante que vous pouvez résoudre de l'accès à la retransmission des associations, des petites collectivités qui n'auront pas les moyens de les financer et enfin l'enjeu écologique je remercie notre collègue Muriel Jorda d'avoir appelé la question importante du raccordement des péniches de manière à ce que nous puissions réaliser à Paris le voeux de Jacques Chirac, nous pourrons bientôt nous baigner dans la Seine et donc cette épreuve en eau libre, qui doit se tenir au pied de la Tour Eiffel nécessite que les bateaux figurant sur le fleuve soit raccordé au réseau des eaux usées, et donc il a été accepté en commission que cela devienne une obligation, c'est important, y compris au terme de l'héritage puisque nous pourrons ensuite c'est très important, continuez de nous dans la Seine, donc vous l'avez compris on peut avec des valeurs qui sont parfois différencié selon les, les, les, les grands et les bancs de cet hémicycle trouver néanmoins des convergences pour soutenir ce projet, un dernier mot, Madame la Ministre, sur les Jeux paralympiques, c'est vrai que on en parle moins, à tort, même si effectivement ces jeux permettent à tous nos concitoyens de de prendre conscience de l'extraordinaire, comment dire, performances des athlètes dans ce domaine et puis au gré d'un projet de loi effectivement pouvoir adapter une partie du métro en Île-de-France aux personnes en situation de handicap, c'est très important, vous l'avez compris le groupe socialiste se réserve de quelques amendements qui ont été déposées, un avis favorable sur ce projet de loi et nous espérons que l'esprit des jours à continuer de traverser ces bon. La parole est à monsieur d'animateur pour le groupe, les indépendants pour 3 minutes.

Depuis l'annonce des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, la presse se fait écho d'une France impatiente et le monde politique à Paris en pleine effusion.

Certes, les organisateurs ont promis de faire le pari de la sobriété, avec un financement assuré réaliste de 3 milliards d'euros chacun. Pour autant, faut-il croire en ses paroles et annonce rassurante. Après je olympiques de Londres en 2012, le gouvernement britannique avait dû plancher sur une belle feuille de route financière afin de gérer les surcoûts et les coûts imprévus de sur la fracture sportive. Le comité olympique Paris 24, se veut rassurant : voilà rappelé 95 pourcent d'infrastructures existent ou seront temporaires, seul le village olympique et médias ainsi que 100 aquatique et l'Arena 2 devront être très de toute pièce. Ce constat semble Colette aussi le coût d'infrastructure, notamment liée aux transports, en effet, la Cité de la Société du Grand Paris est d'ores et déjà mis en cause principalement par le risque de dérapage budgétaire.

Un point évoqué important : la sécurité, avec plus de 11 millions de feu Vert attendu les jeunes 24 sera un événement plus populaire que la Coupe du monde 98 et que l'Euro 2016 dans un contexte de risque élevé et permanent, la protection de nos compatriotes et les touristes devra être une priorité. Nous saluons sur ce point, législatives prises dans ce projet de loi pour assurer la suite de toute toutefois ne cédons pas enthousiasme notre rôle de parlementaire et de porter un regard vigilant sur l'occasion de ces jeux événement ce que nous ferons les dominants scrupuleusement ce projet de loi que nous vous soumettons, elle se propose essayé d'amendements que ma collègue Colette Merlot mélo ou présentera non mélo, excusez-moi, mais j'étais un peu dans le Var.

Merci, la parole est à monsieur Michel Savin, pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Monsieur le président de la commission madame. Et messieurs les rapporteur chers collègues. Je suis très heureux que notre assemblée étudie cet après-midi le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le Sénat, par la voix de son président s'y est déclaré favorable dès les débuts du projet. Et nous n'avons jamais manqué l'occasion de soutenir le comité de candidature. Ce fut notamment le cas avec un engagement écrit de la part de la quasi-totalité des présidents de groupe de notre haute assemblée. Aujourd'hui, le Sénat est pleinement investi aux côtés du comité d'organisation. Notre commission de la culture, a auditionné les différents acteurs de la candidature. Nous les avons aussi reçu dans le cadre du Groupe d'études que je préside et l'ensemble des sénateurs a montré son intérêt pour ce projet aux multiples facettes. Sportive évidemment culturel mais aussi sociétal, environnemental touristique diplomatiques et bien d'autres. Le 13 septembre dernier, nous avons donc renouer avec l'olympisme, 100 ans après avoir accueilli nous derniers Jeux d'été. Notre fierté est immense mais la tâche qui nous incombe le sera tout autant. Nous devrons accueillir le monde et ce dans les meilleures conditions. Ces Jeux de 2024 seront aussi des jeux charnière dans l'histoire olympique. Nous voyons bien que très peu de villes malheureusement se portent candidates. à cause des Budgets qui explose. Des dérives parfois importantes sur l'environnement de la mauvaise gestion des infrastructures et trop souvent de la folie des grandeurs de certains pays organisateur. Tous ces enjeux doivent d'être pensé et réfléchi. Nous devons renouer avec la base de l'de l'histoire olympique avec son essence même, pour proposer des Jeux à taille humaine, profitant à l'ensemble de la population. Nous connaissons l'implication le professionnalisme des équipes du comité d'organisation des colonnes olympiques et paralympiques aussi nous sommes très optimistes sur le la maîtrise du projet ainsi que son bénéfice pour l'ensemble des Français. Madame la Ministre, aujourd'hui, les rapports avec les territoires, leur implication constitue un enjeu : un enjeu primordial pour l'organisation de nos jours. L'ensemble de la génération 2008 devra-t-être au coeur des dispositifs et ces Jeux seront un formidable moyen d'accélérer et de renforcer la pratique sur nos territoires, ainsi que de soutenir et développer les infrastructures, seul le volet héritage de ce projet. La semaine olympique et paralympique qui s'achève est un excellent signal du dynamisme en faveur des jeunes. Ces objectifs partagés avec tous les territoires, et tous les citoyens sont pleinement porté par les organisateurs, le gouvernement et le Parlement. Et je suis certain qu'ensemble, nous parviendrons à offrir à chaque Française et chaque Français une part du Rav olympique. Le Sénat prendra toute sa part dans cette entreprise et nous sommes d'ores et déjà impliqué dans la mise en place de différents projets. Mes chers collègues, le projet de loi que nous étudions ce jour extrêmement important pour l'organisation même des jeux, il est de notre devoir de l'adopter afin de permettre, organisation dans la durée des prêts très restreinte de cette année qui nous sépare de l'événement. Les débats sont nombreuses et passionné sur certains points, que ce soit ici au sein du Sénat ou à l'Assemblée nationale. Mais je suis sûr que nous saurons trouver des accords sur tous ces sujets, ce qui permettra d'organiser les Jeux et de protéger cette organisation. Je tiens à développer certains aspects de ce texte maintenant en amont de notre discussion, la première partie de ce projet de loi concerne les dispositions relatives aux 10 aux stipulations du contrat de vie de la ville haute. La France a pris des engagements clairs et précis vis-à-vis du moins olympique, nous devons les respecter pour assurer la réussite des Jeux. Tout d'abord concernant l'article, comme cela nous a été indiqué lors des auditions, il convient d'étendre la qualité d'organisateur à d'autres organes la vision actuelle étant restrictive. Concernant l'article 2 si les modifications qui sont proposées par notre assemblée n'assure pas une protection totale des Terres et en assure une partie déjà très important. L'objectif de cette loi est bien de renforcer la protection des Terres, c'est là un point essentiel du contrat de ville hôte des engagements de la France ou devant les honorer et respecté, nous y reviendrons à l'occasion de la discussion des amendements concernant la charte du volontariat olympique, il s'agit d'une ambition que nous soutenons pleinement. Cela ne devra toutefois pas nous soustraire Madame la ministre, à une réflexion sur le bénévolat dans le milieu sportif, tant au niveau local et amateur que dans le cas des grands événements sportifs. Pour rappel, l'organisation de l'Euro 2016 avait subi des surcoûts financiers non négligeables, un réseau de la requalification en contrat de travail de certains engagements bénévoles. Nous devons sécuriser ce train ce point à l'avenir et surtout, nous devons apporter devant apporter aux bénévoles des reconnaissance pleine et entière de leur investissement massif pour faire vivre le sport partout sur notre territoire. La seconde partie concerne les dispositions relatives notamment à l'aménagement du territoire, au logement, hier le déroulement. Concernant l'article 13 et l'autorisation de location des résidences universitaires par le COJO nous a été rappelé qu'une réflexion est menée avec le CIO sur les dates des Jeux afin de ne pas trop impacter la rentrée universitaire, ce qui serait une bonne chose, mais la grande inquiétude concernant. Aujourd'hui et qui concerne cette organisation, c'est bien sûr le Grand Paris Express reconnaît que Philippe Perrin avec l'arabe évoqué il y a quelques minutes. Les articles 13 et les suivants vise à sécuriser les dix hâtivement ce projet massif d'investissements dans les infrastructures structurants en Île-de-France. Madame la ministre, à la suite de la publication d'un rapport de la Cour des comptes, le gouvernement a annoncé un possible recul sur la construction de ces lignes de métro, pourtant indispensables au bon déroulement des Jeux en effet une des forces du projet Paris 2024 et la bonne desserte prévue en terme de transport. L'incertitude concernant la délivrance de ces infrastructures fait poser des inquiétudes sur le budget des Jeux. Les décisions sur le Grand Paris Express avoir des répercussions lourd de conséquences, avec la mise en 9 par le COJO d'une nouvelle organisation de transport non chiffrée non budgétisée et non envisagé initialement. Je tiens à souligner que le site qui serait certainement le plus impacté par la construire un en construction de ses lignes de métro notamment la ligne 17 et le village des médias, donc des journalistes, et donc potentiellement l'image de la France qu'il véhiculerait au travers de l'Antartique. J'ose espérer que votre gouvernement madame la ministre tiendra ses engagements et et permettre à la bonne tenue des délais, enfin une part entière de ce projet de loi concerne les dispositions relatives à l'éthique et l'intégralité. C'est là une très bonne chose que de montrer l'exemple de conserver notre Leadership dans la lutte contre les comportements pouvant remettre en cause la sincérité des résultats sportifs, de nos athlètes. Le projet de loi propose notamment de réformer l'Agence française de lutte contre le dopage, alors que celle-ci vient de se faire épingler par le Conseil constitutionnel, c'est une très bonne chose que de s'adapter aux standards juridiques du code mondial antidopage. Concernant l'article 17 bis, je partage la proposition du rapporteur, que nous avons adopté en commission un rapport me semble plus pertinent que la présence de parlementaires dans un comité des rémunérations d'autant plus que je suis convaincu que la gestion raisonnable et responsable des dirigeants du COJO. Concernant la comité d'éthique, nous sommes d'accord avec l'idée du rapport attention cependant à ne pas trop imposé de rapport au COJO qui aura déjà beaucoup d'obligations je ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'un sénateur et un député siège cela permettra notamment de faire le lien avec les collectivités sur l'article 18 et le rôle de la Cour des comptes, soyons là aussi modéré, cessons d'imposer trop de contrôle nous le son, nous connaissons les lourdeurs administratives de la France, les actions qui ont pas la confiance est érigé par le gouvernement comme une valeur forte appliquons donc ce principe voilà dans quelques points qui me semble extrêmement important d'évoquer avec vous, mes chers collègues, la loi olympique est un passage obligé, faisant d'elle une réussite tant dans les mesures adoptées que dans leur application concrète sur le terrain afin que les Jeux de 2024 soit une grande fête populaire, madame la ministre, je tiens aussi à rappeler que différents textes ont été votés et au Sénat et à l'Assemblée et qui, aujourd'hui, ces textes qui sont importants pour le sport sont dans l'attente de décret, nous attendons que ces décrets soit pris rapidement pour que ces dossiers puisse avancer. Mais la ministre tous ces points ont été que je viens d'évoquer ont été adoptés par la représentant national, donc il y a quasiment un an et le monde sportif attend ses décrets pour conclure et dans l'attente de nos débats, d'ici quelques instants, je tiens à vous rappeler, Madame la Ministre, qu'il est de tradition que les textes de loi relatif au sport sur d'adopter à l'unanimité entre les 2 chambres de notre Parlement, j'espère que cette tradition perdure, que le dialogue entre votre votre majorité à l'Assemblée nationale sera positive afin de trouver des compromis lors de la future commission mixte paritaire, je vous remercie. Merci, merci, cher collègue, la parole est à monsieur Michel Laugier pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la ministre. Monsieur le président de la commission, Madame et messieurs les rapporteurs chers collègues. Accueillir les Jeux olympiques et paralympiques nous emplit tous une immense fierté, la victoire de Paris récompense une candidature exemplaire et ouvre de belles perspectives pour l'ensemble de notre territoire par les valeurs qu'il promeut le sport disposent de cette capacité à fédérer une nation et peut s'avérer être un puissant vecteur de cohésion sociale au-delà des très nombreux héritage que les Jeux 2024 seront sur le plan matériel, ils sont ainsi également l'occasion de rassembler les Français, il est toutefois que très peu question de sport dans ce texte, dont les mesures sont principalement techniques, mais nous avons bien conscience, madame la ministre que ce projet de loi visant à honorer le contrat de ville hôte et qu'il est une première étape indispensable 15 ici à saluer l'ensemble des acteurs qui ont contribué à faire évoluer le texte dont nous allons débattre aujourd'hui au fil des discussions, il s'est enrichi, sans pour autant voir son contenu initial dénaturé certains points toutefois retenu notre attention, nous ne montrerons notamment vigilante sur la mise en place des voies olympiques et paralympiques réserver ces voies prioritaires s'étendront sur plus de 360 km épave à raison susciter de l'inquiétude chez nos concitoyens, nous comprenons la nécessité de garantir la sécurité des athlètes, mais la privatisation de ses voix de soeurs et se faire au détriment des usagers et causé un engorgement des routes afin qu'une partie des territoires de soit presque lu de l'organisation des Jeux mais cette région également engager une réflexion sur de possibles dérogations au code de l'environnement, ainsi qu'aux règlements locaux de publicité communaux et intercommunaux octroyée à nos communes, des libertés d'affichage de manière temporaire leur permettra en effet de bénéficier également des retombées médiatiques de cet événement si nous voulons que les Jeux de 2020, 4 soit réellement inclusif, les chantiers de modernisation des transports devront également profiter à tous, et assurer un désenclavement des territoires pourtant le projet du Grand Paris Express a dores et déjà été retardé le report éventuel en 2026 voire 2030, de la réalisation de la ligne 18 30 Orly et Versailles, qui doit desservir 5 sites olympiques dans le département des Yvelines nuirait à la crédibilité des jeux et contribuerait fortement à perturber l'accueil du public, sans compter sur la confiance des Français qui se virer de fait très impacté loin d'être acquise l'adhésion de nos concitoyens reposera également sur le respect de l'éthique et de la transparence sur ces sujets, ce projet de loi comporte des mesures ambitieuses et exemplaire, toutefois, l'article 17 bis a retenu notre attention : le texte adopté par la semaine nationale proposé de faire siéger à titre consultatif un député, un sénateur au sein du comité d'éthique du comité des rémunérations si et l'ce n'est qu'en apparence que des améliorations qui était en réalité les parlementaires aurait disposer que d'une voix consultative et aurait été dans l'incapacité de peser véritablement cette mesure paraissait donc artificielle et cosmétiques à l'aune de ces éléments, notre collègue Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission de la culture, nous a proposé d'associer les parlementaires différemment et nos débats sur ce sujet seront je l'espère, constructif, madame la ministre, Jane évoquer ici que certains aspects dans un projet de loi ambitieux, équilibré, bien d'autres, Ribéry d'être salué le groupe Union centriste soutiendra bien évidemment ce texte, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Vincent Capo Canellas pour le groupe Union centriste pour 4 minutes chers collègues. Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, mes chers collègues, Madame et Monsieur, les rapporteurs le chronomètre en sport comme dans l'hémicycle, étant toujours impitoyable, je vais être assez Direct, ce qui motive ce texte, c'est bien sûr la volonté de respecter les engagements normaux comme pays hôte des Jeux olympiques et paralympiques prend lorsqu'il est candidat, l'objet principal du projet de loi est donc de raccourcir de simplifier des procédures souvent trop longues en respectant pour autant nos grands principes du droit, je savais sur ce point, le travail de nos commissions et de nos rapporteurs : il s'agit en effet du manifestation hors norme, la plus importante à l'échelle planétaire qui rassemble autour des valeurs du sport, un événement qui réunit les pays les plus divers, parfois antagonistes et permet aux échanges internationaux une parenthèse utile il y a un miracle olympique les et paralympiques porte un message universel en cela les territoires qui accueilleront les Jeux savent que leur responsabilité est grande, il s'agit d'abord d'accueillir le monde entier autour des valeurs universelles, mais aussi le permette le déroulement des preuves sportive de réussir une belle fête populaire, il s'agit aussi, et c'est l'exigence du CIO de laisser une trace durable et utile pour les territoires d'accueil et leur population. Les GO. Mais pour paralympique porte l'exigence d'un héritage durable cette exigence, nous devons l'martelé, y compris parfois devant les inspections missionné par le gouvernement, qui s'interroge sur l'utilité d'un héritage olympique réussir les Jeux, c'est assurer le respect du calendrier et, tout comme notre unité, a été essentielle dans la candidature, elle sera déterminante dans la bonne réalisation des équipements olympiques les collectivités autour de la ville de Paris, de la maire de Paris, dans différentes communes dont certaines qui me sont chers au Bourget l'ni en Seine-Saint-Denis mais aussi dans d'autres départements et de nombreuses villes avec la communauté spot sportives au 1er rang de laquelle Tony Estanguet et Bernard Lapasset, ces collectivités ont joué un rôle décisif,

nous faisons le pari que la bonne relation avec la Solideo assurera la prise en compte de cette exigence de proximité, c'est sans doute le meilleur garant au-delà des structures même janvier à l'essentiel, ces collectivités porte ensemble le même message réussir les Jeux, c'est d'abord respecter les engagements pris en matière de transport et d'accessibilité sur ce point, je veux dire ici solennellement que le gouvernement est face à sa propre responsabilité, puisque la réalisation des lignes du Grand Paris Express pour 2024 fait partie des engagements que notre pays a pris auprès du CIO, autant on peut comprendre que soit engagé un examen des échéances du Grand Paris Express, autant il devient difficilement explicable et pour tout dire injustifiable de continuer a tardé à demander à la Société du Grand Paris tout mettre en oeuvre pour bien accueillir les athlètes, les accompagnateurs, les journalistes et les spectateurs, la lettre envoyée par la ministre des Transports, oser le 30 janvier n'a pas manqué d'étonner, elle oublie curieusement de rappeler la nécessité de livrer pour 2024 la gare le Bourget, aéroport, qui est située sur la ligne 17, cette gare desservira pourtant le centre de presse des JO, soit 24000 journalistes le gouvernement me semble-t-il doit réaffirmer très vite cet objectif à vrai dire, il aurait pu et dû le faire avant le 13 septembre et en toute hypothèse, après la décision connue du CIO, il me semble qu'il a déjà trop tardé et ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité sur ce point, il convient donc de se donner à un objectif clair, au moment où une communication publique et de fête organisée et ne pas le faire, chacun en conviendra, n'est pas la bonne façon d'organiser le succès de l'opération, donc les gares olympique oui mais toutes les gares olympique sans un oublié une seule voilà donc il nous mesurons bien sûr la mobilisation chacun à l'aune de ces différents objectifs, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur Jean-Jacques Lozach, pour le groupe socialiste et républicain pour 5 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre Mesdames, messieurs les présidents de Commissions mesdames messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2000 24 à Paris mais d'abord l'occasion de féliciter tous les acteurs de cette belle réussite qui est notre sélection et de se réjouir de voir un siècle après les Jeux olympiques d'été de 2924 notre capital accueillir à nouveau l'événement sportif mondial par excellence, après cette phase intense de mobilisation en faveur de la candidature, c'est un rassemblement, une préparation d'une ampleur très conséquent qui s'ouvrent devant nous la traduction législative de nos engagements et la mise en oeuvre de mesures dérogatoires vise à préparer au mieux le terrain pour ceux qui sont à l'oeuvre pour faire de Paris 2024 grand succès une fête populaire, un moment de Concorde nationale depuis le 13 septembre les pierres de l'édifice à bâtir se multiplient : nomination d'un délégué interministériel constitue si du COJO qu': création de la Solideo, on pourrait dire que ce projet de loi est en quelque sorte de permis de construire, de ces Jeux olympiques et paralympiques, on y trouve en effet les transpositions des obligations qui découlent du contrat de ville hôte signé à Lima, en septembre dernier, c'est l'objet des titres 1 2 et 3 le titre 4 permet de placer la France en tête pour l'reste j'ai relatifs à l'éthique, la transparence et l'intégrité, ce dernier titre est emblématique du degré d'exigence que nous mettons à respecter les valeurs que nous partageons, dont la traduction ne se limite pas au terrain de compétition mais concerne la mise en oeuvre des jouets dans sa globalité, je forme le voeu que ces règles devienne un nouveau standard en termes d'organisation de grands événements sportifs, la nécessité de maintenir la cohérence de ce projet de loi relativement technique a été équilibré par votre annonce Madame la Ministre, d'un projet de loi, Sport et société pour l'année prochaine le miroir de ce concentrer de sport du plus haut niveau que sont les Jeux olympiques et paralympiques réside dans cet objectif de société qui est d'offrir au plus grand nombre, la possibilité de pratiquer au quotidien une activité physique et sportive, le succès de la candidature de l'organisation offre à notre pays une opportunité formidable de progresser vers cette ambition élevée, ça devra faire partie de l'héritage olympique quelques sujets ont pu provoquer des débats dans l'opinion publique, par exemple, les dérogations aux interdictions et restrictions en matière d'affichage publicitaire dans et autour des sites olympiques sont à la fois un engagement présent dans le contrat de ville hôte et un levier de financement très conséquent pour le COJO, n'oublions pas que l'État accordé sa Karentie au bénéfice du colloque et que tout déficit financier de la structure sera pris en charge par la puissance publique la faculté attribué à la Cour des comptes, de pouvoir effectuer un contrôle plein et entier des comptes de la gestion du ou de toute autre structure de droit privé qui pourrait être de créer par la suite me semble constituer un nouveau signe de l'engagement de la France à tenir des exemplaire, le suivi des éléments budgétaires concernant les jeux est facilitée par la création d'un programme dédié dans le PLF pour 2018, nous souhaitons également la mise en place d'une loi de programmation budgétaire 2019, 2024 qui permettrait d'affirmer nettement le caractère pluriannuel de ce projet, je rappelle ici l'initiative sénatoriale à l'origine de la loi du 1er mars 2017 dans ce cadre législatif, nous avions déjà souhaité étendre les obligations déclaratives à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique le Champ du dispositif se trouve donc aujourd'hui complétée de manière pertinente concernant la société de livraison des ouvrages olympiques, je voudrais saluer l'initiative de nos collègues de l'Assemblée nationale prévoyant de doter la Solideo chargée d'insertion et de responsabilité sociale, je suis heureux de constater que les jeunes 2000 24 sur l'occasion de parachever le travail législatives relatives à lutte contre le dopage en complétant le travail de transposition effectués par l'ordonnance du 30 septembre 2015 c'est en particulier en terme de procédure que l'arrivée sera importante en séparant les fonctions de poursuites essaie de jugement demain dans la suite des travaux engagés depuis longtemps dans la loi du 1er mars je salue la modification du code pénal visant à réprimer le délit de corruption sportive active qui pourrait priver en partie cette disposition cette loi illustre l'empreinte accepter consenti du mouvement sportif international via le CIO dans le droit d'un État pour l'organisation d'un événement sportif planétaire se traduit par de nombreuses dérogations dérogations indispensables à une bonne préparation, elle-même liée à la pertinence du contenu du dossier de candidature par ailleurs n'oublions pas que les JO, offre une Exposition unique dans le cadre de la mondialisation, une réalité qui ne serait sacrifié les attentes des téléspectateurs français notamment ses concerts, le nombre d'heures de diffusion en clair d'Ombrie bénéficier le service public de l'audiovisuel se pose par ailleurs la question de la diffusion organisée par une collectivité ou une association sur une place publique ou dans une salle des fêtes, les collègues en ont parlé, je n'y reviens pas, je terminerai mon propos par une citation de Ryad Salem, membre de l'équipe de France handisport candidaté pour Paris 2024 c'était une respiration vitale l'événement catalyseur qui ouvrira les vannes d'une nouvelle dynamique, refusant toute frilosité ou renoncement prématuré en effet le voeu que ces JO de Paris conforte la place du sport dans le discours national culturel, rejoignant ainsi le combat de Pierre de Coubertin qui considérait les JO, non comme une fin en soi mais comme un outil éducatif et enfin exprime tous mes voeux de réussite aux équipes de France participant aux Jeux d'hiver de Pyeongchang à partir de la fin de cette. La parole est à Madame Colette Mélot pour 3 minutes.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais chers collègues. L'organisation des Jeux olympiques, dont nous débattons aujourd'hui porte à Noël, une véritable ambiguïté, les jeux sont une opportunité formidable pour notre pays, mais ils peuvent aussi générer de lourdes conséquences financières, ce projet de loi doit donc nous servir de ligne conductrice pour que ces Jeux olympiques et paralympiques soit un atout durable pour notre pays, prétend aussi une attention toute particulière, le département de Seine-et-Marne, qui est mon département fait partie de ces territoires franciliens directement concernés par l'organisation de cet événement de portée internationale, la commune de Vaires-sur-Marne, aura la chance d'accueillir les compétitions d'aviron et de canoë drainant des milliers de télé de spectateurs sur notre territoire, dynamisant les équipements touristiques, les retombées directes, de cet événement sont incontestables, chantier de 75 millions d'euros, l'aménagement de la base nautique régional est un atout d'aménagement du territoire et de développement économique, les Jeux olympiques nous permettront de mettre en lumière notre savoir-faire et de développer notre offre touristique, la reconversion du site est d'ailleurs partie intégrante du projet puisque le site de Vaires-sur-Marne hébergera après les Jeux olympiques, le pôle d'entraînement national des équipes de France, c'est cela l'enjeu de durabilité des installations olympiques pour autant les infrastructures doivent suivre comment en effet assuré le transport de ces milliers de personnes jusqu'en Seine-et-Marne si les accès ne sont pas réalisés, comment assurer le passage des nouveaux trains dans nos gares, alors même que la plupart des sites ne sont pas adaptées en raison de problèmes dans la construction des quais de gare, comment encore transporter et spectateurs des gares vers les sites si les pouvoirs publics ne mettent pas les moyens pour moderniser les routes et déployer une flotte de transport public digne de cet événement, nous le savons, l'amélioration de la mobilité de France est indispensable à son développement, nous attendons donc un calendrier réaliste et des coûts maîtrisés du Grand Paris Express qui je le rappelle, a été l'un des points décisifs dans l'obtention des JO tant de questions, mes chers collègues, qui doivent guider notre réflexion ces Jeux olympiques sont un défi relevé relevons-le avec témérité et prudence, nos collègues de l'Assemblée nationale ont inscrit dans la loi des objectifs stratégiques en matière de transports franciliens ce travail mérite d'être salué, il importe de poursuivre et de le compléter, c'est l'esprit des amendements que nous vous présenterons une préparation optimale et une vision à long terme sur l'avenir des installations, j'espère que nous saurons vous convaincre de leur pertinence puisque nous parlons d'argent public, je crois qu'il convient de saluer les avancées de cette loi en matière de transparence l'engagement pris de contrôler les intérêts des organisateurs de ces Jeux olympiques des entreprises chargées des projets de construction ou de modernisation est admirable, monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les jeux olympiques et paralympiques doivent être un héritage durable pour notre territoire francilien, fin de semaine dernière, je conclus Monsieur le Président, une équipe de chercheurs de l'université Paris a lancé un observatoire des JO pour surveiller du dérapage budgétaire, faisons nôtre leur mot d'ordre alertées dès aujourd'hui pour ne pas subir dans 10 ans. Voilà, Madame le Ministre Monsieur ministre, il ne vous reste que 6 minutes avant la suspension, je vous propose de les utiliser si vous souhaitez plus de temps à la reprise, nous vous en donnerons Monsieur le Ministre, vous commencez. Merci beaucoup, merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, très je vous prie de bien vouloir m'excuser, j'étais coincé dans ce beau département d'Ariège avec les chutes de neige, les avions ont tous été décalé, ce qui explique mon échelle retard pour cette discussion générale juste juste 3 points en réponse aux différentes interventions, comme le rappelait le sénateur Laugier, l'objectif du titre de et d'accélérer l'ensemble des procédures, il s'agit de pouvoir garder les mêmes droits mais d'accélérer les procédures afin de s'assurer que l'ensemble des infrastructures qu'elles soient pérennes ou qu'elles soient temporaires puissent être livrés à temps, c'est-à-dire dans les 7 années qui en termes de construction est assez court, mais en même temps long et il faut pouvoir dans ce temps imparti livrer l'ensemble des procédures, le 2ème élément sur lequel je voulais insister, cette charte d'insertion sociale, que plusieurs d'entre vous ont mentionné notamment le sénateur Pierre Laurent, cette charte d'insertion, elle a, elle est le fruit des débats parlementaires, au début, inclus dans le projet de loi, elle est donc le fruit de ces débats et elle vise à 2 choses : d'une part, assurer le volet inclusif de ce de ces Jeux olympiques et paralympiques et en même temps, d'assurer l'héritage par la formation par l'accompagnement de l'ensemble des personnes qui vont concourir, participer à l'ensemble de ces Jeux olympiques et paralympiques enfin dernier point sur le volet transport plusieurs d'entre vous ne dont notamment le sénateur cap aucun ont évoqué ce sujet des transports, alors, de 2 points, les transports, on en discutera dans le cas des amendements, il y a des dispositions qui visent à sécuriser ce qu'on appelle le Charles-de-Gaulle Express le Charles-de-Gaulle Express il est, il est bien inclus dans le dossier de candidature en réponse à au sénateur Pierre Laurent, il est bien inclus dans le dossier de de candidatures, s'agissant de la Société du Grand Paris, comme vous le savez, on a agi, essayer d'agir avec méthode énormément de concertation était porté par la ministre des Transports, en association avec l'ensemble des élus locaux, évidemment dans ces concertations l'ensemble des données, si je puis dire, l'ensemble des obligations des engagements et des contraintes sont prises en compte et notamment celles relatifs aux Jeux olympiques, alors je prends bien note bien, note du Point, qui est que le plus vite, ces annonces sont faites le mieux ce sera, y compris pour les Jeux olympiques, mais soyez assuré, en tout cas que le gouvernement agit avec méthode, en prenant en compte l'ensemble de ces, de ces faisceaux de contrainte ou d'obligations. La le ministre, La le ministre, vous avez la parole pour 3 minutes 3 minutes 30. Je réponds : faites notamment au sénateur Kern, eu égard aux interrogations sur la diffusion télévisuelle en fait des Jeux de 2024 je ne à vous apporter en quelques éléments d'information, les droits de diffusion de l'édition des Jeux de 2024 sont actuellement détenus par le groupe Discovery ou l'avait dit : mais enfin, mais font en ce moment, l'objet de négociations pour des sous-licences d'exploitation pour des chaînes gratuites, si cela est conforme au décret relatif à la diffusion des et. Tellement d'importance majeure qui vise à améliorer l'accès du public aux retransmissions des compétitions, les modalités de diffusion des épreuves en public font nécessairement partie de ces négociations en cours, à fortiori, ces droits de diffusion n'ont pas encore été concédées et donc il n'est donc pas permis de déterminer à ce jour, les modalités d'exploitation de droits de cette compétition, dès lors, il me semble un peu aujourd'hui, je dirais, j'aurais pas nécessaire de modifier le cadre juridique en cours de négociation sans intervention du législateur pourrait entraîner contentieux susceptibles d'apporter d'aboutir au paiement d'indemnités considérables à la charge de l'État, je m'engage donc devant vous à poursuivre les échanges francs que j'ai fréquemment gérés, entretenus avec les acteurs de l'audiovisuel pour que les négociations en cours puisse se conclure sur une solution qui permettrait à tous les Français d'avoir accès aux retransmissions des compétitions, il me paraît nécessaire de respecter la liberté contractuelle des acteurs impliqués mais je tiens à vous dire que je me faire économiser près de vos préoccupations merci. Merci madame la ministre, de me permettre de suspendre la séance, elle sera reprise à 16 heures 15 pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est suspendue parce que j'ai 45 pardon.

La séance est repris accompagné du président de la commission des lois du Sénat et du secrétaire général de la présidence, il s'agissait par notre présence, de rendre hommage, au nom du Sénat à un préfet de la République, lâchement assassiné il y a 20 ans, il s'agissait aussi d'être aux côtés de Madame Érignac et ses enfants en leur témoignant à la fois notre soutien, notre affection. Rien ne justifiera jamais la mort d'un homme qui a incarné la République une République une et indivisible, rendre hommage à Claude Érignac, c'est avant tout continuer à nous battre ensemble pour cet idéal auquel je sais que vous êtes tous et toutes, profondément attaché.

L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement sont retransmises en Direct sur Public Sénat sur chacun aura à coeur à respecter son temps et bien sûr avoir comme principe le respect des uns et des autres, la parole est à notre collègue Maryvonne Blondin pour le groupe socialiste et républicain. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'action et des Comptes publics, monsieur le ministre, jeudi dernier, à l'issue du comité interministériel de la transformation public vous avez annoncé plusieurs pistes de réforme de l'État, dont l'extension des recours aux contractuels, alors même que les syndicats réclamaient fin janvier, un nouveau plan de titularisation et une meilleure sécurisation des parcours professionnels plus inquiétant encore, vous évoquez un plan de départs volontaires pour les agents de la forme de la fonction publique cette annonce nous laisse plus que perplexe sur le fond comme sur la forme, d'autant qu'avait, dans un contexte de défiance déjà très fort à l'égard des fonctionnaires, gel du point d'indice, rétablissement du jour de carence, les agents publics attachés aux valeurs républicaines n'ont eu de cesse d'être pointé du doigt ces dernières, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut rendre notre action publique plus efficace en l'adaptant au changement de notre époque et enfant et en optimisant son fonctionnement mais moderniser l'action publique, ce n'est pas la démanteler encore moins lorsque les agents des hôpitaux, des et pas de la police etc manifestent leur souffrance et leur besoin criant de personnel supplémentaire ou lorsque les citoyens voient leur leur service public de proximité fermé et que l'action de l'État peine à être accessible à tous sur l'ensemble de notre territoire, monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des clarifications sur ces annonces et nous dire quels secteurs précis de l'action publique seront concernés par merci. Neto, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des Comptes publics monsieur Olivier Dussopt la parole monsieur le Ministre pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Blondin, votre question me permet de répondre, je l'espère va permettent de répondre espère votre perplexité le 1er ministre avec 500 donc dans l'plantations et d'objectifs qui vont faire l'objet d'une concertation entre le gouvernement, les organisations syndicales et les différents collèges employeurs sur le dialogue social sur la rémunération sur les conditions de recrutement dans la fonction publique, que ce soit par concours ou par la voie de la contractualisation dont nous pensons que les des conditions d'accès peuvent être élargie, nous avons aussi une réflexion à mener sur l'évolution de la carrière des agents leur progression de carrière, leur formation et leur mobilité, il arrive, il arrivera qu'avec l'évolution de telle ou telle technologie des métiers de la fonction publique soit modifié, remise en cause que l'émission soit dans leur utilité même interrogé il arrivera avec la modernisation de l'administration et des établissements publics puissent être qui puisse être reproché et dans ces cas-là, c'est qu'elle apprécie, nous envisageons effectivement de proposer aux agents concernés et strictement à ces agents concernés des plans de départs volontaires, la réalité qu'il existe déjà une indemnité départ volontaire dans la fonction publique depuis 9 ans avec des conditions et des critères d'accès qui sont particulièrement complexe et difficile à mettre en oeuvre, malgré cela, selon les années, ce sont 700 à 1300 personne qui quitte les rangs de la fonction publique de cette manière le plan départs volontaires aura à être discuté avec les organisations syndicales pour répondre à ces agents, je le répète, il ne s'agit pas d'un temps volontaire générale il n'y a pas de lien entre ce plan volante, départs volontaires ou cette technique et le montant, le nombre de postes a diminué dans la fonction publique, ça ne s'adressera qu'aux volontaires, nous voulons garantir Édouard reclassements offrir une possibilité de mobilité supplémentaire, c'est une possibilité, en plus, et non pas un droit au moins.

aux établissements de, des berges morts, de personnes âgées, allez le dire à l'éducation nationale est une des clés d'amélioration de l'efficacité du service public et l'amélioration du management, on vous annonce vont à rebours d'un management efficace. Mais la parole est à. Notre collègue Joël guerrier pour le groupe, les indépendants, vous avez la parole. Madame la ministre, les préfectures ont fermé l'accueil du public pour les mettre et création des véhicules, mais toute la procédure est dématérialisé depuis novembre 2017, nous pouvons désormais considérer que c'est un progrès, puisque finalement plus besoin de se dépasser, les démarches sont facilitées, mais cela n'est pas vrai pour tout le monde, d'une part des sites marchands trompeur sont bien mieux référencés, que les mots par les moteurs de recherche que le site du gouvernement, ils profitent donc du désengagement de l'État pour facturer lourdement leur service, d'autre part sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, des milliers de personnes sont bloquées suite à des dysfonctionnements informatiques, sans compter ceux qui renoncent et qui se retrouvent dans des situations d'illégalité, Madame la Ministre, où est le service public quand un usager incapable de remplir ses obligations se retrouve seul devant une machine sans personne à qui parler pour l'aider dans ses démarches, tous les Français ne sont pas des cyber citoyens nuit 3,0 produit nouvelle précarité citoyenne, accentue la fracture numérique et crée parfois des situations kafkaïennes que penser d'un État qui dématérialise son administration en créant de l'exclusion numérique, madame la ministre, quelle réponse apportez-vous à ces problématiques.

les demandes de titres de circulation concerne chaque année en France, plus de 30 millions d'opérations et en effet, dans le cas de la réforme préfecture nouvelle génération là des médailles dématérialisation de ces procédures, a été décidé dans la triple perspective d'une sécurisation accrue des titres délivrés de l'amélioration de l'efficience de l'administration de l'État, enfin de la simplification des procédures pour les usagers, notamment la fin de l'obligation de se rendre à des guichets d'ores et déjà 2 millions de permis de conduire et 1,5 1000000 de cartes grises ont été délivrées dans la très grande majorité des cas, ces procédures fonctionnent bien et sont un véritable outil de simplification pour les usagers se sont en effet autant de déplacements moins et d'attente devant les guichets, toutefois, comme pour toute réforme d'ampleur des dysfonctionnements sont apparus lors du déploiement de la réforme sur un nombre d'imiter d'opérations des services du ministère de l'Intérieur, ont mis en place un plan d'action pour traiter ces difficultés qui est en cours de mise en oeuvre et qui repose à la fois sur des correctifs informatique sur l'amélioration de la qualité de la connexion portail usagers et sur le renforcement de la chaîne de soutien aux utilisateurs, par ailleurs, certains administrés éprouvent, comme vous l'indiquez, des difficultés pour accéder à des services publics numériques, leur situation a bien été prise en compte dans le déploiement de cette réforme, en effet, dans toutes les préfectures et sous-préfectures qui délivrait des titres, c'est-à-dire plus de 300 communes en France des points numériques ont été mis en place, ils sont animés par des médiateurs numérique capable d'assister les usagers de manière personnalisée, le ministère de l'Intérieur propose donc un accompagnement humain pour les personnes qui sont le plus éloignés de ces nouvelles technologies de cette manière la réforme permet à la fois d'économiser des millions d'heures d'attente au guichet tout en assurant un soutien individualisé des administrateurs des administrés qui en ont besoin, je vous remercie, Dominique Seux. Madame la ministre, je m'attendais à cette réponse dictée par l'administration et qui est correspond absolument pas à ce qui est vécu par des milliers de personnes donc je me porte aujourd'hui pas parole parce que nous avons beaucoup de gens qui sont désappointés, qui se retrouvent dans des situations kafkaïennes, du fait notamment que la 4Matic c'est binaire et quand vous êtes face à un écran et que vous avez pas la réponse que vous avez qui est attendu par l'écran, vous êtes bloqué et vous retrouvez dans une situation complètement incroyable, alors vous allez en préfecture, ce que j'ai fait et en préfecture ou trouvé personne pour vous indiquer quoi que ce soit vous avez personne, alors peut-être qu'il y a quelque peu sous-préfecture qui le fait qui font le nécessaire mais ce n'est pas vrai, de manière et donc moi je pense qu'il faut vraiment prendre cette condition importante et de mettre en place de l'humain, parce que n'y a de ressources de richesse que d'hommes, et cela signifie qu'il faudra au minimum un accompagnement humain à des situations qui sont parfois très tendu, très difficile et qui sont franchement pas dans pas dans le sens que nous devons donner à des méthanisation doit s'accompagner la pas conduire à la déshumanisation et je crois que c'est ça l'essentiel. Merci, la parole et être. Collègue Roger Karoutchi pour le groupe, les républicains. Monsieur le président, Monsieur le 1er ministre votre gouvernement au mois de novembre une circulaire à tous les préfets, leur demandant une grande fermeté à l'égard des immigrés en situation irrégulière ou des déboutés du droit d'asile, à quelques jours du dépôt de votre texte qui passera en conseil des ministres, il bien compris le 21 sur l'immigration et droit d'asile, à quelques jours d'une décision qui a cassé pour le moment, la volonté du conseil régional de ne faire de faire en sorte que tout le monde soit à égalité sur la réduction des tarifs sociaux en Île-de-France, avec évidemment pas de faveur particulière pour ceux qui sont en situation irrégulière comme votre circulaire donné jusqu'au mois de février au préfet pour faire le point monsieur le 1er ministre est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes sur la lutte contre l'immigration irrégulière et sur les déboutés du droit d'asile. La parole est au secrétaire qui est en charge des relations avec le Parlement monsieur Christophe Castaner, maire. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Karoutchi voilà un sujet qui doit nous mobiliser : comment peut-on accepter aujourd'hui que 96 pourcent des décisions de justice de reconduite à la frontière ne soit pas mis en avant évidemment ce phénomène n'est pas nouveau, nous savons tous que ces dernières années et je n'en citerai aucune pour ne pas situer on connaît cela tout simplement parce que la France a longtemps pensé que par la complexité des procédures, nous pourrions faire en sorte que des femmes et des hommes qui, pour les réfugiés qui ont fui leur pays pour cause de menaces de mort sont venus en France et ne serait pas attendre des heures, des jours au pied d'une préfecture, certains ont pensé que la complexité de l'accès à la reconnaissance de droits pouvait les empêcher de lutter de lutter pour la survie et puis il y a aussi les migrants économiques et les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui à travers toute l'Europe et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité se donner les moyens pour que nous puissions mettre en oeuvre les décisions de reconduite à la frontière, quand elles sont nécessaires à la fois assumer notre part de devoir sur l'asile, d'humanité et je ne doute pas que ça puisse nous rassembler tous sur l'ensemble de ces bons pour ces femmes et ces hommes qui ont le statut de réfugié pour lequel on le reconnaît, pour lequel nous devons faire des efforts en matière d'intégration, mais à la fois pour celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester en France qui ont été égarés dans l'orientation et dans l'espérance de pour être accueillis et d'avoir un titre sans difficulté, dès lors qu'il y a une décision de justice, il faut se donner les moyens de reconduire à la frontière, ce qui ne peuvent pas rester, c'est la raison pour laquelle le texte qui sera présenté à la fin du mois de février par le ministre de l'Intérieur, donne les moyens, notamment en se prononçant sur le Duc le les délais de rétention pour atteindre des moyennes qui permettent de monter jusqu'à 90 jours alors que le cadre européen est à 180 jours pour faire en sorte quand on sait qu'une décision sur 2 des autorités consulaires arrive après le 45ème jour nous aurions les moyens de mettre en oeuvre ces décisions de reconduite à la frontière, c'est à la fois l'ambition d'humanité, mais aussi une exigence de fermeté et de vérité à laquelle les Français nous attendent. Seul ministre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand je vous entends, je me dis : j'aurais pu le dire à sa place, il y a quelques années, je l'aurais fait sauf que dans le budget 2018 vous baisser les crédits de raccompagnement à la frontière par rapport à 2017, alors je sais pas comment voulez raccompagner avec fermeté avec moins d'argent, je sais pas, de la même manière, sur bien des sujets, notamment dans le ce que l'on a, en tout cas du texte de loi à venir vous durcissait les conditions, notamment en élargissant les capacités de recours en élargissant la capacité d'action des uns des autres pour retarder, alors moi j'entends bien le discours de fermeté du gouvernement, je ne vois pas dans la pratique, la réalité concrète de cette fermeté et quant à vous dire sur les réfugiés ici tous les 2 élus et tous les élus LR en particulier sont extrêmement attachés à ce que ceux qui obtiennent le statut de réfugié soit bien traité, alors Monsieur le ministre, si c'est le cas, autant il faut mettre des crédits sur leur accompagnement aux frontières, autant il faut des crédits pour réellement bien intégré, parce que pour le moment ça n'est pas le cas.

Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux ministre de la Justice Madame la ministre lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de Bobigny, la semaine dernière la procureur de la République a lancé un appel au secours sur la capacité de la justice à répondre à la délinquance, l'émotion est telle que le journal Le Monde, a lui-même souhaité mettre à ça une cet appel qui a été entendu par tous comme étant un élément qui doit maintenant appeler des décisions fortes bien sûr va au-delà de la Seine-Saint-Denis et interpellé sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de juridictions, il pose le problème de l'effectivité de la justice pénale et de l'égalité de tous devant la sanction il y a des départements où, faute de moyens, le parquet n'a plus la capacité de poursuivre le problème n'est pas nouveau mais il devient insupportable à tous sauf aux délinquants, on fait, disait ce matin encore, sur les ondes, la procureure, on fait des choix on priorisent par exemple les vols à l'étalage ou l'usage de stupéfiants ne sont pas poursuivis en dessous d'un certain seuil, cette réalité, celle de 2ème, par quelle France, elle doit tous nous interpellés la dégradation de la réponse pénale dans ce département où la délinquance atteint malheureusement des sommets est une réalité 418 dossiers d'instruction stagnent dans les rayons, je cite ici la procureure sans réelle perspective ni à court ni à moyen terme, faute de moyens encore le parquet contraint quotidiennement ça réponse pénale ou de la différer et quand le taux national de réponses pénales et de 50 pourcent des affaires poursuivable il y a de 31 pourcent en Seine-Saint-Denis, le procureur pose la question est-ce mission impossible de prendre des mesures exceptionnelles pour un département exceptionnelle et on a tous relevé que, en 2018, semble-t-il, il n'y aura pas de créations de postes au parquet de Bobigny, madame la ministre, dans ce contexte, comment pensez-vous répondre aux inquiétudes du procureur de Bobigny et, plus largement, assurer l'effectivité des moyens des parquets, y a-t-il d'autres juridictions qui soit dans ce cas-là, et comment pensez-vous en la justice égale pour tous dans notre République, je remercie. Monsieur le président, Mesdames laissez n'attriste, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Capo Canellas, votre question est évidemment très percutante et il est exact que le discours de Madame, la procureure de Bobigny a éveillé bien des inquiétudes, je dois dire pour autant que nous sommes extrêmement conscient de cette situation et que j'ai moi-même été alerté sur la situation de Bobigny

dès le budget 2018, augmenter le budget de la justice, de 3,9 pourcent que nous avons créé 148 postes qui viendront renforcer l'effectif des magistrats et des équipes autour des magistrats, je rappelle également que la loi de programmation qui vous sera présenté prochainement viendra dans la durée, renforcer ses effectifs sur Bobigny, vous avez sans doute été mal informé, monsieur le sénateur, parce que nous allons renforcer les effectifs de magistrats du siège et ils passeront de 131 à 137, nous allons également renforcer les effectifs du parquet, qui passeront de 53 à 57 et qui, si le président du tribunal en fait la proposition permettront, ouverture d'une 2ème, chambre de comparution immédiate, les effectifs des fonctionnaires seront pérennisés, ce qui donnera réellement les moyens à cette 2ème, chambre de comparution immédiate de fonctionner ainsi réellement l'action publique sera confortée et pour apporter une réponse pénale, me semble-t-il tout à fait satisfaisante dans le sens de ce qui est exigé ces mêmes réponses seront confortées par 2 autres éléments : d'une part, la révision constitutionnelle qui viendra renforcer le statut du parquet et cela était important pour permettre aux magistrats du parquet de remplir la totalité de leur office et d'autre part, le chantier de la justice qui devront trouver leur achèvement dans la loi de programmation et la loi pénale dont je faisais état il y a un instant donne compte également en terme procéduraux en termes de simplification en terme de transformation numérique des éléments puissants pour que les magistrats du parquet puissent aussi apporter une réponse publique qui soit satisfaisante, c'est exactement l'ambition du gouvernement et nous espérons au groupe lumière répondre aux questions. C'est merci. La parole est maintenant notre collègue Frédéric Marchand pour le groupe, la République en marche la parole. Ma question s'adresse à monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, lors du vote du budget 2018, nous avons constaté que les crédits dédiés à la sécurité dans notre pays apportent désormais aux policiers et aux gendarmes des moyens matériels et humains à la hauteur de leur mission et de leur niveau de sollicitation, le budget 2018 est en résonance avec l'arsenal législatif mis en place à travers la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, face auxquelles nous ne baisserons pas la garde, ni dans la volonté, ni dans les moyens alloués par ailleurs dès 2018 et tout au long de la législature en matière d'effectifs, les 2 forces de sécurité, police et gendarmerie seront dotés de 10000 emplois supplémentaires, conformément aux engagements pris par le président de la République, l'année 2018 sera aussi celle de la mise en place de la police de sécurité du quotidien révolution qui suscite beaucoup d'attentes parmi les forces de l'ordre comme parmi les Français et notamment chez le nombre d'élus locaux, mes chers collègues, pour qui la sécurité est une priorité du quotidien, c'est dans ce cadre qu'une consultation vient de s'achever, elle a permis à 70000 policiers, gendarmes, de s'exprimer, du jamais vu dans l'histoire de notre pays, il ressort de cette consultation que 74 pourcent des personnes consultées souhaitent la suppression d'un certain nombre de tâches indues, nous avons la chance de pouvoir compter sur des policiers formés aux situations les plus extrêmes, aux techniques les plus éprouvées et on ne saurait épuiser cette richesse en mission pour lesquelles l'expertise de la police n'est pas indispensable, monsieur le Ministre de l'Intérieur a souhaité engager une réflexion autour de ces fameuses taches indues pour améliorer le fonctionnement et le quotidien des forces de police en évoquant le possible recours aux entreprises privées de sécurité, le rôle aujourd'hui dévolues aux agents de sécurité privés de prendre en charge sur notre territoire, la sécurité des biens et des personnes dans les espaces privés qu'ils soient ouverts ou non publique, l'objectif de ce continuum de sécurité, on se le discours par Mireille et sécurité pour être, dans quel domaine il est possible d'aller plus loin, pouvez-vous donc Monsieur le Ministre, nous éclairer sur ses missions indues qui pourrait être confié demain aux entreprises de sécurité privées et sur les éléments de méthodes mises en oeuvre, je vous remercie.

tout ne doit pas se réduire à des questions financières, mais en même temps, il me paraît toujours important de lire le projet de loi de finances que certes, cette assemblée n'a pas voté, mais qui a été votée, qui aujourd'hui est la règle de conduite des membres du gouvernement et développe les moyens et sur le ministère de l'Intérieur, sans pour autant user d'un droit de réplique à monsieur le ministre, Karoutchi sur le ministère de l'Intérieur, je voudrais quand même rappeler que c'est un budget en hausse de 6,8 quand tu as la ligne Asile intégration immigration tout à l'heure, nous évoquions une baisse, je suis assez surprise parce qu'elle augmente de 28 pourcent 28 pourcent parce que ça correspond à une priorité politique de ce que nous devons mettre en oeuvre mais, Monsieur le Sénateur, vous poser une question qui est essentiel qui ne doit pas se traduire seulement par la question des dotations financières mais par la coordination de l'ensemble des acteurs sur les forces de police, évidemment, c'est ce que nous devons faire parce que, sur un territoire comme le vôtre, nous ne traitons pas des questions de sécurité, de la même façon à Clarica seul Bailleul ou Lille, il est essentiel que nous puissions par une police de proximité sur les territoires définir au plus près des territoires au plus près des problématiques avec les élus locaux et chacun est ici particulièrement attaché à l'action de nos élus locaux avec les élus locaux, déterminer les meilleures façons d'intervenir et c'est cela que nous voulons mettre Endeavour notamment par la police de proximité, notamment parce que il y a d'autres actions et nous savons que le Sénat travaille actuellement sur la plume, la problématique des forces de sécurité intérieure et de leurs moyens, ainsi que vous l'avez évoqué sur le lien avec. Les c'est que le secteur privé qui intervient sur ce sujet, je crois que la presse, qui sort le mardi soir, mais qui est publique, le mercredi matin, évoquera ce sujet la nécessaire coordination entre tous les acteurs, doit être le coeur de toute action en matière de sécurité au plus près des territoires. Merci. La parole est maintenant notre collègue Yvon Collin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre le 1er ministre à la refonte de la carte des zones défavorisées, je suis, on en parle souvent, trop souvent d'ailleurs mobilise encore aujourd'hui très fortement les agriculteurs dans de nombreux territoires en particulier, en Occitanie, la situation est tendue, très tendu, vous connaissez les points de blocage, les barrages qui paralysent la circulation et les activités économiques en Tarn-et-Garonne, dans le Gers ou encore en Haute-Garonne, mais les agriculteurs continuent de manifester à juste titre leur colère contre le zonage qui va plonger, beaucoup d'entre eux dans la difficulté, pour ne pas dire dans la désespérance : ont-ils besoin de cela dans un contexte où bien d'autres aléas climatiques, sanitaires ou de volatilité des prix bouche bien souvent leur horizon les mois prochains, le mois prochain la carte définitive devra remonter à Bruxelles il y a donc urgence monsieur le 1er Ministre urgence à répondre aux appels de la profession agricole qui demandent le maintien des aides européennes, dans les zones qui, bien que hors montagne en tout du handicap naturel cultiver des Descôteaux rugueux du Quercy, ou des Corbières, reste aujourd'hui comme hier, alors pourquoi changer les règles, il ne faut pas abandonner les hommes et les femmes qui s'y investissent et qui s'y accrochent courageusement depuis toujours car leur activité demeure bien souvent le seul pivot de l'économie locale, alors Monsieur le 1er ministre dans ces conditions, je vous demande de continuer à entendre les agriculteurs et dites-nous comment vous allez porter un projet équitable auprès de la Commission européenne, je vous remercie de voir répond. Bonjour, répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation Stéphane Travert, Monsieur le Ministre, pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Colin je n'ignore rien de la difficulté que traversent les agriculteurs dans ce dossier, je n'ignore rien des inquiétudes qui sont les leurs sur satisfaction des zones défavorisées et aujourd'hui tout le gouvernement et moi en particulier, nous sommes totalement mobilisé pour essayer de trouver des solutions, cette carte, monsieur le sénateur, vous la connaissez, elle a été édifié en 1976 et depuis 1976 la cartographie de la France a évolué, elle a changé et l'Europe depuis une dizaine d'années nous impose de changer cette cartographie et de la réviser ce que d'autres majorité n'ont jamais fait jusque-là et c'est nous aujourd'hui qui prenons la responsabilité de proposer ce nouveau zonage et je sais quelles sont les difficultés, quelles sont les attentes notamment dans votre territoire et j'ai reçu personnellement la semaine dernière, des délégations d'organisations syndicales d'agriculteurs de producteurs inquiets et légitimement inquiets et nous avons essayé de trouver des solutions, nous allons essayer aussi d'accompagner parce que je ne veux te je veux tenir ici un langage de vérité monsieur le sénateur, il serait absurde de dire que tout le monde va rester dans le zonage, il y a des communes qui sortiront et celle-là, il faudra les accompagner et le gouvernement, c'est le gouvernement pardon sera totalement mobilisés pour accompagner ces producteurs qui seront sortis de ces zones, mais pour ce qui concerne votre territoire, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de concerter carte concertation et ce travail que nous menons finement pour affiner les critères qui soient les plus justes, les plus robustes et qu'il soit aussi est plus soutenable financièrement, nous amène à penser que nous pourrons ensemble trouver un certain nombre de solutions concertation équilibre équitable c'est ce ce mode de travail que je souhaite employer pour cette révision des zones défavorisées, j'entends la colère des agriculteurs nous avons demain une réunion importante avec eux vendredi matin, un comité national, j'espère que, ensemble, nous pourrons trouver des solutions pérennes pour la sauvegarde de nos de de notre Patrimoine, la sauvegarde de notre élevage et l'image de la ferme France merci monsieur le sénateur. Merci monsieur Collin non. Oui, merci, monsieur le ministre, j'ai bien compris votre réponse vous souhaitez la concertation, mais sachez que les agriculteurs de ces régions ne se contenteront pas de vagues promesses, j'ai bien compris que vous essayez de compenser, mais il faudra des promesses fermes, qu'elle soit vraiment et j'espère que vous y parviendrez merci. La parole est maintenant le pré-collègue Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen écologistes 2 minutes. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues monsieur le 1er ministre il y a quelques jours, votre gouvernement a annoncé une refonte complète de la fonction publique et du statut de ces agents, le tout accompagné de ce qu'on appellerait dans le secteur privé, un plan social, vous avez déclaré à cette occasion, je cite : avoir conscience qu'il faut parfois bousculer les équilibres, les syndicats dénoncent le fait que ces annonces soient faites sans discussion préalable avec les organisations syndicales et sans attendre la fin de la consultation qui a été lancée, fin de citation monsieur le 1er ministre derrière la brutalité de votre démarche, pourriez-vous préciser devant la représentation nationale vous intentions véritables. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'action des comptes publics, monsieur Olivier Dussopt. nous avons effectivement tenu un comité interministériel de transformation public jeudi dernier, le 1er ministre a annoncé 4 orientations : la première, ses orientations concernant le recrutement dans la fonction publique, avec la volonté de mener une concertation sur les possibilités, les conditions dans lesquelles les possibilités d'avoir recours aux contrats pourraient être élargis et le 1er ministre a dit lui-même dans son intervention, comme le président de la République le lendemain que cela ne signifiait pas la remise en cause du statut auquel les uns et les autres sommes attachés le 2ème axe tient au dialogue social, avec la volonté de de le simplifier le 3ème axe tient à la question des rémunérations avec la volonté là aussi de tenir compte de l'individualisation des parcours de l'implication des uns et des autres, et si je veux, si je peux me permet dans la droite ligne de ce qui a été déjà mises en place avec le depuis 2014 même si seulement 10 pourcent des agents de l'État sont aujourd'hui dans le cadre du Ritz, c'est en terme de régime indemnitaire et puis nous voulons aussi travailler sur la question des mobilités, l'évolution des carrières, ça nécessite de travailler sur la formation des agents, ça nécessite de travailler ensemble avec les organisations syndicales sur les conditions dans lesquelles la carrière se déroule et ça nécessite de penser les mobilités, j'ai dit tout à l'heure, en réponse à la question de la sénatrice Maryvonne Blondin, il y a un certain nombre d'établissements publics qui, parce que nous l'aurions décidé parce que ça serait utile pourrait être amené à être fusionné il y a des métiers de la fonction publique qui, avec l'évolution des technologies peuvent perdent leur intérêt aujourd'hui, non pas que celles et ceux qui lui s'exerce le font mal, mais parce que les technologies deviennent aujourd'hui plus performante pour ces agents-là et uniquement ces agents-là, nous voulons proposer une possibilité supplémentaire, le statut leur garantit un droit au classement ce droit sera maintenue, mais nous pouvons aussi imaginer que certains d'entre eux veulent saisir cette opportunité, qu'elle soit subi ou demander provoquer pour aller vers le secteur privé et notre responsabilité c'est aussi les accompagner : c'est dans ce cadre-là, nous voulons avoir une discussion avec les organisations syndicales pendant toute l'année, qui viennent vous voir ensemble comment appelant départs volontaires pourraient être mises en place uniquement sur les secteurs concernés, ça j'ai pas d'un plan général, je le répète, nous nous à nous à nous n'allons pas nous adresser à l'ensemble des agents publics conclave qui va partir mais simplement à ses agents et en les accompagnant du mieux possible. Merci, Monsieur Bocquet. Oui, ce ministre j'entends votre réponse pour la 2ème fois et je suis au regret de vous dire que vous m'avez toujours pas convaincu au moment où s'expriment très clairement dans notre pays, le mal-être des agents publics dans les centres de détention, les tribunaux les Epad les hôpitaux, les établissements scolaires aujourd'hui même vous annoncez vouloir supprimer 120000 emplois de fonctionnaires qui viennent après des dizaines de milliers de suppressions intervenues ces dernières années sous les gouvernements successifs nos concitoyens expriment malgré les difficultés parfois vécue sur le terrain leur profonde attachement au service public, notre pays non pas attachement à un totem, mais comme la garantie d'égalité d'accès aux fonctions que ses services assume la fonction publique, c'est l'un des piliers de notre République nous pensons pour notre part que ce ne sont pas moins de service public, il faut mais au contraire de nouveaux services comme la petite enfance ou le logement, monsieur le 1er ministre beaucoup pensent comme nous que le marché ne peut pas et ne doit pas être la règle absolue dans la gestion de notre République. La parole est maintenant notre collègue Laurent du plomb pour le groupe, les républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Monsieur le 1er ministre monsieur le 1er ministre ma question parle donc loin de l'avenir d'une filière et de l'avenir de nos territoires, ma question parle de confiance que le président de la République prétendait à Rungis vouloir recréer la confiance dans nos territoires, la confiance avec les consommateurs et les citoyens, comme il l'a dit, or cette confiance, il a rompu lors de ses voeux au monde agricole où il annonça contrairement à Rungis, qu'il était favorable à la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, il le confirme d'ailleurs le 2 septembre à son homologue argentin, il ne faut pas avoir peur de cette ouverture au monde, précise le président de la République, ce n'est pas d'ouverture dont ont peur, les éleveurs, c'est pour la survie de leur exploitation, qu'ils ont peur, c'est pour la sécurité alimentaire pour la pérennité de leur emploi pour l'avenir de nos campagnes, que les Français, en raison aussi d'avoir peur, alors Monsieur le 1er Ministre ma question est simple : avez-vous suffisamment évaluer les effets de la signature d'untel accords. Bon vous répondent : la parole est au secrétaire d'État. Près du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoine monsieur pour 2 minutes. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, je crois que nous avons ici en commun effectivement sur tous les bancs et sur les bancs du gouvernement aussi, la volonté de défendre nos terroirs nos producteurs celles et ceux qui font gagner la France parce que, il faut le dire. Le monde agricole est bénéficiaire dans le commerce extérieur français et c'est grâce à cette excellence et bien que nous rayonnant alors s'agissant, s'agissant du maire et continuent à être mobilisés pour défendre, là aussi, un certain nombre d'intérêts le 1er ministre a reçu il y a quelques jours, Ossétie à Malmström la commissaire pour rappeler un certain nombre de lignes rouges, nous avons à Buenos-Aires et Jean Bizet en est témoin, puisqu'il était là, réactiver une coalition de 11 États-membres qui souhaitent un respect ferme d'un certain nombre de sensibilité agricole et naturellement la France continuera à être intraitable en matière, par exemple, hé bien de sécurité sanitaire en matière tout simplement de contingents pour faire en sorte que le maximum de ces contingents, soit on Hilton pour que véritablement cette ambition de qualité puisque la qualité c'est véritablement ce qui caractérise nos producteurs alors sachez-le dès que le président de la République ou un membre du gouvernement, se rend à l'étranger, nous sommes également là pour essayer de lever un certain nombre de barrières à l'accès, c'est le cas lorsque le président de la République s'est rendu en Chine de nouveaux débouchés souffre à la filière bovine, d'ici quelques mois en Irak au mois de décembre, enfin, a été levé l'embargo sur la volaille, bref, nous partageons cette même ambition et sachez que nous avons des intérêts défensifs, nous avons également des intérêts offensifs et nos producteurs de vins et spiritueux, effectivement, Monsieur le Président, Patriat nos producteurs de lait et je sais que vous êtes particulièrement impliqué dans cette filière au sein du grand Massif Central, hé bien ces producteurs attendent également un certain nombre de débouchés grâce à ces accords, donc il nous revient d'être à la fois en défense, mais à la fois aussi à l'offensive. l'offensive. Du plomb, monsieur le Ministre, cet accord prévoit un accès au marché européen de plus de 100000 tonnes de viande sud- américaine des tonnes de viande au standard radicalement opposée aux viandes françaises des viandes provenant d'animaux ou la traçabilité individuelle ou les principes du bien-être animal ne sont pas obligatoires ou les additifs alimentaires dans la ration des bovins sont autorisés, alors qu'ils sont interdits chez nous et que dire du Brésil, englué dans une affaire de corruption concernant un vaste réseau de commercialisation de viande avariée par ailleurs la viande sud-américaine serait commercialisé à 8,6 euros alors que le même kilo produit en Europe est à 13,7 euros les conséquences d'un thé à la Corse seront donc catastrophique pour l'élevage français, alors Monsieur le ministre, ce n'est pas comme cela que vont forer le printemps en agriculture, ce n'est pas non plus comme cela que vous donnerez le courage tant décrit dans le nième campagne de communication du président de la République, par contre, c'est comme cela que vous donnez, conclut l'impression que votre gouvernement fait le contraire de ce qu'il a dit.

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des Comptes publics les transformations qui traversent notre société, notre économie ne laisse pas la fonction publique, à l'abri et les fonctionnaires sont en première ligne en fait pour faire face aux mutations économiques numérique démographique qui affecte toutes les sociétés du monde occidental, les fonctionnaires sont d'ailleurs les premiers conscient et les premiers demandeurs des transformations, je ne crois pas que la transformation de l'action de l'État va contre l'amélioration des conditions de travail au contraire redonner du sens à l'action de l'État s'est aussi améliorer et transformer les conditions de travail des des fonctionnaires, prenons un exemple : l'seulement 5 pourcent de fonctionnaires changent chaque année d'employeurs publics 0,5 pourcent change de fonction publique, donner des moyens, c'est bien sûr important fixer des caps pour construire des carrières, c'était extrêmement important également dans dans le monde public à l'approche quantitative du rabot, il y a une approche qualitative qui est celle de la construction finalement d'une gestion moderne des moderne des ressources humaines dans la fonction publique de l'État, les annonces que vous avez fait seront aussi des leviers du changement, monsieur le Ministre, comment allez-vous associez le Sénat, la Chambre des territoires qui est aussi intéressé par ces sujets parce que il existe notamment les cadres d'emploi dans la dans la et collectivités territoriales, qui sont des bons outils, quel est le calendrier, quelle est la modalité de cette concertation qui concerne bien sûr les organisations syndicales mais également tous les employeurs publics, je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Bargeton, merci pour votre question qui me permet de revenir sur la manière dont nous allons conduire la transformation et la modernisation de la fonction publique, je l'ai dit tout à l'heure, en réponse à de premières questions, nous avons 4 objectifs : améliorer le dialogue social et il faut avoir en tête qu'il existe 22000 instances représentatives du personnel, de dialogue social et que ça participe à une complexité nous voulons diversifier les modes de recrutement pour garantir l'égalité d'accès pour garantir la diversité dans l'accès à la fonction publique et ça renvoie aussi au débat sur la question des contractuels, nous voulons mieux accompagner la carrière chacun des agents par la formation par l'immobilité et j'ai eu l'occasion de préciser nos intentions tant de mobilité entre les versants que de mobilité vers quand c'est nécessaire quand c'est demandé ces souhaité dans le secteur privé et puis nous voulons aussi travailler sur les questions relatives à la rémunération, nous avons une chance, c'est d'avoir un an devant nous un an de débats un an de dialogue dès la semaine prochaine, désormais des rencontre bilatérale sont organisées entre le ministre de l'action des comptes publics et moi-même, d'une part, et les organisations syndicales, mais aussi le collège, le collège des employeurs pour arrêter le calendrier arrêté la méthode du débat et voir comment nous pouvons avancer ensemble cette réforme peut susciter des interrogations, des inquiétudes et c'est légitime de la part des agents publics, c'est légitime, parce que depuis plus de 20 ans, chaque réforme de la fonction publique, chaque réforme de l'État n'a été abordé que sous un angle budgétaire jamais en interrogeant l'émission jamais en interrogeant les métiers jamais, on se pose souvent la question de l'intérêt des fonctions exercées par telle ou telle ajoute cette année débat nous permettent de répondre à cela et puis par ailleurs, nous ne venons pas uniquement changer la manière de travailler ou la manière dont tout notre administration nous venons avec des moyens parce que nous considérons que pour moderniser, il faut savoir investir, investir dans la formation et nous publierons prochainement le schéma national de la formation professionnelle et nous pouvons nous appuyer sur un milliard et demi d'euros du grand plan d'investissements d'avenir, que le président de la République et le 1er ministre ont orienté vers la formation des agents publics nous venons aussi avec un fond de 700 millions d'euros à l'échelle du quinquennat pour financer les investissements dont ont besoin les administrations pour participer à leur modernisation, soyez assuré que l'Assemblée nationale, quand le Parlement seront largement associés à ces travaux.

Monsieur le président, ma question s'adresse au Monsieur le 1er Ministre Monsieur le 1er ministre les décisions que vous avez prise avec votre gouvernement ne sont pas comprise par les Français, elles ne peuvent pas l'être, car elles ne sont pas justes, il n'est pas juste en effet de rogner le pouvoir d'achat des retraités qui ont travaillé toute leur vie, dont une partie, bien au-delà des 35 heures, il n'est pas juste de les désigner comme des nantis, il n'est pas juste de baisser massivement les impôts pour une petite catégorie de Français les plus riches et de transférer ce coup sur ce dont les revenus sont les plus modestes et dont certains sont exonérés de taxe d'habitation, de longue date mais sans toujours redevables de la taxe foncière comme les retraités, agriculteurs ou ceux qui ont économisé des années durant pour acquérir leur logement, il n'est pas juste enfin d'annoncer une hausse du pouvoir d'achat au travers d'une baisse des charges et de la taxe d'habitation, alors que la fiche de paye, est venu surfer à une myriade d'augmentation, essence, gaz sont à l'hôpital en 2018 vous voulait créer 9 taxes nouvelles et ce sont 4,5 milliards d'euros supplémentaires qui seront prélevés sur les ménages, ne pensez-vous pas monsieur le 1er Ministre que vous avez sous-estimé le fait que les Français sont contraints de faire leurs comptes et qui savent compter. Bon vous répondent : la parole est au secrétaire d'État. Olivier Dussopt. Madame, monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, quelques mots d'abord, Madame la sénatrice pour d'abord confirmer 2 choses : la première chose, c'est que nous allons procéder au dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des ménages et ce dégrèvement sera effective dès le mois de septembre et qu'il permettra d'améliorer le pouvoir d'achat de 80 pourcent des Français avec comme perspective de supprimer totalement la taxe d'habitation à l'horizon 2020, comme l'a dit le président de la République, la 2ème chose pour confirmer, Madame la sénatrice, que l'augmentation de la CSG qui a été votée par le Parlement s'applique aux salariés les 21 millions de salariés mais connaît aussi une compensation par la baisse des cotisations, ce qui se traduit par un gain de pouvoir d'achat s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics mais connaît une compensation qui permet de garantir le pouvoir d'achat, et c'est un engagement qui est pris qui nu s'applique aussi aux retraités, dès lors que la retraite par personne et supérieures à 1200 euros et au-delà, beaucoup d'entre eux verront cette augmentation de CSG compensée par la baisse de la taxe d'habitation, madame la sénatrice permettez-moi cependant d'être dubitatif d'être dubitatif à écouter votre question tout à l'heure dans votre question vous avez accusé le gouvernement d'être responsable d'une hausse que vous avez des impôts que vous avez qualifié de massive, si ma mémoire ne fait pas défaut vous avez soutenu un candidat à l'élection présidentielle qui, 5 ans auparavant, avait été au 1er Premier ministre et qui, pendant les 5 ans pendant lesquels il a été 1er ministre a augmenté les impôts de 25 milliards

que vous êtes dans la position qui est la vôtre aujourd'hui vous devriez peut-être faire preuve d'un peu plus de retenue et d'un peu moins posture. Pascal. Et à 41 secondes. Monsieur le ministre, je le rappelle, votre gouvernement ne s'adresse qu'à une petite partie des Français ce Attila vie sourit réformer notre pays signifie baisser l'espérer lavement obligatoire

vous avez simplement transférer des charges des uns, les plus riches vers les autres, les Français ne s'y sont pas trompés, dimanche dernier, d'ailleurs, lors des élections législatives partielles.

Merci, la parole est maintenant. à notre collègue Maurice anti. Pour le groupe socialiste et. Républicain, vous avez la parole, mon cher collègue, pour 2000. Ma question s'adresse à Madame la ministre des solidarités, de la santé, la presse locale de Martinique et de Guadeloupe s'est fait l'écho depuis le 26 décembre dernier de vives préoccupations relatives à une augmentation des limites maximales de résidus dite LMR de chlordécone intervenu dans la plus totale opacité en 2013 cette augmentation apparaît ailleurs été confirmée par le ministère de l'agriculture en septembre dernier, l'étude des Canaries affirme clairement que 90 pourcent de la population martiniquaise a du chlordécone dans le sang, soit 9 martiniquais sur 10 l'Kawhi : prostate, quant à elle, a révélé le lien significatif qui existent entre les cancers de la prostate et le chlordécone notre il détient le triste record mondial du nombre d'hommes atteints de cette pathologie, son incidence et sa mortalité autant en Guadeloupe qu'en Martinique, ils sont plus élevés que l'Hexagone, il en est de même pour le taux d'accouchements prématurés et les cas de puberté précoce, une fois et demie plus élevé que dans l'hexagone depuis 2008, la ligne de conduite adoptée par l'État était celle de la diminution de l'Exposition des populations au chlordécone alors je vous le demande, Madame la Ministre, cette logique est-elle en train de s'inverser, pouvant nous décemment et en toute honnêteté inciter nos habitants consommer de viande présentant des valeurs toxicologiques de référence 5 à 10 fois plus élevé qu'avant 2013, pourquoi ne pas introduire une demande auprès de l'Union européenne afin de revenir aux normes de 2008, beaucoup plus protectrice pour nos populations, par ailleurs, vous avez plusieurs fois affirmé ces dernières semaines que le lien entre le chlordécone et le cancer n'étaient pas clairement établies, due notamment au manque d'information sur le sujet, dès lors, ne serait-il pas judicieux de relancer l'étude Maddie enfin le Centre international de recherche sur le cancer a classé le chlordécone comme cancérogènes possibles pour l'homme en 1979 mais il n'a jamais été reconsidérée, en dépit de nombreuses informations acquises depuis cette date au regard de cesser les et au vu des résultats de l'étude car prostate le gouvernement entend-il saisir légitimement le CIRC pour un éventuel reclassements du chlordécone comme cancérogènes probables ou cancérogène cancérogène certain, j'espère, Madame la Ministre, que vos réponses seront à la hauteur des attentes des Martiniquais et des Guadeloupéens qui nous regardent avec inquiétude, je vous remercie.

je tiens en 1er lieu à assurer à tous nos compatriotes des Antilles plein engagement et de suivi du gouvernement sur le sujet du chlordécone ou savez j'ai déjà travaillé avant d'être ministre et je continuerai en tant que ministre, il est impératif d'avancer sur ce sujet, de réduire l'Exposition des Antilles, alors vous avez des études scientifiques sont en cours dans le cadre du plan de quand le chlordécone, avec notamment un recueil de données épidémiologiques sur les femmes, les femmes enceintes, les enfants, les personnes et qui vont permettent de mieux identifier les effets à long terme parce que vous le savez, seuls les effets à court terme sont réellement bien connu, il nous faut en effet aller plus loin dans les connaissances scientifiques et vous le savez, également d'un point de vue méthodologique, ces études sont compliquées, car il s'agit d'Exposition très ancienne et qui touche l'ensemble de la population, à des degrés variables, je me suis engagé engager une nouvelle cartographie des sols pollués aura lieu en 2018 concernant les services alimentaires des seuils définis en 2013 au niveau européen ne concerne pas tous les produits, mais uniquement les produits carnés mon ministère est très mobilisée, comme le ministère des Outre-Mer et celui de l'Agriculture et celui de l'écologie, de l'écologie, et je vous l'avez déjà dit lors d'une précédente séance que nous avons sollicité la Commission européenne afin de clarifier la directive sur les seuils concernant les denrées alimentaires, mais je tiens aussi à rassurer la population en 2000 659 prélèvements ont été faits en Guadeloupe 875 en Martinique sur ces produits qui ont révélé un taux de conformité de 98 pourcent alors, Monsieur le Sénateur, je souhaite que nous avancions ensemble sur ce sujet, je peux vous annoncer qu'une réunion sera très prochainement organisée au ministère des Outre-mer, avec l'ensemble des élus de la Martinique et Édouard de la Guadeloupe et les différents ministères concernés afin de faire la transparence sur ce sujet et de décider ensemble de la stratégie qu'il convient de mettre en place, je vous remercie. Si le 1er Ministre Mesdames et messieurs les Ministres, merci notre prochaine séance de questions d'actualité au gouvernement auront lieu le jeudi 15 février je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 17 heures 50 pour la suite du projet de loi relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, la séance est suspendue.

La séance est repris les conclusions de la conférence des présidents réunis ce jour et complétant l'ordre du jour établi par la réunion de la conférence des présidents du 31 janvier 2018 sont consultables sur le site du Sénat, elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observation, d'ici la fin de la séance, j'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure a été publié cette candidature sera ratifié si la présidence n'a pas aussi d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. La parole est maintenant à monsieur Jean-Louis Masson pour un rappel au règlement. Monsieur le président, nous avons il y a peu de temps, modifié le règlement du Sénat pour introduire le système d'examen accéléré des lois afin d'y accélérer des lois qui consiste à faire étudier les lois en commission et en fait ensuite s'éloigne ne donne plus lieu à un vrai débat, il y a plus de possibilité d'amendement, alors on nous avait dit à l'époque que une fallait pas s'en faire, seules les lois peu importante tout à fait accessoire serait l'objet de cette procédure et je suis donc très surpris que sur une loi importante et hier, elle est tellement importante que c'était initialement la seule loi pour laquelle le Sénat avait prévu d'avoir un scrutin public officiel officiel je dirais au cours du 1er trimestre après il y a eu un 2ème jeu on a intégré la loi sur la qualité, la Nouvelle-Calédonie mais donc il y a, c'est l'une des 2 lois les plus importantes, puisque ce sont, c'est l'une des 2 lois où il y a un scrutin public, je suis quand même très surpris que disons on on est enlevé, on est passé, un bloc d'articles de cette loi dans le système des débats accélérés, je crois que c'est vraiment pas bon, où la loi est importante, il faut qu'il y a un vrai débat dans le Sénat en séance publique du Sénat, où la loi est pas importante, mais on se demande dans ces conditions, pour quelles raisons il y a un scrutin public, il est évident que tout le monde considère que cette loi est importante

alors il semblerait que un groupe politique a demandé que certains articles soit sorti il y a eu une petite amélioration mais j'ai bien une petite amélioration et nous sénateur non inscrit, on ne peut pas s'opposer au système puisque vous le savez, seuls les présidents de groupes peuvent s'opposer à ce que telle ou telle disposition soit soumise au scrutin sans ou vote sans débat, c'est-à-dire celui dans un système où le débat public en sciences du sénat ne sert strictement plus à rien, alors moi je voudrais et j'aurais souhaité qu'à l'avenir, seuls les lois tout à fait marginal, comme on l'avait dit au départ : soit l'objet de ce système abrégé d'examen des taxes. Acte et donner de votre rappel au règlement, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 je vous rappelle que la discussion générale et. Closer nous passons à la discussion du texte de la Commission à l'article 1er j'ai une demande de parole de monsieur Assouline. Oui, merci Monsieur le Président Madame Monsieur le ministre des chers collègues, si je prends la parole là c'est parce que par une un artifice de procédure, le sujet important partagés sur ces bancs des retransmissions télévisées des Jeux olympiques, n'a pas, ne peut pas arriver par voie d'amendement, puisque l'article 40 a été évoquée, je veux dire que je respecte complètement la constitution mais que c'est une interprétation puisque, à l'Assemblée nationale qui est régi par la même constitution de la République, ces amendements ont pu arriver à la discussion, donc on peut être pour on peut être content, ce que je défends ou tels amendements mais on ne peut pas dire à discussion parce que même si j'ai entendu la ministre ces amendements pourraient provoquer un contentieux avec le propriétaire des droits de télévision qui est Discovery en 2024, on pourra discuter au budget si l'État veut mettre la main à la poche pour les associations et les collectivités publiques qui veulent être exonérés des droits de retransmission d'un événement majeur qui va avoir lieu sur notre territoire, et c'est ça le sujet important, je veux plaider pour quelque chose qui est lié à ma forte conviction que c'est une chance inouïe que nous ayons pu gagner l'organisation des Jeux, que c'est en même temps un pari et le pari, c'est le pari de l'adhésion populaire jusqu'au bout vous savez bien qu'elle n'est pas acquise, elle est acquise pour l'instant, mais plus on va acheminer plus parce que les financements sont importants parce que beaucoup d'argent va jeu plus il peut y avoir des regards dubitatif ou critique ce que je ne veux pas et c'est pas mon état d'esprit même mon état d'esprit et l'inverse et aujourd'hui les droits achetés par Discovery sont revendus si cher que probablement le service public français ne pourra pas, alors que c'est sa mission essentielle parce que le sport c'est l'événement fédérateur par excellence qui seront en Direct à la télévision alors que beaucoup de choses qui était à la télévision d'voix plus en Direct et ne permettent plus de fédérer et donc c'est un enjeu majeur mais exonérer les petites associations, les collectivités locales qui vont devoir payer des droits d'auteur et des droits de retransmission à ce moment-là, c'est quelque chose sur lequel la représentation nationale a son mot à dire, parce que nous voulons qu'il y a cette adhésion populaire, nous voulons que tout le monde soit au rendez-vous, pas seulement ceux qui ont les moyens, je finis en disant que ce débat devrait avoir lieu, d'une façon ou d'une autre, il ne peut pas esquiver, on veut que le gouvernement prenne à bras le corps, cela et c'est pas par l'article 40 qu'on règle le problème. Je suis saisi de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 1er numéro 40, défendu par monsieur Monsieur le Président, Madame, Madame la ministre, en effet, l'objet de cet amendement du maire au 40 vise à reconnaître comme organisateur des Jeux olympiques et paralympiques 2024 les filiales du CIO. Le comité international olympique, telles que la société audiovisuelle Olympic Broadcasting Services de diffusion des Jeux alors effectivement la la formulation n'est pas une formulation limitative c'est une illustration à travers cette entreprise, cette société n'oublions pas que nous sommes en 2018 que les JO de 2 de Paris sont annoncées pour 2024 qui peut se passer beaucoup de choses d'ici 2024, notamment en terme de création de 2 filiales de filiales de filières à l'intérieur du mouvement sportif et y compris à l'intérieur du mouvement olympique, je prends un seul exemple : je dirais national, c'est ce qui se passe à l'intérieur du football professionnel puisque est envisagée là depuis quelques jours, la création d'une société chargée du développement économique du football professionnel, les clubs professionnels en serait actionnaire et cette société serait notamment chargé de négocier les droits de retransmission télévisée, donc c'est l'exemple type d'une mutation qui est en cours concernant le mouvement sportif et mutations parmi beaucoup d'autres il est bénéfique dans que derrière ça t'amendements il y a des enjeux financiers importants, notamment en terme de fiscalité, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il était important de préciser qui était organisateur des jeux olympiques et paralympiques.

les organes, a indiqué son le COJO, le CIO et le comité international paralympique il établit aussi un régime dérogatoire du droit commun des autorisations de fédérations sportives lors des compétitions cet article semble être trop restrictif comme cela nous a été indiqué par par là lors des auditions par notre commission cette vision est restrictif, car d'autres organes sont considérés comme organisateurs comme la Fédération internationale certaines filiales en vertu du contrat de ville hôte et je pense qu'il faut qu'on cite tiennent les signataires ont reconnu l'importance de garantir la diffusion et la couverture médiatique, mais plus complète des jeux et la plus large audience possible des jeux et accepte de se fait de coopérer avec la Syrie au diffuseur hôte des Jeux au il convient donc pour permettre au PS de l'exploitation des jeux d'inclure Bouygues dans la définition d'organisateurs, c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement qui reconnaît aux filières des trois organise précités, le statut d'organisateur. Merci, quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements. Merci Monsieur le Président, alors le CIO a évoqué la semaine dernière la nécessité de mentionner les filiales du CIO justement afin de préserver le statut de l'Olympique Broadcasting System le BS toutefois : nous n'avons aucune analyse juridique qui est venu appuyer cette nécessité et le caractère très générale de cette mention non limitative des filiales pose problème, notre commission souhaite connaître l'avis du gouvernement sur l'impact juridique de cette disposition, et dans l'attente de cet avis, nous donnons un avis de sagesse. Messieurs les sénateurs. Votre amendement vise à reconnaître la qualité d'organisateur aux filiales du CIO en particulier à la filiale UBS qui exploite la diffusion audiovisuelle des Jeux, conformément aux dispositions du code du sport, la qualité d'organisateur emporte attribution d'un droit d'exploitation au profit de la structure qui la détient, rien n'interdit donc au CIO de confier la gestion de ces droits à une de ses filiales en fait de villes hôtes prévoit en effet que le CIO peut céder ses droits à tous partenaires notamment le diffuseur des Jeux. Il n'y a pas de notre responsabilité de forcer la main au CIO. Si votre demande sous-jacente concerne la fiscalité applicable à au BS il il sera nécessaire d'en rediscuter en prévision de l'de l'examen du d'une loi de finances à venir comme l'accepter le COJO par son directeur général Étienne Thobois votre amendement n'est donc pas nécessaire et j'y suis défavorable. Les Donc ce qu'il y a, dès l'explication de vote Monsieur Samin. Madame la ministre, vous venez de nous indiquer que qui est donc une filiale de du CIO donc cette filiale et est considérée automatiquement, vous venez de le rappeler, comme organisateur par la rédaction de l'article 1 ce qui répondrait à l'objet de de mon amendement de notre amendement donc cependant vous fait aussi état d'une ouverture de statut d'organisation à d'autres filiales, et vous avez rappelé adopte organisations qui sont aussi ralliés rattaché aussi

qu'pourrait tout comme obèse donc se prévaloir du statut d'organisateur, donc il faudrait que soit que tout soit reconnu comme organisateur, niveau de ses filiales, soit il faut clarifier votre position sur l'Euro baisse. Monsieur Masson. Oui Monsieur Président moi je, je considère que, actuellement, je olympique, on tombe dans un système où l'argent est roi et en fait, c'est encore une affaire financière derrière tout ça il y a encore des, des perspectives financières et moi je crois que on assiste globalement à une dénaturation du sport avec des sommes de plus en plus, de plus en plus importante en jeu, ce qui fait que tout le monde se bat pour bénéficier des facilités financières, fiscales et autres, je, je serais plutôt partisan de surseoir actuellement il attendent la loi de finances sur qui qui est prévu et je la voterai pas cette loi de finances Fathi à ce niveau-là, parce que je suis contre ce système mais indépendamment de ça, moi je crois qu'il vaut mieux attendre c'est prématuré, décidé aujourd'hui sur ces amendements. Madame la ministre, vous souhaitez prendre part. Oui, je voulais juste redire que c'est le droit du CO2, de redéfinir à qui ont donné droit pour les filiales mais je suis aussi d'accord avec avec vous pour, pour attendre en fait la loi. Donc je reste sur la position. de rédacteur de cet amendement, de bien vouloir et retirer, sinon je serais obligé de donner également un avis défavorable. Alors que souhaite faire les auteurs des amendements. J'ai nous. Oui, je crois qu'avec mon collègue Michel Sapin la volonté d'une volonté de de clarification, une volonté d'anticipation et c'est la raison pour laquelle ce qui concerne je maintiens mon amendement. Alors, le 1er maintenu le second. Pareil Monsieur le le président, les explications aussi chiffon chaque fois reportées les décisions une éventuelle proposition de loi aujourd'hui, on est quand même dans dans beaucoup d'incertitudes, je pense que les banques que ceux qui ont l'organisation alors notre collègue par de de fortes sommes d'argent oui. Mais aujourd'hui 97 pourcent de l'organisation des Jeux olympiques et porté par le privé, donc il faut sécuriser aussi ceux qui aujourd'hui vont investir dans l'organisation des Jeux olympiques, c'est pas de l'argent public, c'est essentiellement de l'argent privé et donc on peut pas nos membres et à des partenaires privés de venir soutenir et financer les Jeux olympiques, sans avoir des garanties de protection c'est vrai aussi pour les diffuseurs, donc je maintiens, c'est mon amendement. Plus de demandes d'explications de vote, donc je vais mettre aux voix, ces 2 amendements avec 2 avis défavorables commission et gouvernement sur le 1er amendement numéro 40 qui vote pour.

Merci qui vote contre. L'amendement est adopté et l'autre tombe. Je vous en prie. Je voudrais profiter de mon explication de de vote sur l'article nous allons voter pour joindre ma voix à celle de David Assouline qui a saisi cette occasion pour attirer l'attention, je l'ai dit déjà en commission sur ce que je considère effectivement comme un abus de procédure, la manière dont ont été écartés Les et les amendements concernant les retransmissions de droit au prétexte de l'article 40 alors que ça n'a pas été le cas à l'Assemblée nationale et je pense que ça pose un problème sérieux qu'il faudra débattre de l'utilisation abusive de l'article 40. Pas d'autres demandes d'explications de vote sur l'article 1er, je n'en vois pas je mais on voit cette article qui vote pour.

Merci Monsieur le Président, Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mais, chers collègues, c'est un amendement entend assurer le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité national olympique et sportif français, le comité international travaille actuellement sur cette question de l'égalité femme et attend les recommandations de son groupe de travail dédié, la France pourrait être exemplaire en prenant les devants au niveau au niveau du comité national olympique et sportif français, grande cause nationale du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes doit passer par l'adoption de mesures fortes, c'est pourquoi cet amendement propose d'insérer un article additionnel ainsi rédigé après l'article 1er. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur cet amendement. L'objet de cet amendement, présenté par Colette Mélot et pour la parité au sein du CNRS chef donc cet objectif de parité au sein des organes de direction du sport est légitime car le sport concerne autant les femmes que les hommes et par ailleurs le sport féminin souffre d'un déficit d'Exposition

faut-il anticiper sur leur conclusion modifié en modifiant la loi dès maintenant une question et nous souhaitons avoir l'avis du gouvernement sur ce sujet, donc c'est un avis de sagesse de la part de la Commission. Le ministre pour les pays, gouvernement.

une égalité de représentation entre les femmes et les hommes, notamment dans ses instances dirigeantes, vous avez raison il paraît aujourd'hui pertinent que le CNO SF qui représente le mouvement sportif, s'engage dans cette évolution, d'ailleurs, il semble aujourd'hui prêt à se réformer, a exprimé sa volonté de vouloir travailler en ce sens avec nous pour autant la loi olympique et paralympique n'est pas le bon vecteur car ce sujet dépasse très largement le cadre des Jeux, il me semble qu'un sujet de cette importance nécessite un diagnostic affirmé. Néanmoins, en vous demandant de retirer cet amendement, je m'engage devant le Sénat, à travailler avec vous à parfaire vos intuitions et a présenté un volet relatif à une meilleure représentation des femmes dans le projet de loi, Sport et société que nous porterons devant le Parlement en 2019. Merci, Madame le Ministre, alors une demande de retrait, je reconnais que faites-vous. Bon, je vais suivre vous aux préconisations, madame la ministre, je vous fais confiance pour la suite, que vous donnerez à cette requête, parce qu'il me semble que dans la dans le l'article acéré on ne on ne visait qu'à assurer une représentation équilibrée entre les femmes, des hommes et à favoriser la parité demandez pas une parité stricte, est-ce qu'on peut se demander si on ne on ne favoriserait pas le le mouvement en insérant cet cet article dans la loi, se de se demander : mais bon si vous assurer que l'on pourra faire figurer dans un autre projet de loi cette la la parité est une disposition qui peut la favoriser, je vais le retirer, merci.

Je pense que on va demander de retirer pour gagner du temps. C'est pas encore en anglais : d'abord l'avis de la commission ensuite celui du gouvernement. merci Monsieur le Président, alors pour les mêmes raisons, qu'à l'article à l'amendement pardon numéro 19 de Madame Mellow nous donnons un avis de sagesse dans l'attente de l'avis du gouvernement, qui je pense ne va pas varié. Madame ministre.

vous souhaitez reprend de l'amendement, vous exprimer sur Cologne. Son amendement, Monsieur le Président, les 2 amendements 19 et 20 rectifier parce que je pense que nous devons aider le gouvernement nous avons entendu l'engagement de la ministre sur ce point et nous connaissons, il est important de d'avancer et nous le savons bien quand on veut avancer sur ces sujets-là, si jamais le moment donc je pense que c'est important que le Sénat donne un signe en ce sens en soutien à la démarche qui avait été faite par notre collègue, je souhaite que nous puissions nous exprimer sur le 19 rectifier bis, le 20 rectifier bis, si je ne me trompe pas dans la numérotation.

Je vais le mettre aux voix, ne vous inquiétez pas, donc je reprends le 19 rectifier, qui est donc repris par madame de La Gontrie et vous souhaitez vous exprimer en explications de vote, je vous en prie. Merci monsieur le président, je voulais m'exprimer parce que je soutiens la décision que vous ne venez de prendre cher collègue et et au niveau de notre groupe, nous vous suivrons parce que c'est un sujet que nous ne voulons pas encore remettre un an ou 2 ans, Madame la Ministre je merci. Pas d'autres demandes d'explications de vote dans le jeu, mais on voit cette fois-ci.

qui vote contre.

monsieur Savoldelli. Président Madame la la ministre avec une moyenne de 23 équipements sportifs par habitant l'Île-de-France est la région la moins dotée du pays, la Seine-Saint-Denis souffrent tout particulièrement d'un manque avec par exemple un bassin de natation pour 20000 habitants, donc, comment s'étonner dès lors qu'un enfant ces canaux dionysien sur 2 ne sachent pas nager à l'entrée en 6ème c'est à ce titre que notre amendement prévoit la remise par le gouvernement d'un rapport au Parlement pour 2019, un rapport qui puisse pointer précisément les facteurs d'inégalité mais aussi les réponses aux besoins et parce qu'il faut saisir l'occasion des Jeux olympiques de 2024 pour irriguer les associations sportives, il faut saisir cette cette opportunité pour porter une forte ambition de sport pour toutes et tous et c'est le sens de notre amendement c'est justement, rapport à la promotion du sport en banlieue que je voudrais en profiter, Madame la Ministre pour vous rappeler qu'il y a quelques jours, vous avez reçu une belle invitation de la part de l'Union sportive d'Ivry-sur-Seine, c'est un vrai club populaire en Val-de-Marne 41 Discipline 8000 adhérents et celles et ceux qui font vivre le club ce sont des gens qui usent de leur temps, après le travail le dimanche, parfois plusieurs fois par semaine pour faire rêver des gamins pour faire vivre un modèle du sport pour toutes et tous, ils m'ont demandé de relayer leur message issu d'un travail approfondi de leur part sur ce projet de loi l'héritage des Jeux doit devenir revenir au sport associatif, c'est pourquoi je relaie leur invitation ici accepterait-vous Madame la Ministre, de vous rendre à Ivry pour en discuter avec les bénévoles, avec les dirigeants du club pour visiter les infrastructures pour rencontrer aussi ces gamins d'Ivry qui serait fier de discuter avec vous et de donner leur avis sur ce que doivent être ces jeux parce que les champions, on est les champions de demain, ils sont là, ils sont dans tous ses clubs associatifs et j'ai la conviction qu'il n'est pas dans vos intentions de les délaissés, c'est pourquoi je vous confirme avec cette invitation que vous serez la bienvenue à Ivry, parmi ces éducateurs, ces bénévoles et tous ces jeunes merci.

par principe, la commission des lois, et réservé sur les demandes de rapport, c'est un projet de loi qui ne concerne pas directement l'accès à la population de la pratique sportive et, sauf erreur de ma part, le gouvernement a annoncé qu'un projet de loi sur le sport sera bientôt déposé son examen sur le feu, l'occasion d'évoquer ce sujet effectivement qu'il est important de l'égalité à l'accès à la pratique sportive, donc c'est une demande de retrait, à défaut, un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Madame le Ministre. En 1er le merci de l'invitation Monsieur Laurent je viendrai vous voir mais ça ne sera pas une une surprise puisque c'est un département territoire que je connais, donc j'accepte votre invitation, la 2ème des choses effectivement, vous avez dit : le sport est un vecteur incontestable d'de bien être de développement personnel et d'inclusion sociale aussi on va travailler, on a suscité l'activité physique et sportive pour tous pour les femmes comme pour les hommes, les personnes en situation de handicap dans tous les lieux, l'école, l'université, l'entreprise et dans nos administrations dans tous les territoires carencé ruraux et comme urbain les constats en fait sont largement connues mais j'ai souhaité affiner le diagnostic en demandant à France Stratégie de procéder à une revue de littérature pour analyser tous les obstacles qui entravent le développement des activités physiques et sportives, les conclusions du rapport de France Stratégie qui devront constituer une base pour l'élaboration d'une loi dédié sport pour tous en 2019 sont attendus en septembre 2018, elles sont, elles, seront bien bien sûr partagé avec le Parlement, c'est pourquoi je vous demande le retrait de votre amendement merci. Alors, de demandes de retrait souhaite faire l'auteur de l'amendement. Donc, nous allons le monde, j'ai bien entendu votre réponse, Madame la ministre et j'espère que tout ce travail effectivement permettra d'aboutir à un diagnostic partagé, mais nous allons maintenir l'amendement parce que dans ce projet de loi qui est le projet de lancement effectif de l'organisation des Jeux olympiques, cette ambition-là, qui ne figure pas dans le texte actuel explicitement dans le projet, à nos yeux doit y figurer. L'amendement est donc maintenu des demandes d'explications de vote je n'envoie pas je vais mettre aux voix de demandes de retraits ou avis défavorable qui vote pour. Merci qui vote contre. Il n'est pas adoptée à l'article de l'amendement de rectifier bis monsieur ça. Merci Monsieur le Président, cet article vise à consolider la propriété intellectuelle mais symboles olympiques et notamment le terme olympique la rédaction que nous propose à l'Assemblée nationale, aller à l'inverse de ce qui était attendu au lieu d'accroître la protection des termes la protection était restreinte, il s'agissait d'un recul est-ce douaniers des dispositions du contrat de ville hôte, or les propriétés olympiques sont clairement définies par ce dernier, aujourd'hui notre commission et notre rapporteur, ont modifié en partie c'est article la nouvelle écriture assure une meilleure protection dans les domaines commerciaux et promotionnel, cependant elle n'assure pas la protection totale admettent que le terme olympique pourrait faire l'objet d'un usage normal dans la langue de langage commun revient à méconnaître jurisprudence consacrant son caractère de marques notoires. La jurisprudence a en effet admis de manière constante que les termes olympique y compris pris isolé ment est une marque notoire au même titre que je olympique Olympia reconnaître un usage commun viendrait à redire Anne réduire à néant les Zürich prudence existantes et la protection qui est mon amendement a comme effectif de rassurer les partenaires des gens qui vont investir beaucoup d'argent et d'être en phase avec les engagements pris dans le contrat de ville hôte de protection de la marque des droits

Merci Monsieur le Président, à l'amendement de notre collègue Michel Savin, par ailleurs excellent connaisseur du sport répond à une préoccupation très louable, qui consiste à sécuriser les termes propres jeux olympiques pour garantir aux partenaires privés l'exclusivité de l'utilisation des marques olympiques telle est d'ailleurs l'art, l'objet de cet article 2 qui correspond à une demande du CIO et un engagement de la France de la dans le cadre de la candidature de Paris, cependant je me dois de rappeler 3 éléments d'une part le degré de protection dont la jurisprudence de la Cour de cassation fait bénéficier l'ensemble des propriétaires, les olympiques, est très élevé en l'occurrence les marques olympiques sont déjà les seuls à être protégés au niveau législatif dans le code du sport et sont reconnus comme des marques notoires au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle de 1883 en conséquence et comme je l'ai indiqué dans le rapport de la commission, si l'on peut comprendre en termes d'affichage cet article 2 il n'est pas certain qu'ils soient beaucoup plus protecteur que ce qui existait déjà avant, d'autre part, nos collègues des députés ont souhaité préserver la possibilité d'un usage normal de certains termes, il nous faudra parvenir à un accord en CMP pour éviter des délais douloureux pour tous et je suis donc à bien montrer que le Sénat a tenu compte des remarques de l'Assemblée, cet amendement, qui en réalité ne modifie pas réellement le droit serait par contre symboliquement de nature à mal augurer de notre CMP enfin l'adoption de cet amendement serait susceptible de faire courir un risque contentieux en cas de dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité en effet comme vous le savez, le Conseil d'État avait dans son avis, estimait que la protection absolue dont il était prévu de faire bénéficier les termes olympique Olympia olympienne étaient excessives, ce qui a modifié la rédaction de nos collègues de l'Assemblée, le texte adopté en commission de la culture prend cet élément en compte, par contre, en cas de dépôt d'une QPC le juge constitutionnel pourrait trouver pertinent l'avis du Conseil d'État, et donc en censurant cette disposition privé ces termes de toute protection pour toutes ces raisons, mon cher collègue, avec la certitude que je peux vous donner que le degré de protection très élevé dont bénéficient les termes olympique ne sera en rien impacté je vous serais recrues reconnaissant de bien vouloir retirer votre amendement. Merci madame la ministre, qui élève du gouvernement. Monsieur, ça va Monsieur le Sénateur, votre amendement vise à rendre inconditionnel la protection du terme olympique votre amendement, le comité national olympique et sportif français consultés sur la rédaction de l'article 2, telle qu'elle a été votée, tant par la commission des affaires culturelles que la commission des lois, si, si, il a dit lui-même favo favorable, le président du CNR SF estime tout comme moi, que cette rédaction présente un bon équilibre entre une protection suffisamment large de la propriété intellectuelle des termes olympique et l'exigence de la sécurité juridique la rédaction actuelle permet à la fois de protéger les droits des futurs partenaires des Jeux, donc de sécuriser leur modèle économique, tout en permettant l'utilisation du terme olympique dans le cadre du langage courant si cet usage ne présente pas de risques de parasitage de parasitisme pour sa raison, je vous demande le retrait de cet amendement, merci.

des propos du rapporteur, j'espère sincèrement que que les garanties qui seront apportées vous parler de garanties très élevé, il faut qu'il soit le plus élevé possible parce que on parle quand même d'engagement important, terme de partenariat et surtout de partenariat financier et ces garanties seront suffisantes pour protéger correctement les partenaires qui je le rappelle encore vont financer à hauteur de 97 pourcent le coût de de l'organisation de ces Jeux olympiques, j'espère aussi qu'ils répondent qu'ils vont qui est de des charges du contrat de de la ville haute, parce que là aussi il y a des engagements qui ont été pris au moment de l'obtention des Jeux avec la ville haute, qui doit respecter ses engagements, donc j'espère que tout sera sera suivie de près donc bien sûr que, avec les arguments qui sont apportées, notamment avec la position du comité olympique et sportif français, qui vient de l'entendre et et favorable à cette écriture par notre rapporteur, je retirerai mon amendement en espérant bien sûr que ce retrait puisse faire aboutir la commission mixte paritaire et que les choses puissent le déroulé de la meilleure des façons possible en espérant ne pas avoir à regretter le retrait de cet amendement, merci. Donc l'amendement de rectifier, terre et retiré nous en venons à l'examen de l'amendement numéro 41 monsieur Oui Monsieur Breda la ministre, bon, il s'agit pas simplement d'un amendement de type rédactionnel, même si, effectivement, c'est la présentation qui qui en est faite, je veux dire que l'article 2 est un article très important puisqu'il s'agit, cela a été dit, de la protection de la marque olympique, c'est très important bien sûr pour des raisons financières, mais également pour des raisons d'identité des raisons d'affirmation pour l'bon sportif en général et notamment pour le CIO et pour les scènes OSM parce que ce qui est en jeu, c'est en particulier le le périmètre du du du rayonnement de ce mouvement sportif, c'est l'impact de ces initiatives de ces organisations et les jeunes, c'est vrai, sont devenus tellement populaire, en quelque sorte, qu'il génère sur le plan financier, parfois des comportements répréhensibles de la part d'un certain nombre de sociétés, je dirais d'exploitation commerciale, voire de contrefaçon qui, de la part de sociétés qui n'ont absolument rien à voir avec l'organisation de ce type de manifestation et rien à voir avec le sport en général, donc il s'agit bien à travers cet article 2 d'une part, de veiller à ce que ne soient pas

mais il s'agit également de veiller à ne pas multiplier les risques de contentieux concernant l'exploitation et notamment du terme olympique, il faut être restrictif, certes, mais il ne faut pas l'être trop, et donc il faut veiller vraiment à à trouver ce juste mais a entre ces 2 préoccupations, je sais qu'il y a eu des discussions des négociations encore ces ces derniers jours, ces dernières heures entre toutes les parties concernées, que ce soit le CIO, que ce soit les scènes au SF, que ce soit le le gouvernement et la formule la bonne formule parce que qui mieux que l'État et mouvements sportifs

à cette rédaction, là, la rédaction de la commission culture de de la semaine dernière et je pense effectivement que tout le monde serait satisfait de cette formulation légèrement modifié par l'amendement que je propose. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. l'amendement de monsieur Lozach VISA interverti avertir les mots olympiades et olympisme sans aucune conséquence, la Commission avait privilégié la semaine dernière l'ordre alphabétique, à savoir Olympiades arrivant au avant olympisme donc ce qui nous paraissait un ordre comme un autre, je ne suis pas bien certains de discerner l'objet de cet amendement, mais qui est purement Redjep rédactionnelle j'aimais donc au titre de la commission, un amendement de sagesse à titre personnel, je n'ai rien compris. Alors elle invite sa jeunesse, Madame la Ministre. Juste pour dire aussi je dirais sagesse. 2 avis de sagesse sur cette amendement qui interverti 2 termes. La demande explication de vote mais on voit l'amendement qui vote pour.

Merci qui vote contre qui s'abstient, il était adopté, à l'article 3 je suis saisi de 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune, on commence par le numéro 6 présenté par monsieur Laurent. Oui, notre amendement vise c'est donc nous sommes dans le sujet du pavoisement tout en délimitant plus précisément la période de pavoisement surtout notre amendement vise à encourager à ce que les les messages qui seront utilisés dans le pavoisement soit des porteurs d'un message universel de paix et d'amitié, de fraternité entre les peuples, c'est donc un encouragement à à la valorisation des valeurs de l'olympisme qui figuraient de cette manière explicitement dans le projet de loi. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur mais, chers collègues, cet amendement vise à faire débuter le régime dérogatoire en matière d'affichage au terme de l'édition 2020, des Jeux olympiques de Tokyo afin de limiter le régime dérogatoire à une période de 4 ans, symboliquement le régime dérogatoire commenceraient au début de de la période 4 en courant à la fin des Jeux olympiques au début des Jeux olympiques de la fin des Jeux olympiques au début des Jeux olympiques pour les riverains et pour la préservation des monuments historiques ou classé il accorderait un répit de 2 années au lieu de faire débuter cette dérogation à la date de la publication de la loi, rien ne semble un effet justifier que le régime dérogatoire s'appliquent dès 2018 et le pavoisement aux couleurs olympiques peut se faire dans le respect des règlements locaux de publicité et de protection des sites classés remarquables historique jusqu'en 2020. Merci le 27 rectifier bis même jour. Et merci Monsieur le président des amendements analogues, viennent d'être défendu, je ne bornerai donc pas répéter les arguments avancés, je note néanmoins que l'article 3 vise à lever certaines interdictions relatives à la publicité sur le site d'opérations liées à la promotion à la préparation à l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques si une telle suspension des règles applicables en matière de publicité limitée aux emblèmes z'olympique et de l'édition 2024 des je ne pose pas problème majeur le fait de faire débuter l'entrée en vigueur de cette dérogation à la promulgation de la loi, nous paraît prématuré, nous sommes en effet à plus de 6 ans et demi d'ouverture des Jeux olympiques et les événements de promotion peuvent d'ores et déjà se dérouler dans le respect de la réglementation applicable en matière de publicité, madame la ministre, vous avez indiqué à l'Assemblée que le choix d'une entrée en vigueur de l'article 3 à la date de publication de la future loi se justifier lors d'événements comme la semaine olympique et paralympique à l'école, les journées olympiques et paralympiques ou à l'occasion des grandes compétitions sportives organisées en France pourtant, je note que l'édition 2018 de la semaine olympique et paralympique à l'école vient de s'achever le 3 février en application du droit actuel et sans que cela ne pose problème, il nous paraît donc plus sage de faire débuter l'entrée en vigueur de l'article 3 à la à la fin des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020, 4 ans nous paraissent amplement suffisant pour sensibiliser les enfants et plus largement les Français aux Jeux. Merci, il semble que l'amendement 44 ne fera pas défendu Hilton, quel est l'avis de la Commission sur ces 3 amendements, discussions communes. Merci Monsieur le Président, alors ces amendements entendent reporter l'entrée en vigueur des dérogations aux règles de publicité pour le pavoisement olympique sur ce point, je souligne que l'article 3 du projet de loi encadre déjà strictement les possibilités de dérogation aux règles d'affichage ne pourra, elles ne pourront concerner que les symboles non commerciaux liés aux jeu d'autre part, elles n'interviendront que de manière ponctuelle, par exemple, à l'occasion de manifestations et seront circonscrite au site de ces manifestations différer l'entrée en vigueur des dérogations aux règles de publicité plus de 2 ans, ne fera que retarder l'organisation rendre moins visibles, les opérations de promotion des jeux susceptibles d'être organisé il serait dommage de ne pas profiter au plus tôt de la notoriété de cet événement exceptionnel pour promouvoir le sport et la culture dans notre pays, l'amendement 6 propose par ailleurs de limiter les dérogations au dispositif qui comporte également un message universel de paix et d'amitié, de fraternité entre les Peuple cette rédaction pourrait rendre impossible l'affichage de ce qui comporterait seulement le logo Paris 2024, de même que les enseignes pré-enseignes qui sera apposé sur les sites de compétition et à proximité et à proximité au moment des Jeux pour ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable à ces amendements. trois, le 6 le 21 rectifier le 27 rectifier bis, Madame la Ministre. Je pense que vous faites une conviction entre la publicité et le pavoisement le pavoisement des anneaux olympiques les symbole des anneaux olympiques dans l'espace public, il est donc important d'afficher notre fierté d'avoir les et mobiliser tous les Français, dès maintenant, comme je l'ai déjà dit effectivement nous à nous n'allons pas manquer de grands événements, dès 2018, effectivement, nous avons eu la semaine olympique, nous allons avoir les Journées olympiques et paralympiques des grandes compétitions sportives mais aussi des événements culturels et majeur, l'idée c'est de valoriser notre territoire est valorisé, je dirais cette fierté d'avoir les jeux, donc ce sera que sur les des espaces publics et je pense qu'aujourd'hui nous avons attendu son temps, nous pouvons aussi valoriser et utiliser cet espace géré en tant que pavoisement mais pas comme de la publicité.

Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur mais, chers collègues, cet amendement vise à substituer au maire de Paris, le préfet de Paris, compétent en matière de Patrimoine et d'environnement dans la police, de la publicité pour la durée des Jeux olympiques et paralympiques pendant les Jeux olympiques et paralympiques, la mairie de Paris sera fait juge et partie, parti en tant que signataire des contrats de ville hôte avec une application des stipulations du contrat dans l'intérêt du comité international olympique, juge de par sa compétence pour accomplir accorder ou non les dérogations en matière de pavoisement au bénéfice des institutions et partenaire c'est l'objet de cet amendement. la police de l'affichage maire à partir du moment où la commune s'est dotée d'un règlement local de publicité comme la maire de Paris et signataire du contrat de ville hôte avec le CNE SF et que les collectivités territoriales qui vont accueillir des sites olympiques compte également signé des lettres d'engagement, les auteurs de cet amendement évoque le risque d'un probable conflit d'intérêts qui pourrait être préjudiciable à notre Patrimoine, j'avoue que c'est un point que j'ai souhaité effectivement approfondir avec les personnes que j'ai entendu lors des autres auditions en préparant mon rapport, d'une part, il apparaît le que le fait que la maire de Paris ne soit pas partie prenante au COJO chargé des Liens avec les partenaires marketing et signataire du futur accord sur le plan marketing, mais seulement de la Solideo limite ce danger, d'autre part, il semblerait que le préfet de Paris ne dispose pas aujourd'hui des services compétents pour lui permettre d'instruire l'ensemble des demandes à la place des services de la ville, il peut se substituer à la maire de Paris, s'il est saisi pour une défaillance et donc instruire très ponctuellement dossier mais il n'a pas la capacité de traiter de l'ensemble des demandes peut-être madame la ministre pourra-t-elle, d'ailleurs nous donner davantage d'éclaircissement à ce sujet, mais pour ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable à cet amendement. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement. Effectivement, comme vous le savez, quand il existe un règlement local de publicité l'autorité compétente, le maire et non le préfet il y a aucune raison de modifier cette répartition des rôles spécifiquement pour les Jeux, les services de l'État non il expertise ni les effectifs nécessaires en matière de publicité, cela reviendrait à faire signer des autorisations aux préfets, qui serait dans les faits, instruite par les services des collectivités locales, enfin il serait illogique d'établir une règle différente pour Paris et les autres collectivités concernées par les Jeux, je propose donc un retrait de cet abonnement. Demande de retrait Madame Mellow. Je vous remercie pour tous ces éclaircissements sur le plan juridique, effectivement, bon je je me range à vos arguments, c'est une question qui mérite d'être posée, mais bon, j'accepte de de retirer mon amendement. L'amendement est donc retiré, vous pouvez poursuivre Madame nous présentons le 14 rectifier. aux supports destinés au pavoisement les plus les plus hautes exigences environnementales afin de limiter la pollution visuelle et sonore pour les riverains, il s'inscrit dans une démarche de jeux olympiques et paralympiques sobre et respectueux de l'environnement, les dispositifs de promotion de cet événement doivent respecter cet engagement à la préservation de l'environnement. Merci, monsieur le rapporteur pour la commission. Merci Monsieur le Président, effectivement, je comprends le souhait de Madame May, l'auteur de cet amendement de limiter au maximum l'impact environnemental des dérogations mises en place néanmoins les projections sur les façades me paraisse susceptible de causer moins de dommages et d'être de plus courte durée que l'installation de barrages ou de panneaux, elles sont de plus en plus fréquemment utilisée et les procédés sont susceptibles encore d'évoluer d'ici 2024, c'est pourquoi nous donnons un avis défavorable. Madame mais le le pavoisement lumineuse sera bien soumis à une déclaration préalable l'autorité compétente pourra s'y opposer, si elle juge que la dispositifs ne sont pas respectueux du cadre environnemental, en l'occurrence je doute vraiment que les maires acceptent de voir leur ville dénaturé par des projections lumineuses disgracieuse pour cette raison, je suis aussi défavorables pour cet amendement. 2 avis défavorables Madame Mellow. Je vais le retirer, il serait long et fastidieux de dresser une liste de tous les cas d'interférences politiques, religieuses ou économiques dans l'histoire des Jeux olympiques, mais alors qu'il revient à Paris et plus largement à notre pays d'organiser pour la 3ème fois les Jeux olympiques et paralympiques d'été, il nous paraît nécessaire de revenir aux sources de l'olympisme, tels que définis dans la charte olympique l'article 3 du projet de loi prévoit une série de dérogations au code de l'environnement, en matière de publicité limitée à l'affichage des symboles olympiques, parmi lesquels le drapeau, le logo de Paris 2024 la mascotte ou le slogan des Jeux, il nous paraît particulièrement opportun d'élargir cette dérogation aux grands principes qui fondent l'olympisme, nous pouvons par exemple nous retrouver autour du second principe qui a indiqué que le but de l'olympisme et de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique et soucieuse de préserver la dignité humaine, non pour tout autant rappeler à tous : l'article 50 de la charte olympique qui proclame qu'aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou 3 classement olympique je vois également dans le 4ème principe une forte revendication pour l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, il proclame en effet que la pratique du sport est un droit de l'homme et de la femme et que chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité et de fair-play, je rappelle qu'en 2011, la délégation droits des femmes du Sénat avait bien montré qu'en matière d'égalité des femmes et des hommes dans le sport, des efforts restent à accomplir, alors que nous ambitionnons de faire des jeux éthique transparent propre, nous pourrions nous enorgueillir d'encourager cette aspiration à l'égalité, je vous remercie. monsieur le président, alors si des difficile de ne pas souscrire aux principes fondamentaux de l'olympisme, définie par la charte olympique comme, je cite, une philosophie de vie exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps de la volonté et de l'esprit, fin de citation, il paraît tout aussi difficile de parvenir à condenser ces derniers sur une bannière à la fois lisible inédit et d'une dimension raisonnables, c'est pourquoi si sur le fond, je souhaite comme vous Madame Laborde, que les manifestations et événements de promotion des Jeux olympiques qui seront organisés au cours décidé prochaines années et demie soit l'occasion de promouvoir les principes fondamentaux de l'eau de l'olympisme, il me paraît toutefois plus raisonnable que les affiches et bannières qui seront alors comporte uniquement les symboles olympiques et paralympiques, donc c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Tout comme vous je partage aussi les valeurs de l'olympisme, ce n'est pas l'objet de cet article, en revanche, vous souhaitez que les dérogations ouvertes au pavoisement concerne également la promotion des principes fondamentaux et articles issus de la charte olympique, or le contenu du pavoisement telle qu'il a défini dans le projet de loi fait déjà indirectement à la promotion de ses principes et valeurs, c'est pourquoi je suis aussi défavorable à votre amendement.

Merci monsieur le président, comme j'ai expliqué à mes collègues ce matin en commission culture, éducation, communication, il me semble que, à chaque fois que j'aurai l'occasion je vous rappellerai l'article 50 de la charte olympique et comme je ne voulais pas que ce soit classée cavalier, j'avais essayé par le mode du pavoisement de pouvoir vous inciter à faire attention à cet article 50, je vous remercie. Monsieur Laurent. je voulais puisque cette l'amendement déposé rejoint une préoccupation que j'essaie d'exprimer tout à l'heure, je sais bien qu'ici tout le monde dit son consensus sur le soutien aux valeurs olympiques. Mais au moins ces 2 amants rend Mandement ont eu le mérite d'attirer l'attention sur le fait que dans la vie concrète quand même après ça ne va pas de soi, et que si nous voulons une véritable promotion de ses valeurs, il faudra l'organiser y consacrer des efforts surtout que l'envahissement publicitaire, lui, n'aura pas besoin de notre appui, il sera naturel et extrêmement présent si nous voulons que ce qui a fondé l'olympisme soient vraiment présents la tension à à à la préoccupation que nous exprimons devra quand même tous nous mobiliser.

Qui vote contre. Non, il n'est pas adopté le 23 rectifier bis madame Hénault.

dans l'esprit de l'organisation de jeux olympiques et paralympiques sobre écologiquement responsable, il convient de limiter la pollution visuelle et sonore des dispositifs peu polluants doivent être privilégiés dans la publicité sur les Jeux olympiques et paralympiques au nom du respect de l'environnement.

je rappelle d'ailleurs que le développement durable est inscrit au coeur du projet des jeux de Paris 2024 le dossier de candidature mentionne ainsi le principe de jeux propres irresponsable, malheureusement, la rédaction de cet amendement ne me paraît pas suffisamment précises pour figurer dans la loi, comment apprécier si les matériaux recyclables auront ou non été privilégiée, c'est pourquoi la Commission a donné un avis défavorable à cet amendement pour autant ce débat nous donne l'occasion de marquer publiquement notre attention à ce que les Jeux de 2024 soit sobre et écologique. Merci madame la ministre. par les annonceurs, si elle juge que les dispositifs ne sont pas respectueux du cadre environnant.

Il est défendu. Il a défendu l'avis de la commission s'il vous plaît, sur les 47 rectifier. Oui, ce n'était pas le seul signataire. Donc, il n'était pas le seul. Signataire. Moi, j'avais comme seul signataire, c'est pour ça. Merci Monsieur le Président, donc permettez-moi tout d'abord de vous indiquer que les organisateurs des Jeux, que nous avons auditionnées nous ont tous assuré que le but ce n'était évidemment pas de couvrir intégralement le périmètre dérogatoire de publicité le rayon de 500 mètres se justifie pour 2 motifs d'une part, le CIO avait demandé en 2015 dans un questionnaire adressé aux villes candidates pour l'organisation des Jeux en 2024 quelles étaient les conditions d'acquisition de tous les espaces publicitaires existants ou futurs situées dans un périmètre d'un rayon de 500 mètres autour des emplacements envisagés pour accueillir les Jeux, d'autre part, la distance de 500 mètres correspond à celle utilisée en droit français pour déterminer le périmètre automatique des abords autour des monuments historiques, comme ces dérogations ont vocation à délimiter les abords des sites olympiques, il était assez logique de conserver la même distance, il est vrai que les abords ne concerne que les immeubles situés dans le périmètre de 500 mètres et entrant dans le Champ de co-visibilité du monument historique, ce qui est plus limitée, mais la zone des abords est un périmètre protecteur, il n'y a pas lieu de mentionner le critère de la co-visibilité puisque le but de l'article 4 et de lever temporairement les règles applicables en matière de publicité pour ces raisons avis défavorable. le rapporteur l'a très bien rappelé pourquoi, en fait, nous avons choisi ce périmètre, le périmètre de ce 100 mètres celui sur lequel se sont engagés, toute la collectivité haute en transmise tant Des lettres d'engagement au CIO en face de candidature, qui est envisagée depuis le début de l'examen du texte avec le COJO et il ne semble donc pas pertinent de revenir sur ce périmètre. Madame Laborde, l'explication de vote. Oui, excusez-moi, nous nous réveillons tout à l'heure, et donc c'est vrai que par rapport quand même à ce qu'on appelle la co-visibilité, on était un peu perplexe par rapport aux 500 mètres, donc c'est vrai que vous avez donné des explications et comme l'auteur principal n'est pas là, nous allons vous plaît nous plier à vos explications.

Oui, il s'agit d'un d'un amendement qui vise à à à limiter les possibilités d'Exposition publicitaire sur les bâtiments classés historiques, les réserves et parcs naturels, je crois que le risque de vous, nous avons conscience effectivement tout sauf dans un projet de loi qui doit tenir compte des engagements qui ont été pris par la ville, mais le risque quand on lit l'ensemble du projet de sous-Exposition publicitaire n'existe pas le le risque aucune devant lequel nous pouvons-nous trouver est plutôt celui de la surexposition publicitaire qui correspond d'ailleurs un problème de marchandisation croissante du sport, donc nous proposons de limiter en supprimant 2 des alinéa de cet article, les possibilités d'Exposition publicitaire sur les bâtiments classés historiques. 49 rectifier identique au précédent, elle besoin. Comme il est identique, et qu'il a été fort bien défendu, nous nous contenterons de l'explication de notre collègue. Il est défendu l'avis de la Commission, monsieur rapporteur. Merci Monsieur le Président, alors pour limiter au maximum le risque des éléphants blancs, l'une des caractéristiques de la candidature de Paris pour accueillir les JO de 2024 a été de s'appuyer autant que possible sur les équipements sportifs existants mais aussi sur le Patrimoine, l'affichage de publicités commerciales sur les sites olympiques et leurs abords, fait partie des obligations qui figure dans le contrat de ville hôte et auquel la Ville de Paris et le CNE SF ont souscrit, il s'agit par ailleurs d'un élément important de l'équilibre financier des Jeux comme on l'a déjà dit et les recettes publicitaires devraient constituer près du tiers du budget du COJO, je ne peux pas nier que ces dérogations se traduiront par une pollution visuelle, mais ces atteintes au Patrimoine resteront très temporaire puisqu'elles se limiteront à une période de 3 mois autour du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques, par ailleurs, seuls les monuments This historique qui abrite des compétitions seront concernés, quoi qu'il en soit, aucune publicité ne pourra être apposée sans avoir fait l'objet d'une autorisation préalables et des critères précis, en encadrant la délivrance pour ces raisons avis défavorable. Madame le ministre, pour le gouvernement, s'il vous plaît. Alors le projet de loi encadre l'affichage dans 3 domaines dans le temps 30 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques et 15 jours après la clôture des Jeux paralympiques, dans l'espace avec un périmètre dans un périmètre de 500 mètres autour du de chaque site de compétition et, en fonction de la nature des supports et procédé publicitaires qui devront s'insérer dans le cadre de vie environnants et je voudrais juste dire à nouveau, c'est le seul événement où il n'y aura pas de publicité à l'intérieur de l'enceinte sportive, donc il n'est pas dans la volonté, ni dans l'intérêt de personne de porter atteinte ou dégradé les monuments historiques, les sites ou les monuments classés, la publicité sera dans tous les cas, subordonnée à une autorisation préalable, je le redis, qui pourrait être refusée par l'autorité compétente, j'aimais donc un avis défavorable aussi à cette proposition. 2 avis défavorables sur ces 2 amendements pas demande explication de vote, je n'en vois pas je vais les mettre aux voix qui vote pour. Ceux qui votent

les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un rendez-vous qui est majeur pour la jeunesse de notre pays, or l'article 4 concerne les dérogations aux règles de publicité qui s'appliqueront au profit des partenaires marketing olympique alors nous connaissons les 11 sponsors du CIO, nous ne connaissons pas encore les sponsors et les partenaires du COJO il y a un problème spécifique avec l'alcool, il ne faut pas que ces grandes compétitions incite à la consommation d'alcool, car de nombreuses études ont prouvé que la publicité directe ou indirecte qui est produite à ce moment-là en direction de notre jeunesse, développe un impact Direct sur la consommation d'alcool, les alcooliers plutôt une catégorie d'entre eux, principalement les brasseurs pour ne pas les nommer, ont développé des stratégies de contournement des dispositions légales en la matière et cette stratégies, elles sont massives lors du dernière Euro de football l'année il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans en France Les 8 matches qui ont été enregistrés ont généré 20 heures de diffusion et, durant cette période 849 référence référence publicitaire à l'alcool ont été comptabilisés par une étude universitaire diffusé parlant pas ça correspond à une moyenne de une référence publicitaire toutes les 87 secondes et la quasi-totalité, porte sur ce qu'on appelle les marques alibi qui reprennent les logos, les codes couleurs, l'ensemble des référentiels visuelle de l'alcool, sans évidemment citer la marque d'alcool, cet amendement vise donc à exclure du Champ des dérogations en particulier c'est marques alibi pour que cesse le contournement de notre foi en la matière et que cesse l'incitation aux jeunes à consommer de l'alcool lors des événements sportifs, je vous remercie. Merci Monsieur le Président, alors Monsieur Jomier, vous avez raison de souligner que la consommation d'alcool est un enjeu majeur de santé publique et la difficulté de votera amendement réside dans le fait que les dérogations de publicité concerne les parcs de partenaire de marketing olympique du CIO, cette organisation est libre de choisir ses partenaires avec lesquels elle souhaite contracter et il ne nous appartient pas de la limité dans ses choix lors des dernières éditions des Jeux olympiques, aucun alcooliers ne figurer parmi la liste des partenaires du CIO, ce qui devrait peut-être être de nature de nous pouvons d'ailleurs profiter de cette occasion pour adresser comme vous l'avez fait un message vous co-jobs qui devrait choisir ses partenaires dans les prochains mois afin qu'il prenne en compte parmi ses critères de choix cet enjeu majeur de santé publique, dernier élément : l'article 50 de la charte olympique interdit expressément les annonces publicitaires et les publicités au-dessus et à l'intérieur des lieux de compétition, cela signifie qu'à la différence des championnats de football par exemple aucune publicité ne sera visible lors des retransmissions télévisées des épreuves au bénéfice de ses observations, je vous demanderai soit de retirer votre amendement, faute de quoi l'avis de la commission sera défavorable. Même ministre. Monsieur le sénateur Jomier, nous essayons de de déroger à minima la publicité pour les boissons alcooliques est d'ores et déjà encadré en application de la loi il n'y a pas lieu de la compléter pour ce qui concerne les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc un avis défavorable Ministre. Monsieur Jomier. Monsieur le rapporteur, j'entends bien mais l'article IV ne parle pas des partenaires marketing du CIO simplement démarqué partenaire mais. or il y a ceux du CIO je vous donne acte que nous les connaissons Léonce, il n'y a pas d'alcooliers, nous ne connaissons pas les partenaires du COJO, par ailleurs, Madame la ministre, rapporteur, cela ne résout pas la question des marques alibi, je vous ai donné des chiffres qui montrent que la loi Évin a été massivement contourner lors de l'Euro 2016 de football et que les alcooliers en particulier les bras, c'est encore une fois, ont une stratégie avec création de marque qui portent les mêmes codes couleurs qui portent les mêmes logos qui portent les mêmes références visuelles et Audio et qui vise à ce que le jeune fassent lien Direct entre la marque alibi et la marque d'alcool, donc le dispositif actuel est insuffisant, imprécis, certains savent très bien le détourner, ils le font, nous devons protéger notre jeunesse, nous devons poser que les dérogations que je ne remets pas en cause, qui sont accordées au CIO ne porte pas sur l'alcool et les marques alibi donc je maintiens l'amendement. Mon cher collègue, et je ne voudrais pas qu'on puisse croire qu'il y a ceux qui sont favorables à des restrictions aux publicités sur l'alcool et ce qui ne serait pas mais, comme l'a dit aussi bien, Madame la Ministre, que notre rapporteur de la commission d'éducation et des Affaires culturelles, la loi Évin s'applique de plein droit et si vous dites qu'elle est contournée, je ne vois pas pour quelle raison les règles que vous posez, ne serait pas elles aussi et par conséquent des problèmes d'application de la loi, ne sont pas d'une telle nature qui doivent nous conduire à la changer pour les seules publicités qui seraient déployés déployés autour des sites des Jeux olympiques, ou bien il y a un problème pour la loi Évin et nous devons le traité ou bien nous considérons que ce n'est pas le problème de la loi, mais un problème d'application de la loi et ça n'est pas votre amendement qui le résoudra je crois que il n'y a aucune extraterritorialité bien entendu pour les annonceurs qui feront de la publicité à l'occasion des Jeux olympiques, et par conséquent, nous n'avons aucune raison de rajouter des dispositions spécifiques, là où le législateur a déjà pris des dispositions générales. Pas de demandes d'explications de vote, madame de La Gontrie. Oui, Monsieur le Président, j'entends bien les positions des uns et des autres, mais j'entends aussi l'intervention du président de la commission des lois quitte une autorité en matière juridique, alors je lui dirais simplement que, attention, les marques alibi n'existaient pas au moment de la loi Évin, tant qu'on peut toujours considérer qu'il faudrait rectifier la loi Évin, sauf que nous devons aussi être précurseur dans notre mode de protection de ceux qui peuvent être les cibles de cette publicité, donc encore une fois, les marques alibi, c'est un concept qui est assez, comment dire, peu connu de certains, mais auquel nous devons être très attentif et là encore, donnant un signe et montrons notre préoccupation et le fait que nous ne sommes pas dupes des démarches de certains. Plus de demandes, je vais mettre aux voix c'est amendement numéro 39 avec 2 avis défavorables commission gouvernement qui vote pour.

marques. Je président Madame madame la ministre, messieurs les rapporteurs cet amendement une pute aux annonceurs tout dommage causé sur des monuments historiques classés dans le cadre des dérogations prévues à l'article IV du présent projet de loi, il s'agit d'une mesure de Bruxelles, estimant que le contribuable ne doit pas supporter des dégâts causés par des annonceurs. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Merci monsieur le président, Monsieur Marc, votre souhait de garantir que le contribuable contribuables français ne se verra pas imputer les frais de réparation dans le cas où un dommage aurait été causé par un dispositif publicitaire dérogatoire est parfaitement compréhensible, le souci de ne pas trop solliciter financièrement les Français dans l'organisation de ces Jeux, justifie la mise en place de ces dérogations aux règles d'affichage pour engranger justement des recettes publicitaires votre amendement ne paraît par contre déjà être satisfait par les règles générales en matière de responsabilité les l'article 1242 du Code civil prévoit clairement qu'une personne est responsable du dommage causé par son propre fait, ou par des choses qu'elle a sous sa garde, peut-être pourrions-nous cependant demandé à la ministre de nous confirmer que les autorisations de publicité qui seront délivrées par l'autorité chargée de la police de l'affichage comporteront bien une clause précisant que le père missionnaire responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter de son dispositif publicitaire et qu'il est tenu de le maintenir en permanence en bon état et assez frais exclusifs dans ces conditions, je vous propose de retirer votre amendement sinon la Commission a donné un avis défavorable. Monsieur le sénateur tout dommage causé à une propriété doit être réparé par la personne qui la dégradent ceci est déjà prévu par la loi et donc cette loi s'appliquera aussi aux Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Donc, l'avis est défavorable effectivement. L'avis est défavorable également monsieur main. Oui, compte tenu de ces éléments et de la réponse, je m'excuse de la ministre, mais beaucoup plus complète de la part de monsieur le rapporteur, je retire cette amendement.

Même vote même vote le 5 bis même vote il est adopté et à l'article 5 terre j'ai une demande de parole de monsieur Merci Monsieur le Président, donc, cet article a été introduit par les députés et prévoit donc la publication par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'une charte de volontariat olympique et paralympique appliquée aux bénévoles qui participeront donc à la préparation au déroulement des Jeux. Cette charte est une bonne initiative, mais cette charte ne doit pas non plus à nous interdire d'avoir un un réel débat sur le bénévolat 70000 bénévoles seront nécessaires pour assurer le succès le bon déroulement des Jeux aussi il est important de prémunir les bénévoles Les bénévoles contre de possibles abus et de formuler formaliser leurs droits, leurs devoirs et les garanties qui leur sont apportées lors de l'Euro 2016, des contrôles avaient conduit à la requalification en contrat de travail, des contrats, des bénévoles, ce qui avait alors induit des surcoûts financiers financiers non négligeables et une insécurité pour ces derniers, il est important de s'en prémunir à l'avenir, tant pour les bénévoles, des jeunes que pour l'ensemble des grands événements, je sais que des réflexions sont en cours, tantôt gouvernement qu'au sein du Parlement pour réformer le statut du bénévole, mais d'aller trop rapide de l'examen de ce texte n'ont pas permis d'introduire des mesures précises, mais nous restons attentifs sur ce point l'avenir tant pour reconnaître les bénévoles dans le cadre de grands événements sportifs que ce investis quotidiennement dans leurs clubs et associations, il s'agit là donc d'une première étape, je suis certain que la réflexion engagée permettre un traitement plus complet de cette question dans les prochains mois de contentieux, vous Madame la Ministre, pour pouvoir mettre au Parlement, ce débat sur le statut, le rôle et le contrôle des bénévoles merci.

il s'agit d'un amendement qui vise à introduire dans le projet de loi, une référence à la charte sociale, Paris 2024, nous pensons que c'est important, parce que la charte sociale, Paris 2024 unique innovation de la candidature de Paris au même titre que d'autres innovations en matière éthique et environnemental, elle est aujourd'hui, elle fait consensus puisqu'elle a donc cette charte été validé par le COJO, soutenu par l'ensemble des organisations syndicales et par les organisations d'employeurs, évidemment, elle n'a de valeur que si les si elle est respectée, donc, cet amendement vise à mentionner explicitement cette innovation de la charte sociale et a appelé ce qui va de soi, à son respect par l'ensemble des entreprises et partenaires sélectionnés dans le cadre des Jeux olympiques.

à tous les partenaires des Jeux olympiques et la charte d'insertion sociale qui a été, je rappelle ajouter dans le texte par l'Assemblée nationale et étendue par la commission des lois, il apparaît en réalité qu'à la lecture de cette charte, elle n'est pas destiné à s'appliquer aux entreprises car un très grand nombre de ces clauses ne concernent pas les entreprises, vous y verrez notamment, mais des clauses portant sur l'égal accès à la commande publique ou sur la présence des syndicats au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques je crois qu'il faut s'en tenir à notre droit du travail, notre droit commun pour garantir les objectifs qui sont visées par la Charte s'agissant de ces entreprises, c'est pourquoi il s'agit d'une demande de retrait ou d'un avis défavorable à défaut. Madame la Ministre. La charte sociale signée effectivement par les 5 principales organisations syndicales, a pour objet de placer l'emploi de qualité et les conditions de travail des salariés au coeur des je vous proposez de prévoir dans la loi une disposition visant à rendre obligatoire le respect de cette charte à l'ensemble des entreprises et partenaires sélectionnés dans le cadre des Jeux je suis défavorable, je vous dirai pourquoi, en effet, cette proposition n'est pas conforme à la démarche engagée à travers cette charte, il ne s'agissait pas de prendre des dispositions normatives les engagements contenus dans cette charte correspondent à des dispositions de code du travail de fait les partenaires des Jeux olympiques sont d'ores et déjà tenu de s'y conformer au regard des normes en vigueur et du droit du travail français, qui sera mis en oeuvre et respectée durant la préparation et l'organisation des Jeux, l'ambition de la charte est autre : il s'agit de mettre en avant les règles sociales les plus essentielles et fédérer et de fédérer les acteurs autour de leur mise en oeuvre, c'est ce que nous nous engageons à faire, mais ce ne cela ne relève pas de la loi, mais nous nous y impliquer. nous allons maintenir l'amendement et je je suis un peu étonné des des réponses qui nous serons faites parce que on on semble en retrait sur un engagement nouveau qui est pris par la candidature par le coup jour lui-même je, je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure Bernard Thibault qui a été chargé de ce travail, qui siège pour les organisations syndicales au sein de l'OIT, va siéger et dans le COJO et dans la Solideo, il y a donc un engagement fort des organismes qui sont chargés de de garantir la réussite des Jeux, donc on peut éventuellement arguer de telle ou telle maladresse dans la rédaction de l'amendement, mais je pense que ce serait extrêmement utile que la loi encourage au respect parce que on ne peut pas nous répondent que c'est très bien que la charte existe, mais surtout elle est pas obligatoire et donc elle est par définition essentiellement facultatives non 6, si nous prenons la peine et si les organismes qui organise les Jeux ont décidé d'aller dans ce sens, c'est parce que ils attendent effectivement que la charte soit respectée, donc je trouve que ce serait dommage de ne pas mentionner explicitement cette innovation dans la loi. Donc, l'amendement est maintenu de demandes d'explications de vote, je n'en vois pas je vais le mettre aux voix, 2 avis défavorables, je vous le rappelle, qui vote pour. Qui vote contre. Il n'est pas adoptée à l'article 6 je suis saisi l'amendement numéro 38 qui est présenté par Monsieur Théophile. Oui, telle qu'il a été rédigé la la la, alinéa 1 de l'article 6 prévoit que la liste des projets plans et programmes qui sont nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et qui peuvent potentiellement bénéficier des dispositions du présent article doit être fixé fixé par arrêté ministériel, ce dispositif n'est pas satisfaisant quand elle le voit être actualisé à intervalles réguliers en 2 et présente un risque de contentieux non négligeable, qui est de nature à retarder la mise en application du dispositif institué par l'article 6, cet amendement propose donc de supprimer cette liste dans le but d'introduire un peu plus de souplesse. Merci l'avis de la commission Mallet rapporte. Le projet de loi qui avait été transmis au Sénat, utiliser des termes différents pour définir le périmètre des des dispositions du projet de loi et la commission des lois, s'est attaché à harmoniser le terme utilisé pour sécuriser en été, les aménageurs et puis et réduire les risques de contentieux, alors ça s'est traduit de manière premièrement par une harmonisation gérer dans le gérer dans le temps où les termes préparation organisation déroulement des Jeux olympiques et paralympiques ont systématiquement été repris pour exposer quelles étaient-elles les projets et puis aussi par le renvoi, un arrêté ministériel, celui-là même qui est contesté dans l'amendement pour lister les projets, les plans ou les programmes qui devait faire l'objet de ces procédures dérogatoires, c'était une partie de l'article qui visait notamment à régler une difficulté, en réalité, s'agissant de la zone d'aménagement concerté qui doit accueillir un des équipements qui est la reine à 2. Un article qui s'est article 8 qui sera prochainement, si vous en êtes d'accord modifié par l'amendement 54 qui va être présenté tout à l'heure, dans ces conditions, je suis favorable à l'amendement de compromis qui vient d'être présenté et qui supprime le renvoie l'arrêté ministériel, une somme que la rédaction des articles 6 et 8 est suffisamment clair désormais pour se passer de se rend. Madame la ministre, elle avait du gouvernement unissent pardon. Président, mesdames et messieurs les rapporteurs pour exactement les mêmes raisons, qui vient d'être évoqué, j'ai un avis également favorable à cet amendement. Eh bien, 2 avis favorables, je vais mettre aux voix l'amendement qui vote pour. Merci qui vote contre qui s'abstient, il est adopté, l'amendement numéro 9, monsieur Laurent. Ici, nous comprenons parfaitement le besoin de rapidité dans l'élaboration de l'édit de l'exécution des différents de l'infrastructure, nous estimons maladroit de substituer aux procédures de actuel de consultation du public des consultations par voie électronique, parce que c'est à ça on fait que revient la solitude, la simplification qui est proposé et donc nous proposons la modification qui qui est dans cet amendement en ce sens. Merci l'avis de la commission, le rapporteur. La substitution de de la consultation par voie électronique, la participation du public par voie électronique à la procédure de droit commun à tout de même l'Avantage de permet de faire gagner plusieurs mois par rapport à cette première procédure elle ne manque pas de garantie, il y a des garant qui est désigné et la commission des lois, de surcroît, ajouté aux garanties qui étaient déjà prêts prévu pardon dans le texte, de sorte que je suis défavorable à cet amendement qui, présentée par notre collègue Monsieur Pierre. Je serais également défavorable, monsieur le sénateur à cet amendement, l'objectif de cet article VI et d'accélérer tout en maintenant un maximum de droit, ces droits sont maintenus parce qu'effectivement, il y aura, au-delà des mesures classiques de consultations par voie électronique, la nomination d'un certain nombre de par notamment la Commission nationale du débat public, donc je mettrais un avis défavorable à votre amendement. Monsieur Laurent. L'amendement est retiré, nous examinons 34 rectifier bis Madame jours, vous avez la parole. Monsieur le président, nous entendons nous entamons la l'examen du titre 2 qui prévoit plusieurs dispositifs dérogatoires afin d'accélérer la réalisation d'équipements et d'infrastructures qui concourent à la préparation, l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques l'article si cela a été dit, vise à substituer à la procédure normale de participation du public une procédure allégée habituellement applicable aux plans et aux programmes pour lesquels une enquête publique n'est pas requise l'article L 100 même 3 tiré 19 du code de l'environnement prévoit une consultation par voie électronique, d'une durée minimale de 30 jours, il précise que les observations et propositions du public déposée par voie électronique doivent parvenir à l'autorité administrative concernés en temps normal, cette procédure allégée ne concerne pas les opérations de l'ampleur de celles qui ont, pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le gouvernement a donc décidé décidé d'ajouter l'alinéa 2 qui prévoit que nous synthèse des observations et des propositions déposées par le public devra être faite et qu'elle sera confiée à un garant, nommé par la Commission nationale du débat public, l'examen de l'amendement suivant relatif à l'aide d'immunisation des garants et la question corollaire de la rame de leur indépendance, justifier le présent amendement, il vise à ce que ces Garance soit désigné parmi les commissaires enquêteurs ayant habituellement à la charge de conduire des enquêtes publiques de droit commun ces commissaires enquêteurs disposent d'une bonne connaissance de la consultation du public et bénéficient de garanties d'indépendance, Anne, outre le recours à des commissaires enquêteurs permettrait de ne pas allonger la procédure prévue à l'article 6 et améliorer sensiblement la qualité des synthèses des observations et propositions du public. Oui je je suis opposé à cet amendement pour plusieurs raisons : d'abord la désignation du garant permet d'assurer une certaine cohérence entre la phase amont participation du public et la phase aval puisque c'est un garant et qui interviendra dans dans la phase amour ensuite le garant est indépendant, il travaille sous l'égide d'une autorité indépendante qui est le la Commission nationale du débat public, comme vous l'avez rappelé et de surcroît cela brouillerait considérablement le le rôle du commissaire enquêteur, le commissaire enquêteur se prononce sur le fond du dossier l'objet du travail garant qui va recueillir les réponses du maître d'ouvrage, suite à la participation de public, mais qui est également va indiquer quelles sont les évolutions prévues par le maître d'ouvrage, il n'a pas de position à prendre à son rôle est donc très différent de celui du commissaire enquêteur, je serais donc défavorable à cet amendement, rappelons d'ailleurs que le gouvernement réfléchit à la solution et il avait été également écarté, je crois qu'il faut expérimenter cette nouvelle procédure et ne pas l'écarter avant de l'avoir mis en oeuvre. Oui Monsieur Président même Madame la sénatrice, je serai également défavorable aujourd'hui dans le droit commun, vous avez la possibilité de faire une enquête publique par voie dématérialisée ou la possibilité de faire l'enquête publique avec les commissaires enquêteurs, il est vrai que dans le cas présent pour assurer un maximum de droit, on fait une nouvelle disposition qui est l'expérimentation d'une consultation par voie électronique tout en nommant un garant, mais pour que la clarté du dispositif soit totale, il y a un impératif que ce garant ne soient pas forcément ça veut pas dire qu'il ne peut pas l'être, mais ne soit pas forcément un commissaire enquêteur qui, lui, nommé dans le cadre de l'autre procédure classique donc pour ces raisons, je serai également défavorable à cet amendement. 2 avis défavorables Monsieur bonne carrière souhaité la parole. Merci, merci, merci Monsieur le Président, je voudrais soutenir la vie les avis qui viennent d'être présentés sous hommes indifférent, ce qui vient de vous être indiqué c'est les raisons pour lesquelles une procédure spécifique étaient mises à l'occasion de l'événement exceptionnel que ce que seront les Jeux olympiques, je voudrais donner un élément supplémentaire au rejet de l'amendement, présenté il y a une position plus globale de notre assemblée, nous avons en effet travailler dans le cas d'une mission d'information qui était sur le thématique de la démocratie participative, qui était, bien sûr, comme de coutume dans notre assemblée, une mission d'un coffre de d'information de France et une des propositions que le Sénat avait formulées dans ce rapport, sur une démocratie coopératif porté justement sur le fait d'expérimenter les procédures avec garant alors il y a pas de débat entre les garants et les commissaires en enquêteur tout simplement parce que rien n'interdit à des communistes, des gens dont l'activité traditionnelle être commissaire enquêteur d'être désigné comme garant par la CNDP, il n'y a pas de difficulté non plus sur les questions d'indépendance qui est le propre des désignations qui est effectué par la CNDP qui elle-même est une pourquoi nous étions intéressés par l'approche du grand cette en cette matière, c'était d'une part, parce que plus les choses sont faites un non plus, on peut expliquer, on peut espérer qu'elle se passe bien, deuxièmement, que le garant garantit le bon déroulement des consultations mais il te porte pas d'appréciation sur le fond, ce qui, quelque part, permet au maître d'ouvrage, d'avoir plus de liberté et puis surtout, il y a un élément essentiel qui est la compte le ce que j'appellerais le continuum, c'est-à-dire le fait qu'il y avait un hangar en a notamment et qu'ensuite celui-ci puisse, permettent de faire la synthèse et vite, c'est sûr que nous connaissons entre l'amont et l'aval ou plusieurs mois, voire en mai après les procédures d'un moment on se repose la question de savoir quel est l'état du dossier donc sur le fond, au-delà de l'approche spécifique bonjour un pic il y a un vrai intérêt dans notre pays à tenter cette expérimentation à partir du garant et des arts justement de ce rôle sans aucune contradiction avec la fonction traditionnelle des commissaires enquêteurs. Merci, pas d'autres demandes d'explications de vote je n'vois pas donc je mais on voit l'amendement 34 rectifier bis avec 2 avis défavorables commission gouvernement qui vote pour. Qui vote contre. Il n'est pas adoptée, Madame la Ministre, Monsieur le ministre, chers collègues, il nous reste 18 amendements à examiner si vous en êtes tous d'accord : nous pourrions prolonger notre séance pour achever l'examen de ce texte peut-être aux alentours de 20 il en est ainsi décidé, nous en venons maintenant à l'examen de l'amendement 53 rectifier Monsieur Théophile. Oui, cet amendement a pour objet d'accroître les garanties d'indépendance et de transparence de la part de la participation du public, il projette d'éviter le lien de subordination du tiers garant liée à sa rémunération directe par le porteur d'un projet pour ce faire, cet amendement propose que la commission nationale du débat public fixe et finance les indemnités des garants et que le maître d'ouvrage du projet, le porteur du plomb ou du programme, on assure le coup en versant les sommes correspondantes à la Commission nationale. l'avis de la commission Madame la rapporteur avis favorable, favorable, monsieur Ministre même avis. Favorable également des demandes d'explications de vote, je n'en vois pas qui votent pour cet amendement.

Merci monsieur le président, c'est un non concernant des dossiers qui figurent parmi les grands absents de ce texte, l'accessibilité des sites aux personnes à mobilité réduite si les infrastructures et les bâtiments qui seront construits à l'occasion des Jeux de 2024 répondre aux critères d'accessibilité universelle, il n'en va pas de même des infrastructures existantes, loin de là, madame, rapporteur de la commission des lois, intégré en commission un amendement qui vise à faciliter les travaux de mise un accessibilité du réseau de transport en commun ferroviaire francilien, en les soumettant à la procédure de consultation du public prévue à l'article L 123 tiré 19 du code de l'environnement, nous avons bien conscience qu'une telle modification ne suffira pas à elles seules à améliorer l'accessibilité du fait de contraintes techniques forte et aussi d'un manque de financement, elle pourra néanmoins débloqués et accélérer certaines opérations je regrette cependant quant à l'assouplissement ne concerne que l'agglomération parisienne et omettent l'autre ville olympique Marseille en tant que ville hôte des épreuves de voile et de certains matches de football Marseille s'enorgueillit d'accueillir les Jeux et d'abriter, outre les lieux de compétition un village olympique et une fan zone le présent amendement visent donc à étendre au réseau de transports en commun de l'agglomération d'Aix-Marseille Provence la possibilité offerte au métro parisien est inscrite à l'à 6. L'avis de la commission même l'emporte. Je remercie notre collègue, Madame Mireille Jouve de réparer cet oubli avis favorable. Avis favorable au gouvernement, Monsieur le Ministre. Je suis également favorable à cet amendement. Or, avait également 2 avis favorables. La demande explication de vote, je n'en vois pas je mais on voit l'amendement 32 rectifier bis qui vote pour. Merci qui s'abstient qui vote contre, il est adopté, je vais pouvoir mettre au voilà retraite le 6 Pack demande explication de vote qui vote pour. Merci qui vote contre qui s'abstient, il était adopté. à l'article 7 l'amendement 31 rectifier Madame mélo. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher collègue, cet article prévoit, dans un souci de simplification des procédures de dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et les constructions installation et aménagements temporaire dès lors qu'ils sont directement liés à la préparation à l'organisation et où, et au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques 2024 un décret en Conseil d'État définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction d'installation ou d'aménagement dans la limite de 18 mois cet amendement a notamment pour objet de fiabiliser le calendrier d'installation de la structure temporaire sur le Champ de Mars, destiné à accueillir, d'une part les activités du Grand Palais pendant la réalisation des travaux d'aménagement qui sont prévus pour l'accueil des épreuves olympiques et d'autre part, certaines épreuves olympiques et paralympiques à ce double titre, la structure est directement liée à la préparation et à l'organisation, ainsi qu'au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 elle est ainsi au nombres des constructions devant bénéficier des dispositions du titre 2 du projet de loi, le double usage de la structure rend le calendrier de son installation particulièrement tendu et sensible du fait que tout retard peut avoir des répercussions sur les calendriers des travaux d'aménagement du Grand Palais la dispense de permis pour constructions temporaires et donc particulièrement utile l'amendement permet de surmonter une difficulté liée à la rédaction de l'article 7 qui lie le bénéfice de la dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à une durée d'implantation conçu pour les installations utilisées pour les Jeux, il le complète par un cas de dispenses appuyant cette fois, comme le prévoit déjà l'article R 421 tiré 5 de ce code sur la notion de durée 2 chantiers, étant donné qu'il s'agit d'une mutualisation d'une structure temporaire, il serait important de pouvoir lui accorder une dérogation merci. Merci, cher collègue Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission s'il vous plaît. Voilà un sujet à la fois important il est délicat : la durée dispense qui nous serait demandé pour le Grand Palais provisoire du dispense de permis de construire, serait porté à d'une part, la durée du chantier de rénovation du Grand Palais, à laquelle il faudra ajouter les 18 mois qui est la nouvelle durée prévue par notre texte pour l'organisation des Jeux, de sorte que le Grand Palais provisoire pour être installé, donc sans autorisation particulière, permis de construire pendant plus de 3 ans et demi sur le Champ de Mars pour une superficie d'environ 10000 m2. Superficie qui pourrait être augmenté lors des des grands événements, alors on voit bien quel est l'Avantage effectivement de cet amendement, qui dispense le maître d'ouvrage d'un permis de construire, ce qui représente évidemment un gain de temps substantiel, même s'il reste d'autres autorisations à obtenir, sur lesquels des recours serait possible et qu'une pas nuire environnementale et l'autorisation sur le domaine public, on comprend bien aussi qu'il s'agit d'injuste rather il stratégique sur le plan culturel, puisque la Biennale de Paris et la FIAC devrait sans doute s'y installer, il y a aussi des inconvénients qui était véritablement cet amendement est très dérogatoire au droit commun, je rappelle que sans autorisation la durée d'installation et de 3 mois ou 2, un an et là nous dépassons les 3 ans et demi je rappelle aussi qu'il s'agit d'un site extrêmement sensible incite à forte valeur patrimoniale, en réalité, ce type d'ouvrage, réalisé à partir d'un permis de construire précaire qui existe donc c'est donc de l'avis du gouvernement que je demande, sur ce sujet sensible. Eh bien, nous allons l'entendre si monsieur le ministre veut bien nous le donner. Effectivement madame rapporteur c'est un sujet qui n'est pas aisée, mais le gouvernement a émis un avis favorable à cet amendement pour 3 principales raisons : la première raison, c'est que le Grand Palais va écrire un certain nombre de de manifestations sportives, notamment, le cas le Talk Windows mais d'autres et que le Grand Palais ne sera disponible que si les rénovations nécessaires auront lieu et ces rénovations nécessaires ne pour un vol avoir lieu que qui site temporaire peut-être mis en place le 2ème élément la 2ème raison et vous l'avez rappelé Madame la sénatrice, et que il est vrai que le code de l'urbanisme qui stipule et introduit la possibilité d'avoir de telles dérogations le R 421 tiré 5 stipule aussi que ces dérogations peuvent être mises en place dès lors que des sites temporaires liés à l'aménagement du site principal serait nécessaire, donc à ce titre-on peut considérer que, on reste dans l'esprit du code de l'urbanisme que et de l'article R 421 tiré 5 que vous évoquiez, enfin la 3ème raison et madame la rapporteure l'a évoqué, c'est vrai que la dérogation est importante en même temps d'autres autorisations sont maintenus, notamment les autorisations au titre de l'environnement donc pour ces 3 principales raisons à la fois de fond également de nécessité d'avoir le Grand Palais disponible, le gouvernement a émis un avis favorable à votre amendement. Alors l'avis favorable du gouvernement, la commission s'en était remis à l'avis du gouvernement, ce cap, elle ne souhaite s'exprimer avant le vote.

viser spécifiquement un équipement, un lieu pour y appliquer une procédure dérogatoire ça interpelle quand même. Parce que pour le reste, alors.

et puis on va expliquer aux autres collectivités aux autres sites que pour eux c'est différent. C'est de même curieux monsieur Marc.

l'eau avait levé la main. Je vous les ou soulever le fait qu'il n'y ait pas d'autres demandes similaires, c'est vraiment spécifique au Grand Palais, le Grand Palais va être utilisé pour les Jeux olympiques et dans ce cadre-là, il faut faire un certain nombre de mises aux normes d'accessibilité et autres pour pouvoir accueillir les Jeux olympiques, donc c'est : c'est bien la raison pour laquelle il le besoin se fait sentir d'un équipement temporaires, susceptibles d'accueillir les événements qui doivent avoir lieu pendant le temps du chantier au Grand Palais et et donc ce cette structure temporaire sera mutualisé et à la fois par par le Grand Palais et pour les Élysée c'est tellement culturel et par les Jeux olympiques, puisqu'elle sera aussi utilisée ensuite pour les Jeux. Merci Monsieur le Président, président, je voulais juste revenir sur l'interrogation justifiée du sénateur aucun hélas ce contrôle de madame la sénatrice l'amendement que vous proposez ne vise pas l'amendement que vous proposez, mentionne notamment le Grand Palais dans l'exposé des motifs, mais concerne toutes les installations temporaires nécessaires pour la mise à disposition du bâtiment principal, donc je crois ce type que cela lève le l'une des interrogations justifiées du sénateur. Pas d'autres demandes d'explications de vote, donc sur le 31 rectifier un avis favorable du gouvernement, la Commission, semble-t-il, remis à l'avis du gouvernement, mais au voit qui vote pour.

comme vous le savez, un certain nombre d'épreuves des Jeux olympiques par un pic vont avoir lieu dans la Seine et donc un plan baignade a été mis au point pour rendre la Seine baignade l'à l'horizon 2024, nous connaissons tous ceux la complexité de cet objectif qui est poursuivi depuis l'antépénultième, maire de Paris, si ma mémoire est bonne, et donc qu'on peut l'excité qui est due à la multiplication des acteurs concernés, le plan qui a été établi et nécessite un strict respect des délais et du plan d'action de chacun de ces acteurs les dispositions actuelles en vigueur du CG, c'était en cas de défaillance d'un acteur ont montré une difficulté justement a constaté cette défaillance et donc cet amendement vise simplement à confier au préfet d'Île-de-France, la capacité de constater rapidement la défaillance pour pouvoir y porter remède et ne pas prendre de retard dans l'application de ce plan qui, encore une fois, ne pourrait pas souffrir évidemment de dépasser les délais qui sont, je vous remercie. L'avis de la commission Madame le rapporteur. le CIAT résoudra ses problèmes de façon interne et de manière plus générale, je crois que dans le cas de l'organisation des Jeux olympiques, il n'y a qu'une collaboration entre les différents acteurs, y compris les collectivités territoriales qui peut permettre de mettre en date d'une façon assez assez saine, je ne crois pas aux amendements sanction, c'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, le gouvernement émettre un avis défavorable pour 2 raisons : une première qui quelque Lartigue et rédigé, vous mentionnez uniquement la possibilité d'avoir une défaillance, or il s'avère que l'Artic renfort renvoie au elle 34 51 tirer un qui ne parle pas de défaillance à proprement parler qui peut également conduire les fameuses qui aujourd'hui exercent cette prérogative à ne pas vouloir le faire et le transférer aux communes ou aussi en l'occurrence et le 2ème élément, je pense qu'en fait l'article est satisfait en ce sens où le code de l'environnement et notamment le L 171 qui réussissent permettent déjà aux autorités administratives d'aller constater un manquement de l'autorité donc l'autorité administrative a déjà la capacité d'aller constater le manquement de l'autorité compétente donc pour ces 2 raisons Monsieur le sénateur j'émettre un avis défavorable sur la question. Alors 2 avis défavorables Monsieur Jomier, que faites-vous. J'entends les arguments de Monsieur Normandie, donc je vais retirer l'amendement. Moment et retiré, je vais mettre au voilà retient que le 7 bis et demandes d'explications de vote.

c'est pire, parce que en fait la réponse que vous avez donné en me disant ça ne concernera pas que le Grand Palais, effectivement quand je relis c'est bien le cas, mais du coup sur tous les sites, nous allons utiliser ces dispositions voilà je faisait ce qu'on s'interroge, au cours de la navette ou en tout cas en CMP en disant que cette disposition-là que nous venons d'adopter dans l'idée de résoudre un problème ponctuel, ça a été dit par le rapporteur par vous et par l'auteur de l'amendement va s'appliquer à tous les sites parce que c'est une position générale donc, on va tous s'affranchir du permis de construire classique, voilà pour l'avoir à l'esprit. j'en reviens à l'article 7 bis que j'ai mis aux voix maintenant qui vote pour. Qui vote contre qui s'abstient il adopté à l'article 8 l'amendement numéro 54 monsieur Bargeton le présente. Merci monsieur le président, 3 objectifs préside à cet amendement il vise à ceux d'abord, il vise à supprimer la liste des projets fixé par arrêté ministériel, sur la base des mêmes arguments que nous avons entendu dans cette discussion au moment de l'article 6, deuxièmement une précision juridique est apportée afin de couvrir au moins 2 opérations d'aménagement déjà identifié la ZAC de la gare des mines à Paris dans laquelle s'inscrit le projet d'Darren à 2 et celle de la plaine Saulnier à Saint-Denis, qui doit accueillir la piscine olympique, enfin les dispositions relatives à la participation du public ont fait l'objet d'une clarification rédactionnel, je vous remercie. Cela renvoie la discussion que nous avons eues sur l'article 6, la commission des lois, je rappelle, avait cherché à préciser dans un souci de sécurité juridique le périmètre des dispositions dérogatoires du projet de loi nous devions également nous assurer qu'effectivement que l'article 8 s'appliquer bien notamment à la à la accueillant le la reine 2 cet amendement constitue un bon compromis, je l'ai indiqué tout-à-l'heure il les efforts d'harmonisation de la commission et englobe la ZAC précités, je suis donc favorable sur cet amendement.

Qui s'abstient, il est adopté alors. L'amendement numéro 10, monsieur Laurent. Mais c'est le c'est le même amendement que celui que nous avons défendu à l'article 6 donc il est défendu et en même temps je retire parce que de toute façon va avoir le même débat le même vote. Merci donc il est retiré, donc, mais on voit l'article 8, pas d'explication de vote qui est pour l'article 8. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, je mais au bout, l'article 9. Même vote,

Merci monsieur le président, qui promeut notamment le recrutement de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'accès des PME et des TPE à la commande publique, cette charte, qui n'a pas de valeur contraignante, conformément à la réglementation européenne doit pourtant favoriser l'activité économique de ce territoire et faire profiter ses habitants des retombées en termes donc à ce titre, et plus globalement les Jeux de 2024 doivent avoir un le n'effet de levier puissant pour le développement de cette partie de la Seine-Saint-Denis, un effet les estimations prévoient que les JO pourraient générer entre 120000 et 250000 emplois pérennes notre amendement ne revient pas sur l'objectif de favoriser une démarche de responsabilité sociale de la Solideo et à travers elle de tous les maîtres d'ouvrage, il vise à associer à son élaboration, les collectivités locales et, plus largement, les acteurs de l'insertion, je pense par exemple aux maisons de l'emploi, cher à notre collègue Nathalie Delattre, qui dispose d'une connaissance aiguë des besoins et des ressources au plus près des territoires. Merci Madame le rapporteur. Ce que dit notre collègue ma paraît tellement de bon sens que je me demande jusqu'à quel point il nécessaire de l'inscrire dans la loi, ce sera donc à David sagesse. Monsieur le Ministre. J'ai, j'aurais également avis de sagesse. Alors 2 avis de sagesse commission et gouvernement. Qui est pour. Tout le monde et pour la sagesse. Ces contrats. Qui s'abstient, donc il est adopté, donc je vais mettre aux voix l'article 10. Qui est pour

Madame le Ministre, Monsieur le ministre, mais madame et monsieur le rapporteur. Chers collègues, cet amendement vise à créer un régime de recours unique pour l'ensemble des constructions et aménagements pérennes réalisé en vue de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, la durée moyenne d'un recours administratif et de 2 ans, sans compter les éventuels appels et pouvoir en cassation afin d'éviter que les projets de construction en vue ne se heurtent à l'inertie naturelle du temps judiciaire, la création d'un régime de recours unique le semble opportune en conséquence la cour administrative d'appel de Paris aura compétence pour statuer en 1er et dernier ressort sur les litiges portant sur l'ensemble des constructions des aménagements directement liés au jeu. Oui, c'est une solution intéressante, mais il s'avère qu'aucune des personnes entendues au cours de des près de 90 auditions nous avons mené une n'a déclaré avoir besoin de de cette disposition pour tenir les délais de construction, en outre, il n'y a pas d'évaluation de l'impact sur la cour administrative d'appel de Paris et finalement je rajouterai que l'article L 211 tirs, 2 du code de justice administrative permettent déjà de confier directement, par décret en Conseil d'État des affaires au cours administratives d'appel à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration en d'autres thèmes, si le gouvernement s'aperçoit d'ici 2024 d'avoir besoin de cette disposition, il y aura recours, de sorte que c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Ce sera également une demande de repousser ou un avis défavorable et je rajouterai un dernier point ce que Madame la rapporteur vient d'indiquer, c'est qu'au final, le sens de ce titre 2 a été de simplifier les procédures, mais une fois qu'on qu'on dit qu'on a simplifié les profs, les procédures se poser la question de savoir est-ce qu'on aussi en plus les recours, la décision que nous avons pris était de simplifier les procédures, mais pas forcément les recours aujourd'hui possible existant, donc tous les droits au recours sont les mêmes sont maintenus, ce sont des procédures initial que nous simplifions par ce titre de. Madame il y a de demandes de retrait. Je vais le retirer, merci pour ces précisions. D'accord, donc il est retiré, nous passons au vote de l'article 11 heures. Qui est pour. Qui et contre qui s'abstient est adopté même vote pour l'article 12. à l'article 13, une demande de parole de monsieur ça va. Merci sous présidence va être rapide : cet article prévoit que des logements destinés à des étudiants pourront être loués, du 1er juillet au 1er octobre 2000 au comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques pour accueillir les personnes accréditées, cependant nous devons porter une attention particulière au fait que ces logements doivent aussi pouvoir accueillir les étudiants dès la rentrée universitaire qui se fera très certainement avant le premier octobre 2024 et d'important de ne pas impacter négativement le quotidien des étudiants alors que nombre de peintres n'auront pas les moyens de se loger dans le parc privé, dans l'attente de la fin de l'occupation de leur logement pour les officiels par les le comité d'organisation et le si haut pour essayer de décaler les dates de fin de jeu de olympique, il faut peut-être aussi et travailler, que le gouvernement puisse appuyer cette demande pour permettre et d'éviter ces contretemps pour certains étudiants.

Merci monsieur le président, je prendrai la parole sur les articles 13 bis à 13 billets D ans une fois les articles 13 bisser 13 n'appelant pas de commentaire particulier ces 2 articles vise à sécuriser le déploiement de la ligne ferroviaire entre le centre de Paris, entre Charles-de-Gaulle et à clarifier le cadre juridique applicable à cette liaison Charles-de-Gaulle Express ils instaurent un régime dérogatoire à la concession de travaux publics qui sera mis en place pour cette nouvelle instruction fera laquelle sera conjointement exploité par aéroports de Paris, SNCF, réseau et Caisse des dépôts ce régime dérogatoire concerne sa conception, son financement sa réalisation et son exploitation, ils permettront également de déterminer les modalités d'indemnisation en cas de modification ou d'annulation du contrat de concession et de minimiser le risque de contentieux, la création de cette ligne était un engagement pris par le comité de candidature de Paris 2024 auprès du comité international olympique lors du dépôt du dossier de candidature de Paris et qui a été matérialisées par écrit en septembre dernier lors de l'attribution des Jeux olympiques et paralympiques à notre capital, il ne s'agit pas ici de marchander la création de cette nouvelle ligne contre la rénovation de lignes existantes ou d'opposer l'accessibilité nos aéroports à la mer, leur ration des mobilités du quotidien, mais d'avoir une vision pour le développement des transports en commun en Île-de-France et surtout de respecter la parole donnée lors du dépôt de la candidature de Paris ayant dit cela, et à cet endroit, il serait intéressant que nous que nous soyons éclairer sur les intentions réelles du gouvernement en ce qui concerne la réalisation des lignes de métro 15 à 18 du réseau francilien, peut-être monsieur secret d'Data pourra-t-il nous apporter des informations, je vous remercie. Merci, cher collègue, donc l'article 13 bis je suis saisi d'un amendement 11, monsieur Laurent. Oui, je vais moi aussi, à la fois intervenir en fait une seule fois sur l'amendement 11 et l'amendement 12 ans il s'agit de la même question de la réalisation de cette ligne et nous n'avons en l'occurrence, pas le même avis que l'orateur qui vient de s'exprimer sur ce dossier parce que contrairement à ce qu'on nous dit il y a un problème de il y a un problème de priorités. Alors que nous ne sommes pas certains alors qu'il est de du Grand Paris Express soit totalement sécurisé dans son calendrier et dans ses financements, on persiste à à sécuriser à marche forcée, cette ligne les financements ont été dégagés, très rapidement, alors que je rappelle que cette ligne sera coûteuse, elle est contestée, elle ne desservira pas le territoire de la Seine-Saint-Denis, puisqu'elle le traverse sans s'arrêter, elle ne donc elle ne fera donc pas partie d'un héritage dont pourront bénéficier les transports du quotidien et toutes les études, je sais qu'on les conteste, mais de nombreuses études, donc cette ligne de surcroît sera déficitaire dans son exploitation, elle posera donc un énorme problème de financement, à terme, donc nous nous considérons que la réalisation à marche forcée de cette ligne pose un problème, et contrairement à ce que nous dit-elle entre effectivement en contradiction, pour des raisons financières parce que il faudra sécuriser les investissements du Grand Paris Express et pour d'utiliser et pour aussi des raisons d'utilisation décision elle posera des problèmes sur l'exploitation actuelle des transports du quotidien, je remarque sur ce point, c'est mon dernier argument que le gouvernement n'arrête pas de nous dire en matière de fracture infrastructures des transports qu'il faut choisir et qu'il faut privilégier les transports du quotidien contre ce que le gouvernement appelle les grandes infrastructures là l'argument semble réversible puisque on nous dit que la priorité absolue doit être la réalisation de cette ligne, donc il y a quand même un art, une argumentation à géométrie variable, donc nous nous comptons, nous que la priorité, y compris du dossier de candidature reste la réalisation du Grand Paris Express et d'ailleurs quand nous avons auditionné Tony Estanguet, interrogé sur cette question des transports, il ne s'est exprimé que sur les lignes du Grand Paris Express. Merci, cher collègue, donc c'est une présentation du du 11 et du 12 ans monsieur le rapporteur, l'avis de la commission développement durable. Mais, chers collègues, je crois que l'heure n'est plus à s'interroger sur l'opportunité de ce ce dossier mais maintenant de le sécuriser, de faire en sorte que, très vite, il puisse se réaliser et qu'ils soient livrés en 2023 puisque ce ce transport ce mode de transport est inscrit dans notre dossier de de candidature, donc je crois qu'il ne faut plus tarder, il faut maintenant passer à l'action, je crois que l'intérêt public de cette ligne maintenant clairement établi, nous sommes quand même le seul pays d'Europe et du monde à ne pas avoir de desserte dédié entre l'aéroport principal est la capitale, et puis je ne vous parle même pas de l'état de nos autoroutes A 1 et à 3 qui sont en surcharge permanente et le RER B qui, qui, lui-même, bon, il n'est pas à proprement parler parler peut pas être dédié au transport des supporters des touristes et tous ces gens qui viendront les organisateurs assister à ces Jeux olympiques, et je crois enfin que cette ligne va permettent de compléter le maillage que nous attendons tous nous régions de cette métropole cette région métropole parisienne et qu'il va venir très utilement compléter le le Grand Paris Express bien sûr que nous attendons tous évidemment également. Merci donc c'est un avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci monsieur le président, je partage les propos tenus un instant par monsieur le le rapporteur je pense qu'au final, il ne faut pas opposer 2 types de projets que sont d'un côté le le Charles-de-Gaulle Express et de l'autre côté les métro du Grand Paris Express pour plusieurs raisons : la première, c'est que les utilisations ne sont pas les mêmes et on sait bien quelles sont les utilisateurs finaux de ces 2 types de transport, le 2ème élément, c'est que les financements ne sont pas les mêmes dans le cas notamment du Charles-de-Gaulle Express comme vous le savez à partir si même mémoire est bonne, de 2024 ce sont également les voyageurs aériens qui financeront l'installation donc les financements ne sont ne sont pas les mêmes et 3ème élément, vous avez évoqué, monsieur le sénateur, le fait que nous sécurisation par ses 3 premiers articles 13 bis à 13 bis B et 13 blessés le Charles-de-Gaulle Express mais le dernier article sécurisant fait fait les projets de métro du Grand Paris Express au final par notamment les sujets de longueur de 2 trains longueur de gare, donc au final par ce texte vous sécuriser juridiquement à la fois le Charles-de-Gaulle Express mais aussi les métros du du Grand Paris Express

le commentaire de la discussion générale, effectivement, l'ensemble des données, l'ensemble des nécessités relatifs différentes lignes de métro du Grand Paris Express sont actuellement prises en compte, le gouvernement a décidé d'agir avec méthode, avec énormément de concertation des élus locaux en 1er lieu des utilisateurs également et comme le vous le savez, la ministre des transports est en phase finale avec le 1er ministre de consultation pour pouvoir élaborer cette carte des projets de métro du Grand Paris Express très, très rapidement, donc je j'entends totalement votre point le gouvernement agit avec méthode sur ce sujet, mais tient évidemment bien en compte des points que vous avez soulevé monsieur le sénateur. Merci monsieur le ministre, monsieur cap au Canada pour explication de vote. Oui merci monsieur le président, Monsieur le ministre, vous avez élargi la réponse très utilement l'ensemble des questions de transport qui sont liées aux Jeux olympiques, non seulement CDG Express, mais aussi les lignes qui sont, sur ce de Gex pas, je ne suis pas favorable à l'amendement qui vous avons qui sont défendues là parce que je pense, effectivement comme l'a très bien dit notre rapporteur, qu'il faut maintenant aller au bout de cette procédure, il est normal que Paris et Tunis directe avec l'aéroport majeur, c'est un sujet de compétitivité internationale et on mettrait en défaut, la grande compagnie qu'est Air France et le secteur aéroportuaire et le secteur aéronautique français si on n'avait pas au bout de cette opération, je veux également dire que c'est une vision directe et donc il faut à côté du la liaison directe de Paris à CDG, une liaison qui elle va s'arrêter dans les différentes gares et qui permettra au territoire voisin de mieux se rendra à Charles-de-Gaulle, ensuite je partage pas le pessimisme Monsieur Laurent on peut avoir des doutes sur le financement, mais il faut quand même éviter peut-être de dire que toutes les études évoquent un déficit d'exploitation, je crois qu'il a de solides quand même qui sont à l'appui des décisions qui ont été prises par aéroports de Paris, SNCF, réseau pour justifier leur engagement, alors maintenant Monsieur mis sur les questions de de gare on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, le 1er ministre nous a réuni pendant 3 heures et demie dans un très bon climat de compréhension mutuelle, il y a une dizaine de jours et j'ai eu l'occasion d'interpeller et d'indiquer que, s'agissant des Jeux olympiques, il fallait sécuriser maintenant très vite, l'ensemble des gares qui étaient liés à ces Jeux olympiques, le prix sera bien voulu me répond que c'est une préoccupation qui partagé pour les gares voilà, hé bien, nous avons reçu la semaine dernière et l'aide de Madame étaient des transports qui nous a dit que la gare Le Bourget RER étaient dans l'objectif du gouvernement, il faut que, rapidement, le gouvernement disent que la 2ème gare qui est à côté de la gare, dites-le Bourget, aéroport, qui doit permettre à des serres du centre de presse doit faire l'objet de la même attention à ne pas afficher une intention et ne pas afficher un objectif, c'est prendre un risque qui est totalement incompréhensible que le gouvernement choisisse parmi les gares olympique celle si oui cela je suis pas encore certain donc l'affiche, pas du tout d'objectif, c'est la meilleure façon de déstabiliser l'édifice et de faire que je processus technique et compliqué, n'arrive pas à son terme, enfin j'en termine en disant que la décision date du 13 septembre et qu'il est grand temps que le gouvernement mette un avenant tous les moyens au bout de 4 mois, il est temps de 6 mètres pour que cette échéance-là soit bien assurée, merci. Merci, cher collègue madame de La Gontrie pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, on touche un point sensible, il faut pas qu'il y a de de malentendus, de confusion dans les positions des uns et des autres, Pierre Laurent a raison de dire que il y a une grande inquiétude face à la possibilité de financement, du réseau Grand Paris Express dire soulevée par le gouvernement lui-même lorsque a commencé à être exprimée le fait qu'il n'était pas possible de réaliser l'ensemble du réseau dont j'indique qu'il a été lancé à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'est dire que, à la fois le temps a passé et qu'en même temps les volontés politiques diverses, ce sont, s'exprimer sur ce point, sur la question du Charles-de-Gaulle Express, nous avons toujours su, lorsque nous sommes en tout cas francilien qu'il y avait une concurrence possible entre le RER qui avait grand besoin évidemment d'être rénové à cet endroit-là et des lignes qui devait être développé et ce fameux Charles-de-Gaulle Express qui coûte extrêmement cher et qui d'ailleurs ne trouvait pas de financement a été trouvé l'idée du financement privé ou du financement par la taxe sur les billets d'avion, fort bien, mais effectivement cette inquiétude aller réel, il faut effectivement que ce projet se réalise, tant mieux si les financements sont différents des financements publics et donc nous sommes pour notre part, défavorable à l'amendement de suppression, mais il faut bien sûr que le gouvernement entende que ça ne peut pas être déshabiller Pierre pour habiller Paul et et en clair faire financer par des fonds publics, ce n'est pas prévue aujourd'hui le Charles-de-Gaulle Express au détriment du Grand Paris Express mais pour autant, reste toujours cette inquiétude premières qui est que l'on ne peut pas se contenter d'un développement du réseau Grand Paris Express à la perspective des JO et uniquement perspective des JO et je ne parlerai pas des autres lignes qui ne sont, j'ai envie dire malheureusement pour elle, pas concernés par les JO aujourd'hui et donc d'accord sur le fond avec Pierre Laurent, mais pas sur le porte-unité de cet amendement, nous ne voterons pas et encore une fois, le gouvernement, j'indique à monsieur le ministre, que la concertation avec les yeux, il ne faut quand même pas se payer de mots, je veux dire que convoquer les élus dans une réunion sympathique pendant 3 heures pour un 1er ministre qui nous dit que de toute façon il nous annoncera rien c'est un peu le scénario Notre-Dame-des-Landes répétita enfin ne prétendons pas que les, les, les élus ont été conservés concertée en revanche à l'aide de Madame Borne était plus intéressante, même si elle préfigure le fait que sans doute certains territoires d'Île-de-France vont devoir attendre plus longtemps que prévu l'arrivée du Grand Paris Express.

nous ne sommes pas. Convaincu et rassuré parce que il y a dans cette affaire, qu'on le veuille ou non un traitement à 2 vitesses, parce que la ligne du Charles-de-Gaulle Express, elle a trouvé son financement très rapidement, visiblement, j'entends le rapporteur il y a pas de problème de calendrier, elle a trouvé son financement pour le construire, mais le problème de l'équilibre de l'exploitation de cette ligne n'est absolument pas réglé tout le boulot c'est et il y aura des problèmes à venir, et là on se tournera à nouveau vers les fonds publics quand il faudra traiter la question de l'équilibre de la ligne, il faut quand même qu'on est en en tête les hordes de grandeur parce qu'on parle de compléter, c'est une ligne qui va transporter quelques petites dizaines de milliers de voyageurs jour quand je leur ai RER B en transporte très mal aujourd'hui 800000 par jour et je ne parle pas des lignes qu'on est en train de construire dans le Grand Paris Express donc en terme de priorité, il y a quand même beaucoup peu on nous dit ça va compléter le dispositif, il faut rien opposer, sauf que pour le moment, je le répète, il y a une ligne, c'est-à-dire celle qui va qui ne va pas servir aux gens qui habitent la région parisienne qui, elle, est déjà sécuriser, on l'entend, elle va être réalisé très rapidement et sur le Grand Paris Express, on a encore beaucoup de questions et beaucoup de questions sur la sécurisation du financement du calendrier de la réalisation et je voudrais terminer en disant une chose imaginez la situation si au moment où se déroulent les Jeux olympiques et où on parle de célébrations populaires la ligne Charles-de-Gaulle Express donc laquelle aucun en

quand on démarre les Jeux cette ligne fonctionne et qu'on n'a pas réalisé l'intégralité du Grand Paris Express en améliorant les transports du quotidien d'Île-de-France pour la célébration populaire des jeux,

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté sur l'article 13 bis B. Donc, sur l'amendement 12 il a été présenté en même temps je pense que ces mêmes avis de la commission du gouvernement défavorable, c'est même vote. Même vote, donc il n'est pas adopté et sur l'article 13 bis B, c'est le même vote que pour l'article 13 bis, il est adopté. Sur l'article 13 blessés monsieur savants.

mais il y a aussi un impact qui qui qui peut être très négatif sur l'organisation des Jeux si le grand si les travaux sur le Grand Paris Express ne sont pas réalisés, c'est que les organisateurs de France. Trouver une solution alternative qui va coûter beaucoup plus cher dans l'organisation des Olympiques et après il faudra pas qu'on se plaigne que le coût des Jeux olympiques dépasse le coût qui a été annoncé au démarrage les infrastructures ne sont pas réalisées, donc il y a aussi, donc j'appelle aussi le gouvernement a à respecter les engagements qui ont été prises, notamment au au moment du dépôt de la candidature, comment peut-on être crédible par la suite lorsqu'on moment au dépôt des candidatures, on annonce des grands principes, sur les grands travaux pour réaliser ces Jeux olympiques, et que cette ambiance comment déjà à se poser la question serait en capacité de les réaliser en termes financiers, en termes de délais de travaux, donc moi j'appelle le gouvernement pour que ces travaux puissent être réalisés bien sûr par rapport aux arguments qui ont été évoqués tout à l'heure, mais surtout parce que c'est le ce qui nous concerne aujourd'hui sur l'Olympique pour la bonne réalisation à la bonne organisation de ces Jeux, merci. Merci, cher collègue, donc je voilà recycle 13. Qui est pour.

à l'opposition d'abstention, c'est adopter sur l'article 15, donc sur l'éthique et l'intégrité monsieur savants. Rapidement aussi, Monsieur le Président, vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré les pouvoirs disciplinaires de la F. non conforme avec la constitution et le gouvernement d'Ankara jusqu'à 7 ans pour se mettre en règle, ce qui doit permettre, avec cet article cependant une réflexion à mes yeux de et à nos yeux, doit être beaucoup plus large, elle devrait être lancée concernant l'AFLD alors que son laboratoire a été suspendu ces derniers mois que le rapprochement avec l'Institut de sciences du vivant de Saclay est en discussion avec un projet notamment important de relocalisation est en cours parce qu'aujourd'hui, cette agence contre pages et dans des locaux qui sont quasiment insalubre, donc il y a urgence, de répondre à une attente forte de ce qui est aujourd'hui ce qu'qui faisait encore encore la fierté de notre pays au niveau de, de la lutte conte le dopage.

du gouvernement au Parlement sur les moyens financiers de l'Agence de lutte contre le dopage et va évaluant notamment l'opportunité de conférer une partie des droits télévisuels des Jeux olympiques et paralympiques l'à l'agence Damon Mandement entend ainsi engager une réflexion sur les moyens nécessaires à la lutte contre le dopage. Oui le le sujet effectivement des moyens de l'AFLD est important, ce qui a été rappelé par mes 2 collègues indépendamment de je dirais la la réserve très naturel de la Commission sur les rapports, j'indiquerai que la subvention pour charges de service public de l'AFLD a été augmenté de 13 pourcent déjà par rapport à 2017 9 millions 6 d'euros outre ses ressources propres, à hauteur d'un 1000000 5, j'indiquerai également la question des droits télévisuels des jeux relève du comité international olympique qui contribue en contrepartie au financement des Jeux à hauteur de 1,2 milliard et Janica enfin de la discussion sur les ressources de l'AFLD relève du projet de loi de finances et plus précisément la mission Sport, jeunesse et vie associative pour toutes ces raisons, c'est une demande de retrait, à défaut, un avis défavorable. Madame la sénatrice AFLD est aussi une priorité pour le ministère des Sports l'affectation d'une partie des droits télévisuels des jeux à l'AFLD serait ponctuel et et ne permettrait pas de pérenniser ces ressources au-delà de jeu, ce qui est contraire à l'objectif que nous que nous poursuivons, c'est pourquoi il est nécessaire de renforcer les moyens de l'agence dès aujourd'hui l'héritage des Jeux, c'est aussi préparer l'avenir de l'AFLD en stabilisant sa subvention, et en l'accompagnant dans sa stratégie pour le futur et c'est ce que nous avons fait dans le cadre du PLF 2000 2018, avec une augmentation de 10 pourcent de son budget, cela nous permet de rappeler combien la lutte contre le dopage est une priorité pour notre pays, afin de garantir aussi la crédibilité des compétitions et de préserver la santé des sportifs au regard c'est élément votre proposition de rapports ne me paraît pas pertinente, je vous suggère donc de retirer votre amendement. Merci madame l'homme. Oui je je le retire, merci de nous avoir précisé que vous, vous veillez à pérenniser les les moyens nécessaires.

après article 16 l'abondement 25 Monsieur Lozach. Oui Monsieur Président cet amendement concerne la lutte contre les les manipulations sportives et je dirais la lutte pour l'équité sportive en effet Honda profité en quelque sorte de ce texte, qu'on appelle la loi olympique, pour essayer d'aller plus loin en matière d'efficacité dans la lutte anti-dopage et je crois que ce serait dommage de ne pas adopter une position identique en ce qui concerne la lutte contre la corruption sportive. Si la plupart des manipulateurs de compétitions sportives promettent à des arbitres, des joueurs ou des entraîneurs, des sommes importantes pour qu'ils acceptent de manipuler les résultats du jeu de récents cadeaux montrent que le Crime organisé, mais il est désormais plus a menacé un joueur ou sa famille dans le but de le forcer à manipuler sa compétition afin de protéger les Jeux olympiques de Paris 2024, il est nécessaire de punir ces menaces plus fortement que les. Cette corruption, donc je dirais cette année de mandat mais un amendement pardon de bon sens en ce qui concerne la la hiérarchisation des peines parce que, effectivement, on assiste à un développement des des paris en ligne et donc à un développement des actes répréhensibles en la matière, je voudrais simplement donner un chiffre qui montre que les masses financières en jeu sont absolument considérables, il faut savoir que le chiffre d'affaires concernant les mises pour les paris en ligne qui sont pas simplement des paris sportifs, certes, cela représente plus de 400 milliards d'euros par an et d'ébène évident qu'il y aura une accélération de tous ses paris à l'approche et notamment pendant les Jeux olympiques de 2024 donc, le but c'est véritablement d'aller vers une sorte d'éradication de ce risque d'atteinte à la sérénité des épreuves à la sincérité des compétitions. Si chers collègues Madame la rapporteur. Il existe déjà dans le code pénal des accréditations suffisantes pour faire face à ces faits, qui prévoit des peines tout à fait suffisante également, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre. Monsieur le sénateur, je suis aussi défavorable à cet amendement pour 3 raisons : la première, plusieurs incriminations générales du code pénal permet déjà de réprimer ce titre Madame la rapporteure la vie ce type de comportement, c'est le cas pour le délit d'extorsion, les délits de menaces avec l'ordre de rendre il y a une condition des délits de violence 2ème point pour les crimes et délits et contraventions existant au sein du code pénal, les peines varient en fonction de la gravité du préjudice, ce qui ne serait pas le cas avec votre proposition et 3ème raison la preuve de ce délit serait délicate, a rapporté, puisque le ministère public devra démontrer le mobile précis des violences et des menaces exercées sur un sportif ou un arbitre à savoir pour modifier le cours normal d'une compétition, donc ce sera un avis défavorable. Merci madame ministre donc je mais au roi, l'amendement est maintenu, l'amendement 25 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Oui, Monsieur le Président, cet amendement vise à consacrer au niveau législatif, l'existence de la plateforme de lutte contre la manipulation de compétition sportive, c'est la même thématique afin de légitimer la transmission d'informations ou de documents couverts par le secret professionnel, en effet, conformément à l'article 226 14 du code pénal, l'atteinte au secret professionnel n'est pas caractérisée dans les cas où la loi impose. Autorise la révélation du secret dont l'objectif est, là aussi, c'est donc d'être plus efficace dans cette lutte contre la corruption sportive et d'appliquer en particulier de méthodes qui concerne la lutte contre le dopage, c'est-à-dire le décloisonnement des services. C'est-à-dire une meilleure circulation de l'information entre les différentes agences et différentes structures qui sont concernés, créée il y a 2 ans, et présidé par Madame la Ministre des Sports la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives regroupe le service central des courses et jeux, la police nationale, le parquet national financier Tracfin, le ministère des Sports le nous SF, l'Arjel et la Française des Jeux, cette plateforme s'inscrit dans un réseau international qui rassemble autour des 25 plateformes en novembre dernier, la Fédération slovaque de football qui était mandaté par l'UEFA pour faire un rapport sur la lutte contre la manipulation des compétitions indiqué, je cite, que la plateforme française est aujourd'hui la plateforme nationale la plus inspirante notre plateforme nationale fonctionne bien, donc, et surtout elle ne coûte pas un Euro supplémentaire à l'État, tous les moyens, aussi bien humains que techniques sont mutualisés entre ses membres pour gagner en efficacité et aujourd'hui les membres de la plateforme nous disent qu'ils ont besoin pour consolider leurs enquêtes de transmettre des informations pouvant relever du secret professionnel, la chancellerie a fait savoir qu'ils avaient peur que ce secret professionnel puisse inclure le secret de l'enquête pénale pour les rassurer, j'ai rapporté une rectification pour préciser que les communications se font sous réserve des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, cette crainte levée, je pense que nous sommes tous accord ici forcer la lutte contre la manipulation des compétitions et permettent à nos enquêteurs de bien travailler. Merci, cher collègue Madame la la rapporteure. Ainsi qu'il a été précisé cette plateforme existe, elle existe sur une base conventionnelle, et elle fonctionne ainsi, pourquoi la consacrer dans la loi, ça ne paraît pas utile de surcroît, les autorités publiques qui la composent, évidemment c'est change assez naturellement des informations quand aux personnes morales doit privé qui la composent, elle n'ont pas nécessairement avoir connaissance d'informations confidentielles, c'est donc un avis défavorable. Merci madame la ministre. Oui monsieur Lozach si je partage votre objectif je suis toutefois défavorable à votre amendement effectivement la plateforme nationale de lutte contre les manipulations de compétitions sportives existe sous statut conventionnel depuis le 28 juin et fonctionne depuis sans qu'il a besoin d'une disposition législative, donc je suis

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adoptée. Nous passons à l'article 17 l'amendement 43 Monsieur Le le président, le rapporteur de la commission des lois a souhaité encadrer le dispositif de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique prévus pour tous les grands événements sportifs internationaux en le limitant aux délégataire des représentants légaux des organismes organisateur engageant Asada niveau de dépenses fixé par décret, cet encadrement est tout à fait compatible avec le fait de circonscrire les déclarations à la Haute autorité au seul délégataire directe de ses représentants, le présent amendement vise donc à circonscrire le niveau de délégations aux seules délégations Direct afin que l'obligation déclarative ne concerne pas des fonctions exempte de tout risque de conflit d'intérêts ou de corruption et préserve le bon fonctionnement de l'autorité administrative indépendante. Merci, cher collègue Madame le rapporteur. la proposition qui est faite, et qui vise la délégation Direct laissant réalité un certain flou juridique planer car on ne sait pas où arrête la délégation directe et où commence la sub-délégation ce qui va pas rendent très efficace, cette disposition et je rappelle qu'en cas d'erreur, c'est-à-dire dans la mesure où une personne ne respecte pas ces hommes à ses obligations, elle est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, il faut donc prendre des dispositions qui soient d'une grande clarté, c'est pourquoi il s'agit d'une demande de retrait ou, à défaut d'un avis défavorable. Merci mamie. Effectivement, vous proposez de circonscrire le niveau de délégations aux seules délégations Direct mais la ni l'alinéa 6 prévoit déjà de limiter ses obligations responsables des comités d'organisation d'événements sportifs qui disposent d'une latitude importante dans l'engagement des crédits, en effet, les travaux des commissions des lois et des affaires culturelles ont permis de définir un seuil minimal d'engagement des dépenses qui sera fixé par un décret cette solution me semble tout à fait pertinente et satisfaisante compte tenu de ces éléments, il n'a pas nécessaire de restreindre davantage l'obligation de déclaration parce que votre proposition ne permettrait pas de contrôler certaines personnes qui présentent des risques de conflit d'intérêts ou d'enrichissement personnel, donc je préfère que nous préservions la rédaction de la commission et je vous demande de retirer votre amendement. Merci, il est maintenant pour retirer maintenant il est maintenu. Donc, l'amendement est maintenu, donc il y a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté l'amendement 55 le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination Monsieur Président. Madame la Ministre. Ali favorable : avis favorable donc je mais au revoir Mandement 55. Qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, je mais au bout, à l'article 17. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. nous devons bien sûr accompagné l'organisation de ces Jeux leur contrôler si besoin, mais pourquoi vouloir assister et prendre part à ces instances, notamment dans le comité des rémunérations, alors même que cette présence ne sera que consultatif, de plus, je rappelle que que je n'ai pas une organisation publique ne son budget est financé à 97 pourcent pour le privé et 3 pourcent par l'État et les collectivités, donc il me semble que nous devons pas mélanger les genres et c'est pourquoi notre groupe soutient la position du rapporteur qui nous sommes tout à fait légitime. Merci l'amendement 28 bis Madame Jourdain. Merci Monsieur le Président, Madame la ministre l'a rappelé la transparence et l'éthique et l'intégrité sont autant d'idées force que l'on retrouve de manière transversale dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et qui trouvent leur traduction législative dans le titre IV, cela vaut pour la lutte contre le dopage et nous souhaitons ardemment que l'Agence française puisse retrouver ses lettres de noblesse à l'occasion des Jeux, cela concerne aussi la lutte contre la corruption, notamment dans le cadre des paris sportifs, cette exigence de transparence concernant enfin les dirigeants du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques le ces ces derniers seront soumis à une obligation de déclaration d'intérêts et de Patrimoine auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, nous le savons, l'encadrement des rémunérations n'est pas possible du fait de la structure associative du COJO Europe même si ce dernier gérera un budget de 3 milliards d'euros à la présence de parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité de rémunération avec voix consultative, la commission des lois, adoptées à l'initiative de la rapporteur, un amendement pour lui substituer la remise d'un rapport annuel aux commissions compétentes des 2 assemblées dans sa nouvelle rédaction l'article 17 bis prévoit que le rapport détaille les 10 principales, rémunération des dirigeants du COJO et les activités de son comité d'éthique, l'objet de notre amendement vise donc à ce que le rapport du qu'au Japon, mentionne également les activités du comité des rémunérations et du comité d'éthique.

du Parlement sur l'activité du COJO en étant plus précis, donc la commission a donné un avis favorable. Merci madame la ministre. Madame la sénatrice, vous c'était quoi. Ce rapport présente également l'activité des 2 autres organes de contrôle du COJO, le comité de rémunération et le comité d'audits votre amendement vise à compléter l'information du Parlement sur ce point, je m'en remets à la sagesse des sénateurs. Merci madame la ministre, donc je mais voire amendement 28 2 bis avec un avis favorable de la Commission invite sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, je mais au mois, l'article 17 bis même vote. Même vote est adoptée après l'article 17 bus amendement 29 Madame Jourdain. Merci monsieur le président, bien que ce projet de loi suscite une forme de consensus sur l'ensemble des bancs de cette assemblée, nous pouvons constater que le Parlement dispose de capacités d'amendements fort limitée tenant aux engagements pris par les gouvernements successifs auprès du CIO, et au terme du contrat de ville hôte de même le Parlement semble en retrait dans le suivi de l'organisation de cet événement majeur, or il n'est pas inutile de rappeler que les précédentes décisions des Jeux d'été comme d'hiver ont systématiquement occasionné d'importantes dérives, notamment financières, si le budget de Paris 2000 24 à Paris, à ce stade, maîtriser des impondérables demeure, je pense notamment aux dépenses de sécurité impossible à évaluer à plus de 6 ans de l'échéance, l'article 17 bis que nous venons d'adopter prévoit déjà la remise d'un rapport annuel du COJO mais qui ne concerne que l'activité des organismes de contrôle instaurées par le comité d'organisation, l'article 18 prévoit quant à lui à son alinéa 2 la remise d'un rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des Jeux en 2022, ce dernier sera établi dans la perspective d'un contrôle des dépenses publiques, or et afin que la preuve représentation nationale soient régulièrement informés de l'état dans Lancement des différents chantiers ou des nouvelles contraintes et afin qu'elle puisse procéder aux contrôles, on continue de l'action du gouvernement, il nous apparaît utile de commander un rapport annuel au délégué ce rapport retrace les différentes opérations concourant à la préparation à l'organisation et au déroulement des Jeux, notamment les vols équipement, sécurité et transport, il pourrait de surcroît servir de support à des auditions régulières du délégué interministériel devant les commissions parlementaires je note cependant pour ne pas ensevelir notre assemblée sous les rapports que celui que nous proposons, pourrait utilement être fusionné avec celui prévu par l'amendement numéro 18 de notre collègue Madame mélo. Merci, cher collègue Madame le rapporteur. ça n'est pas le Dijonnais bien la Solideo qui est responsable de de la livraison des dans les délais des ouvrages olympiques et paralympiques et à ce titre, hé bien elle dispose déjà du litiges juridiques et notamment du pouvoir de se substituer aux éventuels, maître d'ouvrage défaillant, de surcroît, je dirais que l'amendement est en partie satisfaite puisque près de la tête haute finance prévoit déjà la remise d'un jeune budgétaire qui présentera les dépenses publiques engagées pour les Jeux eux-mêmes et, enfin, je rappelle que la Cour des comptes contrôle déjà puisqu'elle rendra un 1er rapport en 2022 sur les constructions, c'est pourquoi il s'agit d'une demande de retrait et à défaut d'un avis défavorable. Merci madame la ministre. L'état d'avancement des opérations concurrents à l'organisation des Jeux fera l'objet : l'objet d'un vigilance toute d'une vigilance toute particulière du gouvernement, je serais donc en mesure de vous rendre compte de l'avancement de leur préparation en tant que de besoin, notamment en répondant à toutes questions écrites ou orales que vous voudrez bien m'adresser, il n'est donc pas nécessaire de mettre à contribution le dit jobs sur ce point, par ailleurs, je rappelle qu'en 2022, la Cour des comptes transmettra au Parlement un rapport relatif à la gestion de l'organisation des Jeux et elle sera habilitée à contrôler le COJO dès la promulgation de cette loi, j'aimais donc un avis défavorable à votre amendement. Merci madame jour. Merci, Madame la Ministre, pour ces précisions je vais retirer cet amendement. Merci donc l'amendement 29 bis retiré, nous passons à l'article 18 de la prise de parole, monsieur. Merci Monsieur le président, s'il est important que le COJO soit contrôlée pour éviter tout dérapage financier une explosion des coûts, il faut cependant ne pas outrepasser les compétences de la Cour des comptes, ni imposer un contrôle trop rigoureuse aux équipes du collège qui n'ont d'ores et déjà fait leurs preuves dans le bon usage de l'argent public, ainsi la remise d'un rapport en 2020, 200 d'être une solution équilibrée qui permettra d'avoir un 1er, retour sur le déroulé de l'organisation et permettra de prévenir tout déséquilibre. Merci, cher collègue donc jamais au voilà recycle 18 qui est pour. Qui est con. Qui s'abstient, il est adopté, même votre peau, article 19. Même votre enquête adopté et après l'article 19 l'amendement 18 bis Madame mélo. Oui merci monsieur le président, instamment demandé commandeur, rapport du gouvernement au Parlement sur l'impact environnementale de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques : il s'agit donc de dresser le bilan des atteintes environnementales en matière de construction des infrastructures de conséquence de la publicité et de reconversion des sites en bref, un bilan à remettre avant la fin de l'année 2025 merci. Merci, cher collègue Madame la rapporteur. Quand même, de rapports vous laisse penser ce que je vais demander pour cet amendement, je rajouterais tout simplement qu'il n'est pas évident que dans ceux-ci bref délai après la fin des Jeux, on puisse assurer la reconversion des sites

le rapport que vous préconisez ne m'apparaît pas opportun, en effet, l'ambition de faire de nos jeux, un événement marqué par une forte dimension environnementale c'est nettement affirmée dès la phase de candidature, le dossier final de candidature remis en février dernier, consacre un chapitre entier à la durabilité et à l'éco-responsabilité une philosophie qui doit embarquer le secteur du sport en général concernant l'impact de la publicité des jeux sur l'environnement, le lien paraît négligeable dans la mesure où la publicité ne sera autorisée que pendant une durée limitée, qu'elle s'effectuera principalement par voie d'affichage elle conviendra néanmoins de solides et sollicitées le COJO et la Solideo qui sont les euh 2 opérateurs qui mettront en 9 nos engagements de candidature dès cette année, donc je suis donc défavorable aussi à cet amendement.

Je n'en vois pas donc Genève l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents et sont donc adopté je vais lever la séance. Lors du jour du mercredi 7 février 2018 à 14 heures 30 et le soir, nomination des 21 membres de la commission d'enquête sur l'organisation des moyens des services de l'État pour faire face à l'évolution de la menace terroriste après la chute de l'État islamique et un projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, la séance est levée.